Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué. S'il n'y a pas d'observation, je n'en vois pas le procès-verbal États d'adopter sur les réserves d'usage.

portant sur le projet de loi de finances 2019 je n'ai pu être présente et n'ai pu donc participer au scrutin, je souhaite, madame la présidente, vous dire que j'aurais voulu voter pour le projet de loi de finances 2019 je vous remercie. J'informe le Sénat que des candidatures pour siéger au sein de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi habilitant le gouvernement à prendre par ordonnances, les mesures de préparation au retrait du Royaume-Uni, de l'Union européenne ont été, qui ces candidatures seront ratifiées si la présidence n'a pas reçu d'opposition dans le délai d'une heure prévu dans notre règlement. L'ordre du jour appelle la discussion de la proposition de loi adoptée par l'Assemblée nationale instituant des funérailles républicaine, c'est une demande du groupe socialiste et républicain dans la discussion générale, la parole est à monsieur Sébastien Lecornu, ministre chargé des collectivités territoriales, je vous en prie, monsieur minutes. Merci madame la présidente, madame la vice-présidente de la commission des lois, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, Monsieur le président de groupe je suis heureux de me retrouver une fois de plus au Sénat aujourd'hui quasiment en ce moment d'ailleurs une fois par jour pour cette proposition de loi visant à instituer des funérailles républicaine qui a été adopté, vous l'avez rappelé en première lecture par l'Assemblée nationale, il y a plus de 2 ans maintenant, sous la précédente législature, elle revient aujourd'hui au Sénat, c'est pour moi l'occasion de saluer la grande qualité des débats et des échanges qui ont lieu, tant à l'Assemblée nationale qu'ici au Sénat lors de son examen en commission des lois, c'est autant plus important de souligner que le sujet qui nous réunit aujourd'hui est complexe car il touche à l'intime aux croyances, il est souvent dit que le degré de civilisation d'une société peut se mesurer à la place qu'elle qu'elle accorde à ces défunts, j'en suis personnellement convaincu et même si la relation à la mort, a considérablement évolué au cours des siècles, nous leur devons respect et dignité, la proposition de loi répond à une préoccupation légitime : celle de permettre à chaque Français de bénéficier de funérailles dans le respect de ses convictions personnelles et parfois des convictions religieuses en France le principe de liberté de choix des funérailles entre obsèques civiles ou religieuses et garanti depuis la loi du 15 novembre 1987, 1887 pardonnez-moi, ce fut un progrès important annonciateur de la grande loi 1905 adopté quelques années plus tard toutefois tout au long du XXe siècle, les pratiques funéraires des Français ont évolué assez fortement une étude publiée en 2016 par le Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie, le Crédoc permet de s'en rendent compte aujourd'hui 74 pourcent des obsèques sont religieuses et 26 si la cérémonie hélas très majoritairement religieux en cas d'inhumation 87 pourcent des cas cela est beaucoup moins le cas pour les crémations 49 pourcent des cérémonies civiles, or nous assistons depuis quelques années une augmentation très forte du nombre de crémations des décès en 1980 à 35 pourcent en 2016, le constat est donc clair : les Français sont de plus en plus nombreux à faire le choix de la crémation et donc à opté pour l'organisation de cérémonie civile, même si ces dernières restent encore aujourd'hui minoritaire, il ne s'agit donc pas de nier cette évolution sociale importante en France comme à l'étranger et de réfléchir à la meilleure manière pour y répondre, je vois, mesdames, messieurs les sénateurs, 2 approches possibles la première constituerait recourir à la loi, c'est l'objet de votre texte qui prévoit de dispositions : d'une part, demander à la commune de mettre à disposition, je cite, gratuitement, une salle adaptables, afin de permettre aux familles d'organiser des funérailles suivent. D'autre part, permettre à un officier d'état civil, s'ils le souhaitent, de procéder à la cérémonie, ces propositions sont parfaitement louables et partent clairement d'une bonne intention, néanmoins elle soulève un certain nombre d'écueils que vous avez à juste titre, rappelé dans vos travaux, monsieur le rapporteur. Les partage grande partie en tout cas, 4 points me paraissent particulièrement importants : tout d'abord, il s'agit d'une contrainte nouvelle imposée aux communes, sans aucune compensation financière et qui serait donc financé par le contribuable local, en effet, les communes devraient prendre à leur charge les coûts d'entretien sans oublier la mobilisation du personnel municipal pour l'aménagement, la surveillance et la remise en état de la salle, alors que les communes réalise déjà des efforts importants dans la maîtrise de leurs dépenses publiques leur imposer une nouvelle contrainte ne nous paraît pas justifié ensuite la mise en oeuvre de cette proposition se heurte à des écueils pratiques susceptibles de générer des contentieux devant le juge administratif qu'est-ce qu'une salle adaptable dans quelles conditions une commune peut estimer ne pas être en mesure de la mettre à disposition, par exemple, en l'absence de définition précise à la ministre mécontent pourrait se tourner vers le juge, en estimant que la mairie avait une salle adaptable, si ces questions paraissent certains secondaire, elles sont susceptibles de créer de l'insécurité juridique pour les élus locaux, troisièmement, cette proposition de loi pose la question de son articulation avec les missions exercées aujourd'hui par les opérateurs funéraires, en effet, depuis la loi du 8 janvier 93 le monopole des communes sur le service extérieur des pompes funèbres a été supprimé, permettre la mise à disposition gratuite de salles conduirait potentiellement un risque potentiel, en tous cas de distorsion de concurrence, ce choix pourrait s'avérer contradictoire avec la démarche d'allégement des procédures et des normes en matière funéraire qui a amené à réduire voire à supprimer la présence d'agents publics dans différentes étapes des obsèques, enfin je ne suis pas certain qu'il soit opportun de conférer de nouvelles attributions à l'officier d'état civil, dont le rôle consiste à délivrer des actes d'état civil et non à présider des cérémonies par ailleurs je cela soulève 2 autres problèmes tout d'abord, contrairement au mariage civil où il est fait lecture précisément les articles du code civil, aucune disposition n'encadre le déroulement d'une cérémonie de funérailles républicaine ensuite si la loi donne et l'officier d'état civil la possibilité de ne pas y participer cette application, pardonnez-moi l'expression, à géométrie variable est de nature à nourrir des procès potentiels en discrimination pour toutes ces raisons-là, et ce malgré le caractère généreux et louable de ce texte, je ne pense pas que le recours à la loi, soit la manière la plus opportune de répondre aux attentes des Françaises et des Français en matière funéraire, nous pouvons aussi opter pour une autre stratégie qui a clairement ma préférence, faire confiance aux élus locaux inciter plutôt que de contraindre, comme vous le savez, j'ai moi-même été maire de Vernon et présidents de conseil d'un appartement à Alger comme vous, la culture de l'élu local, je connais donc aussi bien que vous en tout cas je je l'espère les potentialités et les intelligences locale et les pentes et notre de nos territoires, au lieu de les contraindre une fois de plus, je préfère leur faire confiance, alors que j'ai annoncé vouloir lutter contre les irritants notamment générées par la loi, autres qui comprendrait que je défende aujourd'hui l'adoption de nouvelles contraintes pour les communes, le droit actuel n'interdit d'ailleurs pas l'organisation de funérailles civiles comme l'a rappelé notamment l'Association des maires de France et l'association des maires ruraux de France en effet nombre de communes mettent d'ores et déjà des salles à disposition sans que cela ne semblent soulever la moindre difficulté particulière, il arrive aussi que des élus interviennent pour y prononcer une allocution enfin la NRF, l'a rappelé, devant vous, monsieur le rapporteur, les usages locaux sont très importants en matière d'obsèques en métropole, mais aussi en outre-mer et il faut plutôt s'en remettre une fois de plus encore à l'Intelligence territoriale certaines communes mettent à disposition des salles d'autres remette des documents aux familles des défunts pour les accompagner dans les procédures administratives : bref, faisons confiance aux élus, je ne le répéterai jamais assez, car ce sont eux qui connaissent le mieux les besoins de leur administrer l'absence de problèmes particuliers, l'existence d'un cadre juridique permettant de régler nombre de situations, notre volonté de ne pas créer une nouvelle norme et notre confiance inébranlable dans les territoires sont autant de raisons pour lesquelles le gouvernement est défavorable à l'adoption de cette proposition de loi pas pour ses intentions mais de messieurs les sénateurs, qui sont juste honorable et louable, mais pour la méthode retenue, je vous remercie. Merci monsieur le ministre, la parole est à monsieur Loïc Hervé rap. Porteur de la commission des lois pour 10 minutes. Madame la présidente, madame la vice-président de la commission des lois, monsieur le Ministre, chers collègues. La proposition de loi visant à instituer des funérailles républicaine que nous examinons aujourd'hui a été adopté par l'Assemblée nationale le 30 novembre 2016 sous la précédente législature. Elle était présentée par notre ancien collègue député Bruno Le Roux et plusieurs de ses collègues de l'Assemblée nationale la semaine dernière la commission des lois du Sénat l'a rejetée en adoptant un amendement de suppression de son article unique présenté par notre collègue Jean-Pierre Grand. En conséquence. Et en application du premier alinéa de l'article 42 de la Constitution notre discussion porte aujourd'hui sur le texte de la proposition de loi telle qu'adoptée à l'Assemblée nationale pour préparer nos travaux, j'ai tenu en autant dans les différentes parties prenantes, les associations d'élus. La fédération des Familles de France. Les opérateurs funéraires publics ou privés, les représentants des cultes. La Fédération nationale de la libre pensée, ainsi que les administrations concernées. La justice ou votre ministère, Monsieur le Ministre. Je me suis évidemment entretenu avec le 2ème, signataire de la proposition de loi Monsieur Hervé Féron, qui était aussi rapporteur au nom de la commission des lois de l'Assemblée nationale. Je remercie notre collègue Jean-Luc Fichet, d'avoir participé aux auditions et au président, Jean-Pierre Sueur, avec qui nous avons pu échanger. Le principe de liberté de choix des funérailles entre obsèques civiles ou religieuses et garanti depuis le XIXe siècle et la loi du 15 novembre 1887 sur la liberté des funérailles. Si les premières tendent à se développer, notamment avec le recours croissant à la crémation plutôt qu'à l'inhumation, les secondes reste encore largement majoritaire en France, elle représente encore 74 pourcent des obsèques, selon une étude du Crédoc en 2016. Les règles actuelles de la domanial étaient publiques permettent d'ores et déjà, l'organisation d'obsèques civiles au sein de bâtiments communaux, l'attribution d'une salle municipale relève toutefois de la seule appréciation de la commune est soumis à une redevance sauf exception. Il arrive également que l'officier de l'état civil s'implique lors de la célébration des obsèques, mais à titre privé et avec l'accord de la peur personne ayant qualité pour pouvoir aux funérailles, je l'ai moi-même fait alors que j'étais maire, la proposition de loi adoptée par l'Assemblée nationale a 2 finalités premièrement. Elle tend à imposer aux communes qui disposent d'une salle adaptable, de garantir l'organisation de funérailles républicaine en la mettant à disposition des familles des défunts. Deuxièmement, elle vise à donner à l'officier de l'état civil, la faculté de procéder à une cérémonie obsèques civiles dans l'hypothèse où la famille le demanderaient. Elles sortent, elle se heurte toutefois de nombreux écueils, vous l'avez évoqué, monsieur le Ministre, que je vais moi aussi tenter de résumer promet recueille l'absence de mention expresse de la notion de disponibilité de la salle, qui pourrait donc conduire à interpréter des dispositions comme accordant une priorité à la demande de réservation de salle pour définir républicaine et générer alors des conflits d'usage. 2ème écueil, l'absence de définition du caractère adaptable de la salle qui ne manquerait pas de susciter des contentieux devant le juge administratif 3ème écueil, l'absence de mention des cas dans lesquels la commune pourrait légitimement refuser la demande de mise à disposition 4ème accueille l'ambivalence de la notion de funérailles républicaine plusieurs représentants des cultes, on fait remarquer qu'une cérémonie d'obsèques religieuses. N'était pas moins républicaine qu'une cérémonie strictement civil, de fait, en vertu du principe constitutionnel d'égalité devant la loi, la commune pourrait-elle légitimement refusé la demande d'une famille souhaitant utiliser une salle pour l'organisation d'obsèques religieuses. La question se pose d'autant plus que certains opérateurs funéraires m'ont indiqué que cela se faisait déjà. 5ème écueil le coût induit pour les communes qui devrait mettre à disposition aménager et entretenir gratuitement sans compensation financière, une salle adaptable, alors même que les dispositions de la proposition de loi aurait une incidence marginale sur le coût global des obsèques, celle-ci nécessiterait en effet toujours l'intervention d'opérateurs funéraires habilitée à assurer le service extérieur des pompes funèbres. 6ème accueille le caractère singulier de la nouvelle compétence confiée aux officiers d'état civil qui ne relèverait pas du chant traditionnel de leur mission en principe toujours en lien avec l'établissement, la publicité d'un acte de l'état civil qui génère alors les droits et les obligations. Au demeurant, préparé. Et présidé une cérémonie funéraire ne s'improvise pas, à cet égard les dispositions de la proposition de loi pourrait introduire une distorsion avec les agents des régies, associations ou entreprises de pompes funèbres obligé d'être diplômé pour exercer leur profession de maître de cérémonie et les officiers de l'état civil qui pourrait conduire une cérémonie d'obsèques sans diplôme ni habilitation en la matière, par ailleurs, il est impossible, il est possible, pardon, de s'interroger sur la latitude laissée aux élus de refuser de procéder à une cérémonie civile l'éventuel refus l'officier d'état civil pourrait être interprété comme une rupture d'égalité, voire une discrimination et faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire alors que le contentieux, la mise à disposition de la salle relèverait lui du contentieux administratif. Mais chers, collègue, je partage l'objectif recherché par les auteurs de la proposition de loi de prendre en considération le développement des obsèques civiles dans notre pays et je suis bien entendu favorable à ce que les communes lorsqu'elles le peuvent mettre à disposition des familles, une salle à cet effet. Elles le font déjà et d'ailleurs sans difficulté particulière, comme l'fermement souligné les associations d'élus, notamment l'Association des maires de France et des présidents d'intercommunalités, il n'est donc ni nécessaire ni utile de créer une nouvelle obligation à la charge des communes sans compensation financière ni même de rappeler une faculté qui existent déjà, comme le proposent certains amendements le Sénat attache la plus grande importance à la qualité de la loi et à son caractère normatif et s'effondre finalement aussi la fonction de la commission des lois, dans cette maison pour l'ensemble de sa raison, mes chers collègues, la commission des lois vous invite à rejeter la proposition de loi est adopté les amendements de suppression de son article unique déposée par nos collègues Jean-Pierre Grand et Alain Marc, je vous remercie.

présidente, monsieur le ministre, monsieur le président de la commission des lois, monsieur le rapporteur du chers collègues, la proposition de loi instituant des funérailles républicaine que nous examinons aujourd'hui a pour objet de faciliter l'organisation d'obsèques civiles au sein de salles municipales Alcan tout d'abord à imposer aux communes qui disposent d'une salle adaptable, de garantir l'organisation de funérailles républicaine en la mettant à la disposition des familles, elle vise ensuite à donner à l'officier d'état civil, la faculté de proposer à cette cérémonie d'obsèques civiles dans l'hypothèse où la famille le demande toutefois cette proposition de loi semble dénuée de pragmatisme, déjà en 2016 j'étais alors débuter, j'avais fait évoluer le texte initial à la faveur d'un amendement adopté en séance publique, en remplaçant l'expression adapté de de la salle municipale par Leterme adaptables, afin d'essayer d'apporter un peu de souplesse à l'organisation conférer aux communes, notamment celles de petite taille, donc n'avait pas été tenu compte dans la modestie des moyens, faut-il rappeler que dans certaines mairies, le maire lui-même ne dispose même pas d'un bureau occupant celui du secrétaire de mairie je relève en outre que le caractère gratuit, la mise à disposition de salles contrevient aux règles de la daube annualité publique en effet l'occupation luxation du domaine public donné lieu au paiement d'une redevance, même minime, enfin, nous avons tous au sein de cet hémicycle que les mères ont suffisamment de travail responsabilité surtout dans les communes modestes où il s'implique dans de nombreuses tâches qui ne peuvent, faute de personnel ne leur imposons donc pas une nouvelle charge, laissons-les s'occuper uniquement de leurs missions traditionnelles, monsieur le Ministre, mes chers collègues, il paraît inopportun de légiférer sur ce sujet, dans la mesure où le droit en vigueur permet déjà à l'organisation d'obsèques civiles en mairie sans pour autant contraindre les communes au risque de porter atteinte à leur libre administration. Il apparaît également inapproprié de créer de nouvelles obligations à la charge des communes sans compensation financière pour toutes ces raisons, le groupe les indépendants ne votera pas en faveur de cette proposition de loi. Merci, la parole est à Madame Patricia et Richaud pour 7 minutes. Madame la présidente, monsieur le ministre, monsieur rapporteur, mes chers collègues, nous sommes réunis aujourd'hui pour examiner la proposition de loi votée à l'Assemblée nationale le 30 novembre 2016 et instituant des funérailles républicaine. S'il est vrai qu'il y a bien un domaine qui ne souffre pas de sur-transposition de normes et d'abondance de règles, c'est bien celui de la liberté des funérailles. En effet, les règles qui s'appliquent dans ce domaine sont celles de la loi du 15 novembre 1897 et plus particulièrement celles liées à l'article 3 qui stipule que tout majeurs ou mineurs immense en état de tester peut régler les conditions de ces funérailles, notamment en ce qui concerne le caractère civil ou religieux à leur donner et le mode de sa sépulture. C'est seulement en cas de contestation sur les conditions des funérailles et après décision de la juridiction compétente que la décision serait notifié au maire qui serait dans ce cas, chargée d'en assurer l'exécution. à travers la proposition de loi instituant des funérailles républicaine nos collègues députés proposent donc que les maires et les collectivités locales soient intégrés automatiquement dans le dispositif législatif en vue de faciliter l'organisation d'obsèques civiles au sein des salles municipales, mes chers collègues, à ce jour en France 30 pourcent des obsèques civiles sont civils et c'est le service extérieur dépend funèbre qui a une mission de service public, conformément à l'article L. 2223 19 du Code général des collectivités territoriales qui lui confère l'organisation des obsèques en ajoutant un article au code général des collectivités territoriales, comme le propose cette proposition de loi, ce sont donc de nouvelles responsabilités pour les mères de nouvelles charges financières pour les collectivités. Pour avoir été mères de la serre une commune des Hautes-Alpes, je peux témoigner que le maire en particulier et les élus municipaux en général participe si nécessaire à l'organisation des obsèques en fonction des circonstances et des besoins sans que le législateur n'ait eu besoin d'en préciser les modalités. Les élus locaux qui sont présents quotidiennement dans leur territoire savent répondre avec humanité à la détresse des familles et mettre en place les moyens matériels en cas de nécessité. C'est aussi pour ça que nous sommes élus. Pour créer du lien avec les citoyens pour s'adapter aux besoins ponctuels pour faire preuve de discernement, c'est pourquoi je me range à l'avis de nos collègues de la commission des lois, dont je salue le travail et la rigueur confiée aux officiers de l'état civil de nouvelles compétences qui ne relève pas de leurs attributions traditionnelles n'est pas sans conséquences un nouveau cadre juridique serait par conséquent nécessaire puisque nous sortirions du Champ de l'établissement ou de la publicité, de simples actes d'état civil. Chers collègues, vous le savez, 49 pour 100 des maires s'interrogeait récemment déclare qu'ils ne se représenteront pas en 2020, je ne pense pas que ce soit en instaurant de nouvelles obligations en matière d'obsèques civiles que nous allons susciter de nouvelles vocations d'élu local et provoqué un engouement pour un engagement citoyen. Vous l'aurez compris dans la mesure où le la législation en vigueur permet déjà l'organisation d'obsèques civiles au sein de bâtiments communaux, comme les communes l'autorise, lorsque les communes

Madame la présidente, monsieur le Ministre, mes chers collègues. Nous sommes simplement confronté à un sujet de principe qui est au fond qu'elle est dans l'effectivité du déroulement célébration funèbre la conséquence du principe de liberté de choix consacré en effet par la loi de 1887 qui fait partie, au fond de ce cortège de loi postérieure à la consolidation en 1879 de la République avec la loi sur les communes, la loi sur les syndicats, la loi sur le divorce, on pourrait poursuivre la liste. Et donc, puisque cette liberté de choix existe et je préfère ne pas évoquer le pourcentage. Car quelle que fût la proportion. la proportion. Testant qui choisissent la les obsèques civiles il faudrait me semble-t-il s'intéresser à l'exercice concret de de ce droit qui leur revient. Et donc, à la différence des orateur précédent, y compris le ministre, je ne considère pas comme nouvelle la mention dans la loi qui, de toute façon, comporte un très grand nombre d'articles facultatif relatif la à l'organisation des funérailles dans le code des collectivités territoriales, je ne considère pas comme vaine la mention du choix pour les communes de pouvoir accueillir dans une salle municipale, une partie, celle qui est destinée au public le plus large d'une célébration funéraire. C'est ce qui me conduit. à souhaiter qu'un texte soit adopté et a proposé un texte assez substantiellement différent de celui de nos collègues du groupe socialiste. Parce qu'en effet il ne me paraît pas adaptée l'enfer une obligation générale pour toutes les communes, alors que certaines ne dispose pas de la capacité locale d'offrir cet cet espace de rencontre, il ne me paraît pas non plus judicieux de fixer le principe de la gratuité alors que pardon, mais si tout le reste du déroulement d'une célébration funéraire était gratuit, nous nous en serions aperçu depuis quelques temps.

Sous l'effet d'ailleurs d'une concession municipale, elle va payer l'usage de la salle pour la partie de célébration publiques, donc il ne me paraît pas nécessaire pour la le respect du principe de liberté dénoncer dans ce cas-là, le principe de gratuité et donc dans la formule que j'ai proposé au cas où le Sénat voudrait bien dans sa majorité, aborder le sujet. Il me paraît logique que lorsque la commune dispose d'une salle destinée à l'accueil du public, ce qui est le cas d'un assez grand nombre, on applique à ce cas-là, d'utilisation de la salle les mêmes conditions tarifaires que pour n'importe quel autre réunion de public, comme par exemple une activité associative. Troisièmement, je ne crois pas nécessaire ni même véritablement justifiables l'entrée en scène, si j'ose dire, de l'officier de l'état civil, l'officier de l'état civil et détenteur de droits et d'obligations qui tiennent aux règles de l'état civil. Lesquelles font mention. De la naissance. Du mariage et de la confiance, la confection de l'acte de décès. Donc, chaque fois, il nous l'avons tous souhaité ou à peu près chaque fois que l'officier de l'état civil, intervient, il a pu, il intervient pour appliquer des obligations légales évidemment l'accueil d'une célébration familiale ou amicale n'a pas le caractère d'une obligation légale et ne requiert pas l'intervention de l'officier d'état civil qui aurait, dit-on, pas le texte appliquer donc il me semble également que cette mention non, non, véritablement justifiées et enfin la proposition de loi comporte une mention que je comprends tout à fait puisque, dans la logique du droit funéraire mais qui est que le service proposé par la commune, offert par la commune ne soit destiné qu'aux habitants de la commune. Ce qui le droit commun en matière funéraire mais comme précisément les dans la cas cas la prestation de service qui pourraient être donnés par la commune, c'est-à-dire la mise à disposition d'une salle étaient possibles pour certaines communes et pas pour d'autres, il ne me paraît pas très cohérent. D'empêcher, par exemple, une commune un peu plus peuplé et doté de moyens dans une, dans un espace rural de proposer d'accueillir aussi les familles de communes voisines, c'est donc ce qui me conduit à préconiser une formule beaucoup plus flexible et beaucoup plus, me semble-t-il, cohérente avec l'état général du droit communal et en particulier de sa composante funéraire mais en revanche je trouve dommage que les conclusions d'une majorité de la commission, consiste à dire qu'il n'est pas souhaitable d'en débattre, car monsieur le rapporteur, madame la représentante de la commission. Monsieur le rapporteur. Il ne me semble pas du tout inutile que soit proposée aux conseils municipaux comme le propose déjà le code des collectivités territoriales si les communes veulent adopter des compléments au règlement général dès les les ordonnancement funéraire de proposer aux conseils municipaux de cadrer par une délibération, les conditions dans lesquelles, si elle le souhait. Elle propose l'accueil de familles dans une salle municipale, les conditions de réservation. La durée de utilisation de la salle la facturation. Conforme au droit local choisi par le conseil municipal et donc la fin de non-recevoir légèrement sur-argumenté, m'a-t-il semblé. Choisi par la commission n'est pas la seule solution aux problèmes que nous évoquons, et au nom de l'exercice concret et égalitaire. Entre les citoyens

aux besoins des familles concernées D. O. D. décédé concerné serait une bien meilleure réponse à la question posée par nos collègues. Merci, la parole est à monsieur Pierre-Yves Collombat. Pour 6 minutes chers collègues. Madame la présidente, monsieur le ministre, chers, chers collègues, il me paraît difficile de voter en l'état, une proposition de loi qui impose des obligations et des charges nouvelles. à des communes et à des élus qui n'en manque pas, je partage l'objectif des auteurs de la proposition, en ce qu'il répond à l'attente de tous ceux qui ne se reconnaissant d'aucune loi, aucune foi religieuse d'aucune obédience spirituel fut-elle fédéral. Veulent partager un moment de recueillement et de souvenir à l'occasion du décès d'un proche, il est des moyens, des moments où la symbolique en effet est essentielle et la la reconnaissance publique, même sans engagement en fait partie, j'avais la faiblesse de penser que l'amendement de réécriture que je proposais, au nom de mon groupe et ou d'autres ayant le même effet répondraient aux objections que pouvait susciter le texte initial, visiblement, il n'en est rien, pourtant, l'amendement que que je que je propose, supprime en particulier l'obligation de fournir un local, encore moins l'obligation de fournir un local adapté par cas présentant des caractéristiques particulières supprime toute obligation pour les élus de jouer un rôle, à cette occasion, si telle n'est pas leur volonté, tout est facultatif.

Une salle municipale, leur permettant d'organiser des funérailles laïques 2ème modification je pense que laïque ou civil, plus adapté à la circonstance par dérogation au 1er alinéa de l'article, etc, du code de propriété des personnes publiques cette mise à disposition et gratuite, on y reviendra la commune apporte son concours à l'organisation de ces funérailles dans la limite de ses possibilités, donc tout à fait, c'est à chaque fois, c'est à la commune, c'est aux élus de décider la forme et jusqu'où ira leur concours. Et que l'on ne Vienne pas me dire que les pompes funèbres privée offrent déjà ce service, quand c'est le cas, c'est toujours en lien avec un service global et souvent un qui a une crémation ne correspond pas forcément aux souhaits de tout le monde est inutile aussi de faire observer qu'untel service n'est pas gratuit. Contrairement à ce que j'ai entendu il est courant que les communes mettent des salles à disposition d'associations ou de particuliers, sauf seul important alors le fait que tout le monde soit mis dans le même sur un pied d'égalité, qu'il n'y a pas de favoritisme, que l'on ne Vienne pas non plus me dire que le texte n'étant pas après, prix prescriptrice et superfétatoire. Le code général des collectivités territoriales ne manque pas de tels textes, d'ailleurs on a passé toute la soirée hier en mettant en faire d'autres. et tout était tout était libre, tout était prêt, tout est facultatif, très bien, très bien, j'en cite dans l'des conseils départementaux le fonctionnement des groupes d'élus peut faire l'objet de délibération, sans que puisse être modifiée à cette occasion les décisions relatives au régime indemnitaire des élus

le conseil régional peut engager des actions complémentaires de celles de l'État, etc, etc le CG c'était et plein de ce type de mention on trouve pas ça normal, de plus un texte non prescrits petit peut avoir des effets indiquait incitatif, qui ne sont pas insignifiants, comme l'a fait remarquer le Conseil d'État dans son étude de 2013 au droit souple que d'aucuns appellent le droit mou, étude qui d'ailleurs a fait l'objet. Au Sénat, d'une d'une audition et de la commission des lois, qui a été particulièrement intéressante et qui a mobilisé, qui nous a beaucoup intéressé, on n'a pas trouvé ça ridicule, comme dit le vice-président d'alors du Conseil d'État, Jean-Marc Sauvé, je le cite : il n'existe aucune contradiction entre la reconnaissance du droit souple, ainsi que son extension et une meilleure qualité du droit en donnant un plus grand pouvoir d'initiative aux acteurs et, au-delà, plus de responsabilité le droit souple contribue à oxyder à oxygéner notre ordre juridique, hé bien, chers collègues, oxygène, on notera au juridique par un emploi raisonné, il peut pleinement contribuer à la politique de sa boutique sur des normes et à la qualité de la réglementation, c'est pas moi qui le dis, c'est le vice-président du Conseil d'État comment autrement, expliquer que l'on puisse lire

c'est exactement le cas ici le parrainage civil qui me semble un peu plus approprié que celui de baptême civil est l'exemple même des services que les communes qui le désire peut rendre à leurs administrés, il est représentatif de ce que pourrait être des funérailles laïques ou civil comme on voudra-t-elle que le permettront la proposition de loi ainsi modifiée, je ne vous ai certainement pas convaincu, j'en suis certain mais trop de bonnes raisons juridiques me laisse à penser

Monsieur le ministre, madame la présidente, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, donc nous examinons ce jour une proposition de loi adoptée par l'Assemblée nationale, sous la précédente législature, visant à instituer des funérailles républicaine que notre groupe politique a souhaité ce au sein de son ordre du jour réservé. Comme je l'a été dit par des orateurs précédents, ce texte vise à donner un cadre législatif à une pratique qui est déjà largement exercée par les élus locaux, en particulier dans les communes rurales, en effet, il est fréquent qu'un maire mettent à disposition une salle municipale lors par exemple de la disparition d'une personne investie dans la vie quotidienne de la commune afin de pouvoir lui rendre un hommage ou tout simplement lorsqu'une famille en fait directement la demande. Notre souhait est précisément de faciliter les démarches de ces familles qui, en l'absence d'informations suffisantes et 2 dispositions légales sur ce sujet se retrouvent parfois en situation de vouloir faire un choix en inadéquation avec les dernières volontés de leurs proches défunts, faute d'alternative connu. Avec cette proposition de loi, une commune aurait désormais l'obligation de mettre une salle municipale disposition des familles qui le demandent, bien évidemment, si et seulement si elle dispose d'une telle salle, il ne s'agit pas bien sûr d'obliger les élus à en aménager une. Et seulement. Si cette salle et je cite adaptable, ce qui a été précisé tout à l'heure. Ce qui donne une certaine latitude aux maires en matière d'appréciation de ce qui est une salle dite adaptable. L'article unique du texte précise en outre que la mise à disposition de cette salle est gratuite et qu'un officier d'état civil de la commune peu et seulement peut procéder à une cérémonie civile, on peut dire, un objet de civils mais aussi on peut dire, un élu tout simplement peut être présent au moment de la cérémonie civile. Aucune obligation ne serait donc faites aux j'ai lu sur ce point. Je tiens à préciser enfin qu'il n'y a aucune ambiguïté sur application ou non des élus lors du déroulement des obsèques civiles. Cette proposition de loi vise avant tout à assurer une égalité de traitement entre les familles, sur l'ensemble du territoire français, elles doivent disposition disposer de la même. Information et avoir la possibilité de se recueillir, dignement, on a lieu laïc. Suite à la perte d'un proche dans une configuration et un lieu conforme à leurs souhaits. Lors de l'examen de ce texte en commission des lois, un certain nombre de doutes ou le questionnement été formulées et ont amené cette dernière à retenir un amendement de suppression de l'article unique proposé par le rapporteur Loïc Hervé, mes chers collègues. J'attire votre attention sur les conséquences fâcheuses qu'entraînerait l'adoption de cet amendement par notre assemblée, à savoir le projet le rejet pur et simple de l'article unique et donc de la proposition de loi sans possibilité d'examiner les autres amendements qui proposent quant à eux d'en modifier le contenu en effet. Dès lors que la rédaction actuelle du texte ne semble pas satisfaisante aux yeux d'un certain nombre de nos collègues et mettent ainsi fin à la perspective d'un vote conforme de notre assemblée, l'amendement numéro 11 proposé par notre collègue Alain Richard me paraît à même de recueillir l'assentiment d'une majorité d'entre nous. En proposant de donner toute latitude au conseil municipal de prévoir ou non l'usage d'une salle communale accessible au public en faveur des familles qui le demandent et de déterminer les conditions et les modalités de cet exercice, ce qui suppose de pouvoir aussi passer des conventions avec le centre funéraire local mais je rappelle qu'on va évoquer toujours la gratuité mais aujourd'hui des obsèques pour une famille, c'est d'un coût minimum de 5000 euros, donc quand le la gratuité de la salle communale, ça peut aussi participer à elle, alléger la facture, si cet amendement était adopté, nous nous rallierons également à son 2ème amendement modifié on intitulé de la proposition de loi car nous sommes ici dans un esprit constructif, et avant tout pragmatique. Nous souhaitons que ce texte puisse poursuivre son itinéraire parlementaire et être une fine et adoptée définitivement par le Parlement afin que les familles qui le veulent puissent réellement et rapidement s'en saisir. Mais pour cela il nous faut avoir la possibilité technique. D'examiner ces amendements et donc de ne pas adopter la proposition de suppression de l'article unique qui nous sera soumis en 1er lieu. Je précise que la question de gratuité aussi. mes chers collègues, pour conclure, je voudrais souligner que cette proposition de loi comporte une dimension symbolique forte repose sur le triptyque notre devise républicaine de liberté, d'égalité, de fraternité, liberté, tout d'abord de pouvoir choisir des conditions de son départ, liberté pour les familles vraiment conclure de faire respecter ses choix. écoutez, je vous remercie de votre attention. Madame la présidente, monsieur le ministre, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, les rites jalonnent la vie des individus tout autant qui structurent la vie sociale du groupe auquel ils appartiennent, il n'existe d'ailleurs pas de société sans rite à la matière, la Révolution française, a confié un lag important aux communes, elle a un effet vu la reprise en main de grande services auparavant, auparavant assuré par l'Église, Jean Jacques Rousseau a estimé qu'une société républicaine, elle ne saurait être édifié sans l'appui d'une forme de transcendance, il en a appelé donc à sacraliser lettre ensemble collectif et en faisait même à la clé de voûte du contrat social. Ainsi, l'article 1er du décret du 20 septembre 1792 prévoit que les municipalités recevront et conserveront à l'avenir les actes destinés à constater les naissances, mariages et décès, ce mouvement a entraîné la définition d'actes et de cérémonie civile comme le mariage, mais aussi le parrainage République instaurée par un décret du 20 prairial, an 2 il n'a pas eu depuis de consécration normative, le parrainage républicain relevant ainsi de la coutume avant de tomber en désuétude, bien plus récemment, nous nous rappelons que l'article 42 de la loi égalité et citoyenneté définissez un cadre pour l'organisation des parrainages républicains, répondant à une demande exprimée par certaines familles et cet article a été déclaré non conforme à la constitution par le Conseil constitutionnel, nos collègues du groupe socialiste nous invite aujourd'hui à nous pencher sur un autre rituel prévoyant l'institution ne fait funérailles républicaine, la loi du 15 novembre 1887 a reconnu à tout citoyen de la liberté de choisir le caractère civil ou religieux de ses funérailles longtemps monopole des cultes, nous constatons ces dernières une ces dernières années une volonté croissante de nos concitoyens, de bénéficier d'une cérémonie funèbre non religieuse, cette évolution est aussi corrélée par le développement de la pratique de la crémation dans ce contexte que prévoit le texte que nos collègues du groupe socialiste, on choisit d'inscrire dans leur ordre du jour réservé l'institut Les évoque l'institution de funérailles républicaine, qu'en est-il réellement le groupe RDSE s'interroge sur les conséquences pour les communes de l'application de ce texte, l'article unique renferme plusieurs dispositions qui chacune soulève des questionnements la première concerne la notion de salles municipales adaptable selon la rédaction issue des travaux de l'Assemblée, la seconde réside dans l'emploi de l'indicatif prévoyant que la commune met à disposition une salle communale et quelles garanties l'organisation de funérailles républicaine de plus, le texte prévoit explicitement que cette mise à disposition soit gratuite, c'est donc réellement une nouvelle obligation qui est faite aux communes, comme cela a été rappelé à cette obligation, ce double la possibilité pour un officier de l'état civil de procéder à la demande de la famille du défunt à une cérémonie civile faisant un parallèle avec une autre cérémonie bien connue des élus locaux, le mariage républicain son roulements et par plusieurs obligations notamment la lecture d'articles du code civil concernant les devoirs en en matière de funérailles, pas de pareille obligation, pas de cérémonial préétabli, il apparaît donc inopportun de prévoir explicite comme explicitement qu'un officier d'état civil puisse jouer le rôle de maître de cérémonie, enfin, se pose la question de la possibilité d'organiser des funérailles religieuses au sein des salles communales, nous le savons et les auditions menées par monsieur le rapporteur auprès d'opérateurs funéraires le confirme certaines cérémonies funéraires religieuses ont déjà lieu dans des salles municipales, cela nous interpelle et ne nous a pas échappé que les 2 amendements de suppression de l'article unique en fait l'objet d'un avis favorable de la commission des lois leur adoption amènerait à un rejet de l'ensemble du texte, or je dois dire, et hormis les réserves que je viens de rappeler que nous sommes d'accord avec les préoccupations des auteurs de donner plus de solennité aux cérémonies républicaines si cette proposition de loi a été déposée Cedex et que des communes et des maires ont été confrontés à des situations délicates cette PPL dans trouve ça toute sa justification au vu des réserves émises précédemment et afin de ne pas opposer une fin de non-recevoir à cette proposition de loi, le groupe RDSE aurait trouvé plus judicieux de travailler sur le texte initial en l'améliorant, c'est pourquoi nous nous retrouvons autour de la proposition faite à l'amendement 11 par notre collègue Alain Richard cette rédaction ne plus de souplesse aux communes pour s'organiser en évitant les écueils du texte adopté à l'Assemblée, d'aucuns pourraient objecter que la modification ainsi faite n'apporterait pas d'avancée majeure par rapport à la situation actuelle, il est vrai que certaines communes procèdent déjà à la mise à disposition de salles communales pour la tenue de funérailles, mais elle aurait l'Avantage d'inscrire cette possibilité dans le CGC c'était elle pourrait d'ailleurs se doubler d'une meilleure information des communes sur les possibilités offertes en matière de funérailles civiles l'objectif n'est pas d'institutionnaliser cet acte pour créer une religion républicaine, mais bien de reconnaître que certains rituels et symboles sont nécessaires pour faire vivre l'idéal républicain, dans le cas où ce texte n'était pas adopté une réflexion pourrait être menée sur la rive, la revalorisation des cérémonies républicaines mariage parrainage ou encore cérémonie d'accueil dans la nationalité française, en conclusion, le groupe RDSE ne votera pas l'amendement de suppression de l'article unique, préférant plutôt l'examen du texte et l'amendement de notre collègue alors Alain Richard merci.

Monsieur le ministre Madame la présidente, mes chers collègues, nous sommes donc ici pour examiner la proposition de loi instituant des funérailles républicaine présenté par Bruno Le Roux et plusieurs de ses collègues et adopté à l'Assemblée nationale en première lecture le 30 novembre 2016, ce texte vise à imposer aux municipalités de mettre à disposition des familles qui en font la demande une salle dite adaptable gratuite afin de garantir l'organisation des funérailles républicaine, il vise également à confier à l'officier de l'état civil de la dite municipalités la faculté de procéder à une cérémonie d'obsèques civiles dans l'hypothèse où la famille du défunt le requérait ce débat me fait penser au débat que nous avions eu dans cet hémicycle, en mai 2015, sur une proposition de loi relative au parrainage civil ou baptême républicain, selon l'expression souvent consacré si notre commission des lois, soucieuse d'assurer une égalité de traitement entre tous les citoyens avaient approuvé le principe de consécration dans la loi de la pratique du parrainage civil qui fait aujourd'hui l'objet d'une application inégale sur le territoire, elle avait cependant écarté la proposition de faire de fait simples coutumes un acte officiel obligeant les communes. Comparaison n'est pas raison et le sujet qui nous intéresse aujourd'hui est différent mais ils puissent d'une certaine manière, ses racines, de la même inspiration. Celle d'imposer à une municipalité, une nouvelle obligation par rapport à un acte de la vie civile, qui jusqu'à présent n'avait jamais donné lieu à ce type d'obligation pour les municipalités, et pourtant ça se fait. J'ai été moi-même maire pendant 28 ans, d'une commune de 5000 habitants dans la banlieue d'une grande île à Reims pour ne pas la citer, où j'ai personnellement participé à des parrainages civil et accompagné à plusieurs reprises des familles pour des obsèques civiles. Et lorsque la famille souhaité pouvoir disposer d'un local pour se réunir, hé bien nous mettions à sa disposition une salle municipale, moyennant location de la même manière que nous l'avons toujours fait quand les familles des jeunes mariés demandent une salle pour le vin d'honneur d'un mariage tous les maires que je connais et qui dispose d'une salle font de la même manière. Qui plus est, je constate aujourd'hui que les familles qui doivent organiser les obsèques de l'un de leurs proches s'adresse de plus en plus souvent que l'on habite en ville ou à la campagne, à une société de pompes funèbres, lesquels se sont multipliés sur le territoire depuis une quinzaine d'années pour organiser l'ensemble des actes à faire tant sur le défunt pour la conservation de l'Exposition du corps que pour l'organisation et le déroulement des obsèques, ainsi que la réunion de famille et des proches qui suit l'inhumation ou la crémation, j'aurais donc tendance à dire que si la proposition de loi qui nous est soumise, aurait pu avoir sa raison d'être, il y a une quinzaine d'années ou plus, elle n'a plus aujourd'hui la pertinence qu'elle aurait eu à cette époque, ce n'est pas au moment où le problème d'organisation des obsèques civiles ou non et que ce soit en ville ou à la campagne, c'est l'objet d'une véritable offre de la part des sociétés de pompes funèbres, incluant la mise à disposition d'une salle que l'on va imposer aux communes de mettre à disposition un local d'autant plus que cela est toujours possible, si la commune ne souhaite, y compris à titre gratuit, il y a donc pas lieu de légiférer quant à l'intervention d'un officier d'état civil, maire ou adjoint pour organiser une cérémonie à l'occasion de Flex ville cela ne relève pas du chant traditionnel de ses missions, quel rôle aurait-il dans la conduite des obsèques, alors même que préparer et présider une cérémonie funéraire ne s'improvise pas, mais il me semble que dans la pratique, rien ne l'empêche, non plus, il m'est arrivé. à plusieurs reprises les déjà dit d'accompagner une famille au cimetière, dans le cadre d'obsèques civiles et j'ai toujours souhaité tant que j'étais maire et je l'été 28 ans qu'un adjoint le fasse si jeune et si j'étais moi-même à 100. Il m'est arrivé de prendre la parole quand la famille le souhaiter et que je connaissais suffisamment le défunt pour pouvoir en parler mais à quoi cela servirait-il l'office, l'officier d'état civil de prendre systématiquement la parole pour les obsèques d'une personne qu'ils ne connaîtraient pas, pas plus, parfois d'ailleurs que le reste de la famille, surtout à notre époque où la famille est dispersé, s'agirait-il alors. Bah oui, ça je est-il alors de créer un vide civils qui, en quelque sorte viendrait combler un vide, par rapport à un rite religieux, cette proposition de loi, vous l'avez compris risque donc de compliquer un peu plus la vie des collectivités territoriales et des mères sans pour autant améliorer dans bien des cas, la pratique actuelle car je constate en tout cas dans ma commune, dont j'étais 28 ans, mère qui avait, pas de problème de ce de ce côté-là pour de nombreuses raisons, je crois, donc il n'est pas raisonnable d'imposer de nouvelles obligations pour les communes dans ce dossier, parce que comme je l'ai dit, cela est largement réglé aujourd'hui avec les entreprises ne pompes funèbres et parce que la pratique montre que ce n'est pas nécessaire de manière générale.

Madame la présidente, monsieur le ministre madame la vice-présidente de la commission des lois, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, notre Haute assemblée aujourd'hui saisie d'une proposition de loi instituant des funérailles républicaine que nous pourrions nommer aussi obsèques civiles eux ce texte vise à donner une base juridique aux pratiques de certaines communes qui répondait aux demandes des personnes souhaitant des obsèques civiles, il prévoit que les communes qui disposent d'une salle municipale adaptable peuvent la mettre gratuitement à la disposition des familles qui en font la demande, pour organiser des funérailles républicaine et leur permettre de se recueillir, il a également pour objectif de créer un nouveau rite républicain propres obsèques en permettant la présence de l'officier d'état civil chargé de procéder à la cérémonie civile, or je m'interroge sur l'utilité d'une telle démarche en effet la possibilité de choisir des funérailles républicaine est déjà reconnu par la loi depuis la fin du 19ème siècle, dès lors, pourquoi légiférer sur ce sujet, dans la mesure où le droit en vigueur permet déjà, organisation d'obsèques civiles dans les locaux des mairies, c'était le cas dans ma commune, pas plus tard que samedi dernier, pourquoi légiférer en créant une nouvelle obligation à la charge des communes sans compensation financière pourquoi légiférer au risque de porter atteinte à leur libre administration pourquoi légiférer en ouvrant la voie à un nouveau rituel laïque, le maire n'est pas un maître de cérémonie de service funéraire, il n'est pas ordonnateur des pompes funèbres, de grâce, ne ridiculisait pas la fonction municipale transformant par la loi le 1er magistrat de l'Crau de la commune un croque-mort, même si ce métier ets hautement estimable,

laissons les mers libres en la matière, ils connaissent leurs administrés, ils ont à coeur d'être au service des que citoyen ils savent déjà répondre à leur demande, notamment quand on dit chaque fois que nous légiférons beaucoup trop aussi parce que cette proposition de loi apparaît inutile le groupe les indépendants ne la votera pas. Mes chers collègues, je me permets d'adresser un salut tout particulier. à la tribune à une délégation de 2 jeunes citoyens qui porte fièrement d'autres écharpes tricolores, Soyez les bienvenus au Sénat. La parole est à madame Nicole Duranton pour 7 minutes. Monsieur le ministre, Madame la Présidente, mes chers collègues, après le mariage, le parrainage civil maintenant les funérailles républicaine, le sujet n'est pas nouveau, il avait déjà été débattue en 2016, à l'Assemblée nationale puis transmis au Sénat, sans avoir fait l'objet de discussions, les intentions sont louables, mais le texte présente plusieurs écueils : la présente proposition de loi, par son article unique prévoit la mise à disposition obligatoire quand celle-ci existe d'une salle municipale adaptable pour l'organisation de funérailles républicaine mise à disposition qui serait rendue gratuite par dérogation, cérémonie qui, à la demande des familles mobiliserait un officier d'état civil, encore et toujours, contraindre les communes, il a été plusieurs fois mentionné comme argument le fait que des familles qui ne souhaite pas donner de dimension religieuse à l'enterrement de leur défunt se serait souvent vu contraints d'accepter des obsèques religieuses, cette affirmation est fausse, vous le savez comme moi les personnes résolu à éviter l'Église à tout prix ne feront jamais le choix de funérailles religieuses, surtout lorsqu'elles ont la possibilité de s'y soustraire aujourd'hui la liberté de choix existe, l'organisation des funérailles en France est régie par le principe fondamental de liberté des funérailles définie à l'article 3 de la loi du 15 novembre 1887 selon lequel il est possible de choisir entre le caractère civil ou religieux à lui donner pour cela, les pompes funèbres exerce une mission de service public au titre de l'article L. 22 23 19 du Code général des collectivités territoriales, elles, sont chargés notamment de l'accueil de l'accompagnement des familles de la gestion de l'utilisation des charmes funéraire du transport des corps de l'organisation des obsèques donc et de la fourniture de cercueils corbillard du personnel et des objets et prestations nécessaires, le texte de la présente proposition de loi prévoit que par dérogation aux premières alinéa de l'article 21 25 1 du code général de la propriété des personnes publiques cette mise à disposition soit rendue gratuite, autrement dit à la charge de la commune, donc des contribuables locaux car pour citer Margaret Thatcher l'argent public n'existe pas, il n'y a que l'argent du contribuable cela engendrerait en effet une des coûts supplémentaires, comme ceux de l'aménagement du rangement d'une tête Y H de la salle du chauffage, de l'électricité des heures supplémentaires, du personnel retenu pour l'occasion l'article unique de cette proposition de loi est ainsi rédigé : que la mise à disposition de la ça adaptable et rendu obligatoire, pourvu qu'elle existe, on ne lit pas, elle peut mettre mais mais comment comment feront les petites communes aux locaux rares où les plus grandes aux locaux sur zut sur utilisé ayant été maire d'une commune rurale, je n'avais pas de capacité à mettre à disposition une salle pour l'organisation de funérailles ne pouvant pas un air et cette obligation seront-elles pénalisées elles le feront du moins et injustement dans l'estime des familles à qui on avait promis une telle mise à disposition parce qu'inscrites dans la loi, la commission des lois, que je salue pour son travail rejoint d'ailleurs la position de l'AMF, qui est opposé à ce que ses funérailles républicaine devienne une obligation supplémentaire à la charge de nos communes, le texte prévoit également qu'à la demande des familles, un officier des tâches civiles puissent prendre part à la cérémonie pour l'encadrer ou prononcer un discours, c'est leur confier des compétences qui ne relève pas de leur attribution traditionnels comme établir ou publié les actes de l'état civil, comment face à cette demande pourront répondre les communes qui manque de personnel et de disponibilité des élus car c'est bien là le but de cette proposition de loi, ce n'est pas pas lié à un défaut de choix entre funérailles religieuses aux funérailles civiles qui existe déjà, mais de donner un caractère rituel et sacré à ces obsèques civiles, qui sont d'ailleurs appelés dans le texte de loi funérailles républicaine lors de l'examen du texte à l'Assemblée nationale, ses défenseurs n'avait pas hésité d'ailleurs à parler de leur volonté de voir une religion civile qui permettrait de générer une passion pour le régime républicain, mais la République est un système de gouvernement, elle n'a pas fait à faire intrusion dans le cheminement de vie des personnes ni à avoir une vocation spirituelle ou religieuse, ce n'est pas son but, on ne doit pas créer une religion républicaine durant les débats du débat, le député Philippe Gosselin, membre de l'Entente parlementaire pour la famille avait souligné à juste titre, que tous les professionnels du funéraire ont une formation bien précise, parce qu'il faut savoir s'adresser à une famille endeuillée, ce n'est pas un maire ou un adjoint qui sera le mieux à même de remplacer ces professionnels en résumé ce texte qui est clairement une tentative d'insertion de l'État dans la vie privée de nos concitoyens n'a pas de légitimité et sera une fois de plus, une charge supplémentaire pour les mères qui ont déjà beaucoup à faire, alors même que tout existe déjà, c'est la raison pour laquelle mes chers collègues, je voterai l'amendement de suppression de l'article unique et je ne vous je voterai contre cette proposition de loi, je vous remercie.

présidente, madame la présidente, monsieur le rapporteur, mes chers collègues n'est pas question, mes chers collègues de revenir ici sur la longue quête des athées les matérialistes des non-croyants enterrer leurs morts à leur gré le débat qui anime à la Chambre en mai 1882 alors qu'était débattue la proposition de Clovis Hugues tendant à autoriser les obsèques publiques des républicains en offrit tous les arguments et pourtant qui dirait que les termes de notre débat ont changé l'orateur ne déclarait-il pas, alors nous voulons le jour où nous allons dormir dans Le Grand Sommeil, suivant l'expression de Bossuet Bossuet voulant avoir la conviction d'être accompagné par nos amis qui s'ils ne viennent pas saluer en nous une âme immortelle viendront du moins salué dans notre cadavre ce qui a été une âme, ce qui a été la vibration d'une conscience de volonté est aujourd'hui partagé par plus d'un tiers des familles qui souhaitent des obsèques civiles dans une société qui vit pourtant une des, c'est que la sécularisation évidente qui voit les questions religieuses envahir toutes les sphères de la vie sociale, comme si, en réaction, la Team revendiquer sa liberté alors suprême, devons-nous alors contre ce mouvement aller contre ce mouvement où l'anticiper et donc l'accompagner en nous reposant sur les principes fondamentaux de notre République, le 1er étant le principe d'égalité dont on sait qu'il revient à la puissance publique de le garantir, y compris contre les revendications religieuses dans un pays laïc, la religion ne peut envahir la vie sociale et civique et la loi de la République, être mis en concurrence avec la loi de Dieu, chaque citoyen doit pouvoir être reconnu, indépendamment de ses convictions personnelles, or celles et ceux qui n'adhère pas une religion sont privés aujourd'hui de ce moment de recueillement qui ne devrait pas avoir lieu à l'entrée du cimetière où devant la tombe, comme cela est encore le cas, les proches du défunt devrait pouvoir se rassembler dans un lieu ni commerciale ni religieux, un espace municipal semble alors l'endroit idéal pour une réunion civile dommage pour respecter le principe d'égalité des citoyens aussi face à la mort, le sujet n'est pas nouveau : en 2007 puis en 2009, il a été soulevée à l'Assemblée nationale, sans aucune réponse concrète soit apportée, puis en décembre 2016 l'article unique de cette proposition de loi a alors été adopté à une très large majorité, à l'exception de l'extrême droite, un large consensus s'est alors dégagé parce que beaucoup de communes répondent déjà à cette demande des familles, la loi offre certes, depuis le 15 novembre 1887 la possibilité de choisir des funérailles civiles mais dans les fêtes, les familles ne sont pas toujours informés de cette alternative et cela fut le cas par exemple pour le rapporteur du texte, Hervé Féron, qui, dont le père des obsèques religieuses dont il ne voulait pas. Cette proposition de loi permettra ainsi d'inscrire ce droit et de le faire connaître, elle est donc pas inutile comme certains le pensent, comme il n'est pas inutile non plus de rappeler que notre pays est un pays laïc, alors que la loi de 1905 et remise en question, elle s'inscrit aussi ainsi dans la lignée de la pratique des parrainages républicains ou du mariage civil, cette liberté réaffirmé aurait-elle un coût non car elle s'exercera dans la limite des locaux existants, mais qu'une commune possède une petite salle adaptable et elle devra alors être mises à disposition de celles et ceux qui autour du cercueil désire ce court moment d'intimité et de recueillement, on leur paye mais permet simplement une dernière fois de se retrouver autour de leurs défunts et de prendre le temps nécessaire pour dire au revoir. Je dois avouer avoir beaucoup de mal à comprendre l'argument selon lequel des dépenses supplémentaires sont nécessaires, il y a certes le nettoyage et l'électricité, le chauffage pour les quelques heures mais cela ne vaut-il pas pour toutes les cérémonies et toutes les réunions cela la grève aura-t-il le budget communal, sincèrement je ne le crois pas, cependant, je comprends parfaitement l'émoi que peut susciter l'introduction de la notion de gratuité auprès des communes déjà accablés par les baisses de subventions et qui pensent qu'on leur impose des charges supplémentaires, c'est pour cela que nous sommes ouverts à une nouvelle rédaction du texte, encore faudrait-il que nous ayons la possibilité de débattre enfin je voudrais citer Victor Hugo dans notre collègue Jean-Pierre Sueur vient de nous rappeler l'importance qu'il attachait à notre assemblée celui-ci écrivit dans son testament, je donne 50000 francs aux pauvres, je suis convaincu, avec le poète que des funérailles républicaine peuvent aussi être l'expression d'une spiritualité laïque, j'ai le sentiment intime avec ce texte, que nous sommes en phase avec l'évolution de notre société et les demandes de nos concitoyens alors ce texte peut poursuivre son parcours parlementaire, si nous sommes capables de nous entendre sur l'essentiel, ce que nous souhaitons, c'est avant tout donner une base juridique aux pratiques de certaines communes afin de garantir l'égalité entre les personnes souhaitant des obsèques civiles et celles souhaitant des obsèques religieuses, notre groupe et donc ouvert à accepter un texte qui préserve ce principe comme le fait l'amendement numéro 11 proposée par notre collègue Alain Richard je vous remercie. Mes chers collègues, nous sommes très chanceux cet après-midi puisque je vais encore une fois salué une jeune délégation que qui portent également fièrement l'écharpe tricolore et il encore une délégation de 2 jeunes citoyens un petit peu plus haut, soyez les bienvenus au Sénat. La discussion générale est Close, la commission n'ayant pas de bon gré de textes, nous passons à la discussion des articles de la proposition de loi adoptée par l'Assemblée nationale sur l'article unique, je suis saisi d'une demande de prise de parole de Madame Marie-Françoise Pérol-Dumont que j'invite à prendre à nous présenter son intervention. Chers collègues, Monsieur le Ministre, dès lors que pour citer à nouveau boss, oui, nous entrons dans la vie avec la loi d'en sortir, comment nous législateurs, pourrions-nous nous exonérer de contribuer à offrir la possibilité d'un cadre funéraire digne au 30 pourcent de défunts qui sont inhumé civilement, il s'agit juste de respecter le principe d'égalité honorer ses morts en traitant cérémonieusement leurs cadavres et non seulement un fait culturel universel, c'est souvent aussi l'impératif moral le plus solide, le Devoir ultime que s'impose en toutes circonstances les différentes sociétés humaines ainsi s'exprime l'anthropologue Grégory de la place, mais force est de constater que les familles, chargé d'organiser les obsèques civiles d'un proche sont encore parfois démuni pour répondre à se devoir ultime que faire face au vide législatif lorsque surgissent surgissent des difficultés pour obtenir une salle permettant un accueil digne de la dépouille de l'être cher en vue d'organiser un temps de recueillement alors même que l'on est déjà dans la peine, ce n'est heureusement pas, et cela a été dit par plusieurs collègues toujours le cas, nombre de communes proposant tout naturellement une salle municipale, dès lors qu'elles sont sollicitées et qu'elle dispose d'une telle salle, il s'agit ni plus ni moins, de permettre l'extension de cette pratique en la sécurisant juridiquement alors que le principe de liberté pour chacun de choisir le caractère civil ou religieux de ses obsèques, date de la loi du 15 novembre 1987 alors que l'Association des maires de France, chers collègues, l'auriez-vous oublié, a rappelé dans son vade-mecum de 2015, sur la laïcité, son souhait, je cite, de voir les maires de France, mettre à disposition des familles qui le souhaitent une salle communale lorsque c'est possible, aux fins de célébrer des pubs funérailles non religieuses, le vote de cette PPL porté par le groupe socialiste nous semblait devoir faire consensus dans cette assemblée, ce texte, adopté il y a 2 ans par une majorité d'élus à l'Assemblée nationale d'élus issus de divers bancs n'apporte pas de contrainte majeure pour les communes, il ouvre des possibilités, il ne génère pas des obligations, il ne génère pas de coût conséquent il n'enlève aucun droit à quiconque, il ne relève d'aucun jugement de valeur, il ne relève d'aucune idéologie, il vise tout simplement à respecter la diversité des convictions en actant par la loi, l'ultime liberté pour chaque homme de bénéficier de funérailles dignes en donnant un cadre législatif à leur organisation, chers collègues, en votant ce texte éventuellement amendé des judicieuses propositions de notre collègue Alain Richard nous ne pénaliseront pas les communes dont chacun ici connaît les difficultés, au contraire, nous, acteurs ont leur rôle éminent dans la chaîne de l'avis de son début à la fin, au moment où les élus communaux s'interroge de plus en plus sur leur mission, nous adapterons leur réalité fondamentale nous nous opposerons pas croyants et athées, nous contribuerons tout simplement à mettre toutes les familles sur un pied d'égalité. En votant cette proposition de loi nous donnerons corps aux propos de Monsieur de la place que j'ai déjà citée en nous imposant des devoirs funéraire les morts instaure et maintiennent la culture les morts finalement conclure, chers collègues, nous ce que nous sommes. Nous allons examiner à présent 2 amendements identiques de suppression l'amendement numéro 1 il nous est présenté par Monsieur Grand je vous en prie. Merci à un président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Chacun comprendra que. Je ne suis pas philosophiquement opposés à la possibilité d'offrir à chaque Français un libre choix pour leur ganisation d'obsèques, tout ce qui a été dit et qui vient de l'être dit par notre collègue je le partage. Je le ressent au plus profond de moi-même. Mais malheureusement. Nous nous adressons à une France diverse à des communes diverses à des mairies diverses à des infrastructures diverses que nous ici, dans cette assemblée, nous ne pouvons ignorer. Les obsèques civiles peuvent prendre diverses formes selon les orientations et les conditions philosophiques de chacun, cela se pratique déjà couramment dans les complexes funéraires publics ou privés, nous y avons tous participé instituer des funérailles républicaine qui sont de fait des obsèques civiles dans les communes pourraient devenir de fait partenaire dans l'organisation, revient à créer une nouvelle charge obligatoire ou facultative, comme le propose un amendement notre collègue Alain Richard pour les communes et les maires pour les communes autorisées au ne pas autoriser cette pratique de mise à disposition d'une salle municipale pour célébrer les obsèques républicaine ouvrira automatiquement des débats passionnés dans les conseils municipaux. quelle que soit leur décision, les communes qui n'offriront pas cette possibilité, pourront se le voir reprocher par les concitoyens on ouvre voilà un débat sans fin qui malheureusement débordera et peut même dérivé en débat et comportements malsains. Nous savons tous ici que dans les communes des initiatives une ici pas même judicieuse prennent souvent un caractère polémique aussi face à une profonde lassitude des élus locaux. à quelques mois du Rouvray vainement conso ses conseils municipaux préservant les maires et permettez-moi mes chers collègues, de vous dire au regard de mon expérience de plus de 34 ans de mer. Que les situations sont parfois terribles imaginez. Et. Une une un village avec une salle municipale, qui pourraient être mises à disposition, parce que la loi le permet désormais à disposition d'une famille endeuillée par un deuil cruel, je pense en particulier à ceux qui sont, qui soulève les plus grandes, les plus grandes émotions la jeunesse. Vendredi, le samedi, mais nos salles municipales le vendredi, le samedi, tout est prévu, les mariages et ceci, vous imaginez le drame humain et naturellement le maire n'aura maire choisira, choisira bien naturellement ce que choisira le maire, ce que vous auriez choisi ce que j'aurais choisi de décider, c'est évident,

je vais peut-être être beaucoup plus pragmatique que mon collègue Jean-Pierre Grand, mais je crois qu'effectivement, je propose de supprimer 7 heures cet article parce que Danone 1er temps il apparaît inopportun en instituant des feuilles, des funérailles républicaine de créer une charge nouvelle pour les communes, les maires à leur qualité d'officier de l'état civil, ça a déjà été dit, tout est déjà possible, tout est déjà possible, je le disais tout à l'heure, samedi dernier, dans mon village, EDF des funérailles civiles ont eu lieu dans une salle communale sans que cela ne soulève 2 problèmes : en quoi que ce soit, alors pourquoi justement légiférer pourquoi légiférer je ne sais pas, mais nous avons, par exemple en Aveyron, des communes qui auront 30 52 70 habitants et elle va le rester communes ne veulent pas forcément devenir des communes nouvelles chère Françoise mais mais mais elles ont le droit, puisque rien ne les y oblige, et c'est comme une là ont parfois une toute petite mairie et une mini-ça le défaite ou une petite salle où les gens peuvent se réunir, alors pourquoi vouloir demander à ces communes-là d'avoir une salle qui serait obligatoirement affectés à ces funérailles républicaine, d'autant que, d'autant que les contraintes qui sont aujourd'hui liés aux salles accueillant du public sont de plus en plus importante et pèse sur les mers, ainsi que sur les finances communales pour toutes ces raisons et bien moi, je souhaite que nous supprimer cet article. Bien, mes chers collègues, je vais mettre aux voix les amendements numéro 1 et 14 de suppression de l'article unique constituant l'ensemble de la proposition de loi l'adoption de ces amendements vaudrait rejet de l'ensemble de la proposition de loi et à présent nous passons aux demandes. Et puis, question de vote je suis saisi d'une demande par monsieur Madame la présidente, je vous remercie particulièrement Monsieur le Ministre, mes chers collègues, mes chers collègues, il y a, je le pense véritablement un usage de la procédure. Qui risque de nous empêcher de nous exprimer sur le fond et je voulais mais véritablement sincèrement. Monsieur Grand sincèrement vous expliquer ce qui se passe en commission des lois, la semaine dernière, c'est tout à fait régulier, le texte a été repoussée, il n'a pas été voté, donc il n'y a plus de texte, nous arrivons à la séance suivante, monsieur le rapporteur de la commission des lois, et on doit s'exprimer sur LES amendement arrive l'amendement de suppression. Je fais observer de nombreux témoins sont là, qu'il n'y a pas de sens, a supprimé quelque chose qui n'existe pas, puisque le texte n'existe plus, c'est c'est évident, la commission a repoussé le texte. Connaissant bien le règlement, la procédure, notre président, Philippe Bas, il dit mais je mets au mois aux voix l'amendement de suppression de suppression de ce qui n'existe pas, tout le monde comprend et et il nous dit après puisque cet amendement est adopté, tous les autres amendements tombe. Donc il est impossible, nous, nous avons déposé une proposition de loi qui nous paraît nécessaire excellente fin nous le nous la défendrons très bien, mais nous pensons qu'il est préférable que cette proposition de loi soit votée amendée plutôt qu'elles disparaissent purement et simplement bien, or il se trouve et mes collègues, on pourra le démontrer que toutes les objections, je dis bien toutes présenté par Monsieur le Ministre et présenté par le rapporteur tombe dès lors que l'on prend en compte l'amendement d'Alain Christ char d'ailleurs elle tombait déjà que l'amendement de Pierre-Yves Collombat, en grande partie, donc l'amendement dit qu'il s'agit d'une possibilité pour la commune et fait disparaître toute intervention de l'officier d'état civil et l'amendement dit que la commune des libertés modalités mes chers collègues, ce que j'ai l'honneur de vous demander dans les quelques secondes qui reste c'est la chose suivante : si vous voulez, il ne pas adopter mais je je parle à chacune, chacun ne pas adopter cet amendement de suppression la possibilité existerait que ce texte soit voté dans des termes con correspondrait davantage à ce que beaucoup souhaitent et que l'on fasse un travail positif ces coupures, mais c'est très clair, madame la présidente, je pense, merci. Avant de donner Avant de donner la parole sur les autres demandes d'explications de vote et afin que vous soyez parfaitement et. Claire et sur le positionnement de la commission des du ministre que j'ai omis de consulter préalablement et je les prie de bien vouloir m'en excuser, j'ai donné la parole à notre rapporteur lui demander son avis sur ces 2 amendements de suppression.

Doux comme indiqué lors de la discussion générale, je partage l'objectif des auteurs de la proposition de loi. Comme cela vient d'être dit par Jean-Pierre Grand afin de faciliter l'organisation dans les communes de cérémonie civile toutefois pour dire toutes les raisons que j'évoquais et j'ai pas été le seul à les évoquer, il ne me semble pas utile de légiférer sur le sujet dès lors que le droit en vigueur permet-elle déjà l'organisation d'obsèques civique par les communes, vous avez évoqué Madame le vade-mecum de l'Association des maires de France, il y a je crois un guide hébreu bonne pratiques qui étant en cours d'élaboration au sein de la DG Cl et je pense que ce sont des outils à disposition des maires qui permettent de faire un droit souple et qui sont tout à fait en mesure de répondre à nos collègues élus, beaucoup de communes, d'ailleurs, pratiquent déjà ces cérémonies civiles sans que des difficultés particulières nous était remontée, les associations d'élus que j'ai consulté notamment l'Association des maires de France sont défavorables à toutes nouvelles obligations mises mises à la charge des communes sans compensation financière, donc je le dis, la commission des lois, rend un avis favorable sur ces 2 amendements au demeurant monsieur Sueur je ne peux pas entendre qu'il s'agit ici d'un artifice de procédure, je lis l'article 42 de la Constitution du 4 octobre 58 la discussion des projets, des propositions de loi porte sur le texte adopté par la commission, saisie en application de l'article 43 ou à défaut sur le texte dont l'assemblée a été saisi, nous sommes bien en train de discuter du texte qui a été adopté à l'Assemblée nationale, nonobstant le vote de la commission des lois, et si bien d'ailleurs ce quelque chose qui a été précisées en commission en disant que, quelque part, c'était d'une forme de respect à l'égard des auteurs et je serai plus grave encore, sur la suite de ce que je, je veux dire et que ce soit bien pris du, ça n'est en aucun cas un procès d'intention au regard de l'actualité, nous sommes en train de délibérer au Sénat, sur un projet, une proposition de loi extrêmement intéressante mais au regard de l'actualité, je vous invite quand même non pas relativise mais regardez comme la réalité en face. réalité en face. Quel est l'avis du gouvernement. Oui merci madame la présidente, mesdames, messieurs les sénateurs. Je vous en prie. Nous écoutons monsieur le ministre pour l'avis du gouvernement sur ces amendements de suppression. Madame la présidente, je ne reviendrai pas sur le les éléments de forme du droit parlementaire qui ne me regarde pas entreprendre reviens sur les amendes font que j'ai exprimé à la tribune, il y a un instant, j'essaie d'être le plus cohérent du monde et je le redis publiquement pour le journal officiel pour vous et même d'ailleurs pour moi évidemment l'intention sous-jacente est intéressante dans la proposition de loi telle qu'elle a été imaginée par les députés, telle que vous la reprenez cet après-midi monsieur le Président Canet récemment terminé était évidemment intéressant, mais d'autre part, cela fait désormais bientôt 2 mois que je suis ministre en charge des collectivités territoriales et j'organise et j'essaie de tout faire pour qu'on aille vers véritablement un mouvement de simplification et véritablement de faire en sorte que les libertés locales et la confiance ses élus soient véritablement la nouvelle pas doctrine, mais en tout cas le nouvelle manière de s'y prendre avec les élus locaux, élu local que j'ai moi-même été que je suis encore aujourd'hui, je le disais hier soir sur la proposition de loi de Madame, elle, sur les communes nouvelles, nous étions d'ailleurs moins nombreux pour débattre de cette proposition de loi, il faut aussi que désormais on choisisse clairement, peut-être qu'on n'y arrivera pas, mais à trancher définitivement ancien débat soit on dit confiance locales souvent dit Girondins, soit on dit décentralisation sont dit confiance aux élus et auquel cas, on leur fait confiance, aussi, sur cette question funéraire et donc on ne légifère pas, soit on dit plus clairement, mais les 2 se tiennent, intellectuellement, on dit qu'au fond, il faut quand même guidé les choses car on ne fait pas complètement confiance aux élus sur certains aspects et on veut l'égalité mais c'est pas un gros mot que je dis tendez je suis désolé, la loi de la République, elle est là aussi pour garantir des principes d'égalité sur le territoire, donc, et vous dites très clairement avec une démarche qui est la vôtre, non, tenez un principe d'égalité, vous voulez des choses plus contraignantes et plus obligatoire et donc vous voulez l'écrire dans la loi, je veux dire les 2 visions se respecte mais ce que je veux quand même vous dire, sans faire de politique, c'est que lorsque nous prenons-nous parfois au gouvernement ou que lorsque vous nous proposons des mesures qui peuvent être contraignantes au titre de l'égalité tous les bons à juste titre d'ailleurs peut-être parfois nous reproche à nous d'être jacobin et autoritaire et dès lors que l'on va sur des chemins de simplification, de souplesse, de confiance, on veut mettre justement un peu plus de considération dans dans la capacité au maire, officier d'état civil d'organiser avec pragmatisme avec Intelligence, avec compréhension avec humanité les choses dans sa commune, on me dit non, il vaut mieux l'écrire dans la loi, donc moi je respecte complètement notre manière de voir les choses qui surprend un peu de, de, de, de distance par rapport au débat global, mais pour le coup, je me dois d'être cohérent avec ce que j'ai commencé à faire depuis 2 mois et sur lequel je vais continuer, je l'espère, de le faire avec vous, c'est que je pense que si il y a un besoin de liberté locale si un besoin d'oxygène à l'échelle locale, hé bien, et donc il ne faut pas l'écrire dans la loi et c'est pour cela que clairement j'émet un avis favorable aux 2 amendements tels qu'ils ont été présentés. La parole est à madame la vice-présidente de la commission des lois Madame Catherine Di Folco. Merci madame la présidente, monsieur le Ministre, je voulais simplement rappeler à monsieur sueur qu'il n'y a pas eu d'artifice, la commission des lois, si monsieur Sueur, vous avez bien dit ça, la commission des lois a fait son travail de façon tout à fait normal L à examiner un texte qui vient de l'Assemblée nationale de ces travaux, il n'est pas sorti de textes de commissions, donc c'est bien celui de l'Assemblée nationale que nous examinons aujourd'hui et si je reprends le règlement du Sénat et son article 49, il est dit les amendements sont mis aux voix dans l'ordre si après amendement de suppression et ensuite les autres amendements en commençant par ceux qui s'écartent le plus du texte, donc nous avons satisfait à la procédure. Pierre, je vous en prie, à présent, nous poursuivons dans les explications de vote, je donne la parole à monsieur Ouzoulias. Merci madame la présidente, monsieur le ministre, chers collègues, hier nous avons débattu longuement du voile et de la loi qui interdit le port du voile dans l'espace public en France vous nous avez expliqué que le comité des droits de l'homme de l'ONU ayant rendu un avis contraire, bien que il n'y ait aucune valeur juridique et aucune Cancès hanche juridique de cet acte, il était essentiel, essentiel, pour réaffirmer les valeurs de la laïcité et je vous cite, alors qu'il y avait aucun objet juridique, vous nous avez dit et on vous a suivi sur ce point qu'il fallait réaffirmer les valeurs de la République, vous l'avez dit, et nous avons voté, nous avons accepté ce débat qui est un débat fort sur la laïcité Madame Duranton, je suis désolé, mais nous n'avons pas les mêmes valeurs de la laïcité, la laïcité, c'est pas la religion de l'État, la laïcité n'a pas de rites spécifiques elle opposerait à une autre religion, la laïcité, c'est l'organisation des relations entre les citoyens et les citoyennes au sein de la République, ce qui n'a rien à voir, 1er point. Dans leurs Dans leurs relations entre et par rapport à la République, il existe déjà 2 actes fondateur que vous le vouliez ou non, le baptême civil organisé par la loi du 20 prairial, an 2 8 juin 1794

1er point 2ème point il existe à côté du mariage religieux un mariage civil qui ne s'y oppose pas, il est complémentaire, on peut faire les 2, généralement, c'est ce que c'est, c'est Merci, ma question est celle là alors qu'il y a un baptême, alors qu'il y a un mariage, pourquoi, pourquoi il n'y aurait pas une cérémonie d'enterrement, selon les mêmes principes pourquoi expliquez-nous philosophiquement qu'est-ce qui empêcherait de poursuivre la vie du citoyen et de citoyenne dans le corps social et dans le corps de la République par cette ultime cérémonie je ne comprends pas, et je pense qu'il serait bien que vous ne vous réfugiez pas derrière des arguments techniques liées

Madame la présidente, monsieur le Ministre, mes chers collègues, lorsque j'ai lu pour la première fois cette proposition de loi proposée par nos collègues socialistes, je me suis posé aussi toute une série d'interrogations, comme l'ont fait, tout à l'heure monsieur le rapporteur, et Monsieur le ministre pour rendre ce texte, à mes yeux, acceptable, je me suis permis de proposer 4 amendements qui sont d'ailleurs inscrits à l'ordre du jour pour remédier aux critiques à tout le moins, les plus flagrantes que je pouvais faire à l'égard de ce texte, premières propositions d'amendement visait à revenir sur l'obligation faite aux communes de mettre gratuitement à disposition une salle pour célébrer ses funérailles civiles 2ème amendement visait à revenir sur la possibilité qu'a, en fonction de cette PPL, l'officier d'état civil de procéder à la cérémonie civile parce que je pense que franchement l'officier d'état civil, a bien d'autres choses à faire que cela et que, comme l'a dit tout à l'heure à la fois le rapporteur mais également, comme l'a dit monsieur le ministre, il y a à tout le moins une égalité à mettre en oeuvre dans cette intervention intervention de l'État de l'officier d'état civil et enfin les 2 derniers amendements visaient simplement à compenser financièrement pour les communes qui ferait cela les coûts, les charges occasionnées par cette manifestation pour cette compétence nouvelle je rappelle, mais faut-il le faire ici tout ce qui leur est tombé sur le dos déjà assez commune depuis quelque temps, à la fois le Pacs, l'immatriculation, les modifications la rupture, mais également le changement de nom de prénom à l'état civil, le changement de nom dans un cas particulier échappé grâce au Conseil constitutionnel, mais mes chers collègues, mais je suis sûr que ça va revenir au parrainage civil et tout ça gratos, donc à tout le moins, il faut compenser financièrement, je suis maintenant face à la proposition de monsieur Grand et de monsieur Marc visant à supprimer cet article unique, vous l'avez compris en fonction de la règle qui peut le plus peut le moins, moi je voterai sans état d'âme, ces 2 amendements. La parole est à monsieur Bonhomme pour explication de vote. merci madame la présidente, monsieur le ministre, moi je crois que ce débat n'a pas besoin d'une idéologie particulière je trouve cousin mettez là ou n'en a pas besoin, les maires, comme ça a été dit ma par collègues ont depuis des années, se plaignent de manière continuelle de l'alourdissement des charges nouvelles des rôles nouveau, ça a été dit par le parti et tout un tas d'autres d'autres missions, et là on va toucher quelque chose de d'extrêmement délicat, donc je crois que cette PPL n'a, n'a pas, n'est pas opportune, tout simplement parce que la ritualisation de la mort n'a pas vocation à être institutionnalisé au niveau d'une mairie, je crois que l'argument économique, il a été donné, ça va créer une charge nouvelle l'argument juridique : on nous a opposé le vide législatif mais pourquoi créer un un plein législatif alors qu'il y a une pratique, qui donne la part des personnes satisfaction et surtout et surtout qui ne mettent pas les maires dans une position délicate,

autour d'un décès, donc je crois que on va mettre en va déchaîner les passions va mettre inutilement les mères en position difficile et délicate qui ne seront pas comment traiter cette situation et je crois vraiment que cette cette ajouter des difficultés là où il n'y en a pas actuellement et puis surtout, je crois que cette PPL elle vraiment le signe de l'air du temps, on en a eu la fessée à la semaine nationale et là aujourd'hui on a ce texte-là qui, finalement, la traduction de d'une saturation des symboles, on s'attache à des symboles à tout propos à tout propos ah, en plus du problème de du juridique, et je crois qu'on se laisse emporter par cette ce mouvement général, qui est tout à fait, qui tout à fait dommageable, la parole est au maire à la parole effectivement l'esprit girondin, c'est-à-dire la confiance aux élus et je crois que c'est tout le contrat qui nous est proposé par ce texte. La parole est à madame Gate pour explications de vote. Madame la présidente, monsieur le ministre, monsieur le rapporteur, madame la vice-présidente de commission, mes chers collègues, je voudrais tout d'abord dire avec beaucoup de sincérité, que le sujet dont nous débattons aujourd'hui est un sujet et nous le savons tous ce qui est un sujet extrêmement privé et d'une grande gravité le l'intention que vous portez vous honore et je crois que, ici personne sur ces bancs ne peut contester cet instant un peu particulier qui relève à la fois de la vie privée, mais que certains d'entre nous rattachent à des convictions religieuses ou philosophiques, maintenant moi je partage ce qui a été dit par monsieur le ministre, peut-on demander aujourd'hui au travers de votre texte à créer, comme l'a dit Pierre Ouzoulias une cérémonie républicaine de funérailles, on n'en est plus à la mise à disposition d'une salle adaptable et mon cher Pierre, le baptême, pardonnez-moi, dans ce temple de la laïcité est un sacrement eux religieux éminemment catholique donc il vaudrait mieux parler de parrainage républicain si je fume, permettre de de corriger quand nous parlons d'une salle adaptable qu'est-ce que ça veut dire adaptables aux besoins et aux attentes d'une famille qui sont particulières dans des situations extrêmement douloureuse qui crée chez les familles une émotivité tellement forte que ces familles vont s'en prendre aux maires qui pourra ou qui ne pourra pas mais cette salle à disposition donc je crois que nous, engendrant des risques de contentieux extrêmement importants, entre autres, parce que le mot adaptable et justement indéfinissable et je pense qu'on ne peut pas demander à la République de gérer notre vie privée, si nous sommes une république laïque, il convient d'entendre et de reconnaître que les éléments de la vie privée en dehors de l'enregistrement des actes d'état civil ne relève pas de la République sincèrement Michel Collet peut-on demander à un maire de devenir un prêtre de la République et d'officiers non non mais d'officier dans des cérémonies qui seront conformes aux aspirations philosophiques de chacun, La parole est à madame. Pour explication de vote. tout d'abord je voudrais évoquer le propos de monsieur Louis qu'Hervé qui a, qui a laissé entendre, j'espère que ces mots ont dépassé sa pensée sur le fait que, finalement, considérant l'actualité à Strasbourg, c'est bien ça que vous viviez je pense, hé bien, nous ne pourrions nous ne pourrions pas débattre d'un texte proposé par le groupe socialiste, bon il faudrait arrêter tous les travaux, monsieur, mais je le regrette, nous devons délibérer, nous devons légiférer même si manifestement vous avez décidé de mettre à mort, permettez-moi l'expression, par ces 2 amendements, le texte que nous souhaitons faire débattre tout simplement ici même, ce que nous voulons, par ce texte, c'est permettre à de très nombreuses nuits française de pouvoir enterrer leurs défunts dans d'excellentes et de meilleures conditions que celles qui sont prévues aujourd'hui, vous ne le souhaitez pas en tout cas pas dans les conditions que nous avons imaginé et dans ce cadre, nous étions prêts à prendre en considération. Et je parle bien commissionnaire à prendre en considération les propositions constructives porté par notre collègue Alain Richard, mes chers collègues, nous sommes dans une niche dite socialiste républicaine, nous souhaitons pouvoir porter notre texte jusqu'au bout, en tout cas pouvoir en débattre jusqu'au bout par vos 2 amendements, vous décidez de nous empêcher de mener à bien ce débat, nous le regrettons manifestement un scrutin public va être sollicité en la matière, je crois que ce ne sont pas des bonnes méthodes pour les relations entre les groupes dans cette haute assemblée, quelles que soient les arguments pouvoir aller jusqu'au bout de l'analyse d'un texte fait partie je pense des bonnes manières que nous devons adopter entre nous je regretterai donc au nom de mon groupe que vous puissiez nous empêchait par votre décision de mener à bien dans les bonnes conditions ce débat. La parole est à madame. Pour explication de vote. Non Madame Pérol-Dumont merci madame la présidente, très sincèrement, mes chers collègues, j'ai trouvé un peu regrettable les leçons sur la confiance accordée aux élus locaux, si nous n'accordions pas la confiance aux élus locaux, nous ne serions pas sur ces bancs, mes chers collègues, de quelque côté que nous siégeons donc le principe est qu'effectivement, représentant du territoire, élu par les élus locaux, nous faisons confiance aux élus locaux et nous avons, pour la plupart d'entre nous étaient pendant de longues années, élus locaux ou responsables d'exécutif, mes chers collègues, pour revenir au fond mais qu'est-ce qui chers collègues de la majorité sénatoriale qu'est-ce qui vous inquiète autant dans ce texte de vouloir brider le débat de vouloir empêcher le débat par cet amendement de surprises, de suppression, j'ai bien vu finalement un certain malaise chez notre collègue cher Jean-Pierre Grand lorsqu'il a, il a présenté cet amendement, il me semble que oui, ce sont des arguties, l'idée de coûts supplémentaires pour les communes, l'idée de débat que cela pourrait générer et vous savez bien, au fond de vous-même qu'il ne résisterait pas au au débat que nous souhaitons avoir ensemble ici pour amender ce texte et de largement dans le sang bleu dans le sens que vous souhaitez non il me semble, et je ne voudrais froisser personne qu'il y a derrière tout cela, autre chose, il y a chez certains. Le refus d'admettre les obsèques non confessionnel, il y a le refus d'admettre que la spiritualité n'est pas le propre des religions que oui on peut vouloir des obsèques civiles tout en relevant d'doute une d'une spiritualité, tout en voulant entendent rencontrer un temps d'échange alors, mes chers collègues, ces débats sont derrière nous depuis plus d'un siècle et ne les remettons pas à l'ordre du jour, et s'il vous plaît, travaillons ensemble pour améliorer ce texte dans le sens que vous souhaitez. Finalement, quelques mois, nous avons assisté. à la position de la droite sénatoriale sur les écoles privée hors contrat. Nous avons assisté à la position de la droite et Nathan qui a refusé notre demande de commission d'enquête sur la pédophilie dans l'église et nous assistons aujourd'hui au refus de la possibilité pour nous électeurs. De pouvoir organiser des funérailles républicaine je croyais en arrivant au Sénat arrivé dans une institution qui défendait, bec et ongles la laïcité je découvre aujourd'hui le pouvoir. De la religion dans l'engagement qui est le vôtre. Sachant que nous sommes tous ici des élus locaux et que j'entends des arguments, j'entends des arguments chacun disant tout cela se passe bien et cela n'est pas un problème, et pourtant nous refusons que ce soit dans la loi. La 2ème chose que je voudrais dire c'est au rapporteur de la commission des lois, lorsque monsieur le rapporteur. Alors que Paris a été dévasté, le 1er décembre. Nous recevons tous sur nos mails. Mail des services de la séance, nous informant que le groupe, les républicains, a décidé d'inscrire dans sa future niches, comme l'on dit un texte sur la sécurisation des passages à niveau, on comprend qu'effectivement il y a une cohérence lorsque les gilets jaunes s'apprête à Reder filer encore une fois, samedi dernier, que faites-vous dans cet hémicycle vous voté l'allégement de l'exit tax alors lorsqu'on prétend que il faut que dans cet hémicycle, nous soyons en phase avec ce qui se passe dans le pays et qu'on ose à court d'arguments Monsieur Hervé à court d'arguments voulant vous opposer à toute force à cette proposition de loi vous osez instrumentaliser de manière indécente. Ce qui s'est passé à Strasbourg, je vous renvoie à votre papa faiblesse l'exit tax et votre formidable proposition de loi sur la sécurisation des passages à niveau, donc vous allez vouloir encore une fois plié le genou devant l'engagement religieux, pour notre part, nous soutenons notre proposition de loi. La parole est à madame sur La parole est à Madame Lherbier pour explication de vote. totalement pratico-pratique, chers collègues, Pierre, vous avez demandé tout à l'heure pourquoi des parrainages républicains des mariages républicains et pas des des funérailles écoutez c'est très simple, était maire d'une commune de 1500 habitants alors autant un mariage et un baptême on le prépare à l'avance

temps de canicule donc tout d'un coup ils sont rendu compte il y a des enfants, des personnes âgées, des bébés, on va pas pouvoir le faire au cimetière, comment on se retourne, hé bien, franchement c'est indécent de mettre un accord entre 2 buts de basket, sachant que 2 heures après, il y avait le tournoi des petits poussins de la Nièvre qui venaient se retrouver c'est indécent de mettre un corps dans la salle qui est préparé pour le marché de Noël parce qu'il faut improviser etc, on n'a pas qu'est ce qu'on appelle un local approprié, on

je crois que tout le monde sait s'est exprimé et à travers les explications de vote, on a déjà, on peut mesurer quels sont les arguments des uns et des autres, alors il existe au sein de toutes les commissions qui travaillent la possibilité pour le président de la commission ou le rapporteur d'appeler en priorité un amendement pour d'abord le faire voter, c'est une procédure qui est utilisée régulièrement par la commission des lois par toutes les commissions en tant que président, à votre place, madame la présidente, je l'ai vu se mettre en place plusieurs fois, ce serait quand même quelque chose d'intéressant de pouvoir au moins débattre sur le 1er amendement qui est l'amendement de monsieur Richard ça n'empêche aurait rien au résultat final, puisque si vous voulez voter contre cette PPL, vous pouvez le faire, vous aurez la possibilité de le faire mais ça permettrait quand même peut-être d'avancer un petit peu et de répondre au demande du groupe socialiste qui souhaite débattre qui souhaitent amender une PPL sur lequel vous avez vous-même fait remarquer, fait d'un certain nombre de remarques et si remarque sont prises en compte par Alain Richard et par d'autres mais ça permettrait au moins de s'exprimer et en fin de compte, le vote vous appartiendrait puisque vous demander un scrutin public, vous pouvez le garder et ça nous permettait de débattre tranquillement, un peu plus, alors il y a là je comprends bien qu'ils sont pressés de passer de faire passer rattrape notre proposition de loi mais ce serait à mes yeux un peu plus démocratique. La parole est à Madame Lherbier pour explication de vote. Oui, mais la présidente je voterai les amendements de substitution avec grand plaisir parce que au départ quand j'ai déposé les amendements, c'était justement pour soulager les obligations faites aux maires, je trouvais que c'était quand même incroyable de devoir encore imposer aux maires des contraintes, le fait de, de réfléchir sur les différents moyens pour aider les familles en deuil, on peut en avoir sans y être contraint, toutes les mères, tous les maires, Paul forcément la leur concitoyens dans des moments douloureux, c'est pas la peine de le mette dans la loi et donc c'est avec plaisir que je me rallie à l'amendement de monsieur, de monsieur La parole est à Monsieur Detraigne pour explication de vote. Rapidement, j'avais demandé la parole à la suite d'une intervention de notre collègue Marie-Pierre de La Gontrie qui nous qui disait, je cite, que qu'on voulait empêcher d'organiser des funérailles républicaine, c'est pas du tout cette question-là, on veut pas empêcher d'organiser des des funérailles républicaine, la preuve c'est qu'il a et ça existe aujourd'hui, on estime qu'il n'y a pas besoin de mettre dans le marbre l'obligation de, de, de pratiquer des funérailles républicaine j'étais enfant, coeur, j'ai été interne dedans chez les Frères des écoles chrétiennes, j'ai été grand clergé et j'ai et j'ai présidé au moins une dizaine de fois à des funérailles républicaine c'est pas antinomique, voilà, il y a pas besoin de loi. Et enfin, la parole est à monsieur Grand pour explication de vote nous écoutons notre collègue. Mes chers collègues. J'avais justifier mon mon amendement par le fait que dans les conseils municipaux autorisés ou ne pas autoriser ouvrirait des débats et que ces débats dériveurs et dans les conseils municipaux, nous venons de donner aujourd'hui l'exemple dans une assemblée extrêmement sage qu'il est resté mais où est sorti naturellement un débat sur la religion contre la religion pour la religion pour la pour la laïcité contre la laïcité, imaginez-vous dans les villages, imaginez-vous les conseils municipaux dans les villages, voire dans des communes plus grandes sa dérive aura de la même façon, avec beaucoup plus de brutalité, voilà pourquoi je crois que cet amendement est justifié ce soir encore plus à l'issue de ce débat qu'avant le débat. Monsieur fiché pour explication de vote. Oui, madame la présidente, monsieur le ministre, j'avoue que je suis un peu stupéfait de voir comment on peut rendre complexe, quelque chose qui est infiniment simple et ce que cache cette complexité parce que de de quoi il s'agit de demander aux municipalités de mettre à disposition la salle municipale pour le déroulement d'obsèques civiles, c'est tout, alors après, vient la question de la gratuité ou non, c'est un problème qui peut se régler à travers des amendements qui sont proposés, donc je ne vois pas pourquoi autant de passion, sur un service qui peut être rendus aux familles parce qu'on évoque très peu, la situation des familles mais je puis vous dire que cette proposition, à partir du moment elle devient possible dans toutes les communes, c'est une réponse aux familles qui saute à un moment donné dans l'ignorance et qui, je le trouve dans l'obligation d'avoir des obsèques religieuses, là où elle ne voudrait que des obsèques civiles, ne serait-ce que pour respecter la volonté des défunts, donc je suis, je souhaite vraiment que l'on réfléchisse tous ensemble avant de voter cet amendement de suppression parce que je vais vous dire très honnêtement que nous avons proposé de reprendre cette proposition de loi votée à l'Assemblée nationale, nous étions tous convaincus qu'il n'y aurait aucune difficulté à un vote unanime sur une proposition aussi simple, je vous remercie. Monsieur le rapporteur, vous souhaitez prendre la parole madame la vice-présidente Catherine Di Folco. Celui que Madame la Présidente, merci, je voulais répondre à Monsieur Berreri puisque effectivement vous nous faites part de la faculté, que la commission a d'appeler un article en priorité, ce n'est pas la position de la Commission, au terme de ces travaux d'hier donc, la, la Commission a souhaité examiner le 1er amendement, celui de Monsieur là, a donné un avis favorable, donc je maintiens la position de la commission d'hier, merci. Merci madame la présidente, monsieur le ministre, chers collègues pour pourquoi compliquer un objet, un objectif qui a définitive, elle est très très simple, dans le respect des des confessions et et des croyances de chacun, que de créer de proposer, d'une certaine manière, nouveau service public à notre population Dan, jeune contexte de société dans un contexte sociologique ou moi je remarque comme nous tous ici, que les familles sont éclatées et qu'à l'eau qu'à l'occasion de funérailles, souvent, les gens viennent de très très loin, à fortiori sur nos territoires ruraux et Hewlett indispensable que les familles puissent se rassembler : ça ne coûtera pas un centime à nos communes à nos mairies, on met bien à disposition des salles des fêtes pour les familles qui le souhaitent, ça ne coûte rien, ça ne pousse pose le problème à personne, je crois qu'on on va et vous allez chercher des arguments qui n'ont pas lieu d'être pour quelque chose, encore une fois, de très très simple mais qui répondrait à une attente profonde et justifiée de la population française. Bien, mes chers collègues, je mise aux voix les amendements de suppression. Sont de l'article unique constitue un ensemble de la proposition de loi instituant des funérailles républicaine, j'ai été saisi d'une demande de scrutin public par le groupe, les républicains, le groupe Union centriste et le groupe les indépendants sur des amendements et 14. Je vous rappelle l'avis de la commission défavorable à vie du gouvernement est également défavorable, il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article. débuts de la cuisse pour TF1 Gourette suffisamment de suppression. Je je reprends l'avis de la commission et favorable sur les amendements de suppression, c'est bien ce que je vous ai annoncé, on est d'accord, il va être procédé au scrutin public dans des conditions fixées par l'article 56 du règlement. Et le scrutin va être ouvert dans quelques instants, le scrutin. Voter

le scrutin est clos, j'invite les secrétaire à procéder au dépouillement du scrutin.

le résultat du scrutin numéro 39 sur les amendements identiques numéro à 14 rectifier, compte tenu de l'ensemble des délégations de vote accordé par les sénateurs au groupes politique et notifié à la présidence, nombre de votants 343

Je vais suspendre pour quelques instants, la séance 7 sera reprise dans 5 minutes.

dans 5 minutes. L'ordre du jour appelle l'examen de la proposition de résolution en faveur de la création de paiements pour services environnementaux rendus par les agriculteurs,

Dans la discussion générale, la parole est à monsieur moto G, auteur de la proposition de résolution pour 10 minutes chers collègues. Monsieur le président, monsieur le ministre, chers collègues, la proposition de résolution que nous soumettons aujourd'hui à notre débat a été élaboré par les sénateurs Cabanel et et et Tissot ainsi que moi-même, elle est présentée au nom de groupe socialiste et républicain, chers collègues, au moment où je m'exprime devant vous des tracteurs ont pris place devant la préfecture de départements, le Gers, à Auch, le sujet d'aujourd'hui, vous le savez, est celui de la redevance pour pollution dit les agriculteurs qui se manifeste ainsi ne porte pas de gilet jaune, mais ils connaissent eux aussi les conditions de vie difficiles qui justifient leur mobilisation pour connaître la dignité qui la leur, je m'avancerais à dire qu'ils en ont assez des apitoiement, d'où qu'ils viennent, je m'en garderai donc qu'en vous disant qu'ils attendent de nous que par nos propositions, nous les aidions à vivre décemment de leur travail et ils disent régulièrement, nous voulons des prix pas des primes, le système actuel le permet-il, on ne sait que nous le permettra-t-il demain pour tous, on peut en douter, mais on le souhaite, bien entendu, à partir de là, notre Dave dans notre notre devoir à leur égard et de proposer en nous projetant à l'écoute des attentes de la société et des grands enjeux que nous devons relever collectivement notre agriculture est incontestable m'aime contestable ment à un tournant de son histoire, changement climatique, raréfaction de l'eau, ressources naturelles épuisement de notre biodiversité concurrence économique exacerbée insuffisance et une stabilité des revenus, autant de défis qui rendent aujourd'hui le métier d'agriculteur de plus en plus difficile et incertain à ces contraintes climatiques économique et conjoncturelle, s'ajoutent des attentes sociétales de plus en plus forte en terme de préservation de notre environnement et de qualité des produits et des aliments que nous consommons ces attentes se transforme malheureusement souvent un critique et elle participe d'une forme de détérioration de l'image du métier d'agriculteur depuis quelques années, la grille bashing, ça suffit, et nous vous suivons là-dessus monsieur le ministre, il faut expliquer aux consommateurs, aux citoyens et les agriculteurs ont pris conscience de cela, ce que l'on fait, comment on le fait avec quelles contraintes et dire aussi ce que l'agriculture et les agriculteurs à portent à la société, au-delà des apparences immédiates qui limitent leur rôle au seul acte de production pour nous et cet homme, point essentiel : il ne s'agit pas de stigmatiser les agriculteurs mais au contraire de prendre en compte et de reconnaître à terme l'ensemble des effets bénéfiques de leur action sur la société, face à ces nouveaux et nombreux défis aux mutations sociétales et environnementales qui sont engagées, nous devons apporter de nouvelles réponses les orientations que la Commission européenne a posé pour les principes de la future PAC nous engage aussi à discuter, à proposer des pistes au gouvernement, les paiements pour services environnementaux PSE apparaissent comme un outil pouvant nécessité économique et prise en compte des enjeux climatiques et environnementaux mais au préalable, il est important de se mettre d'accord sur les mots, nous retenons comme définition du PSU, les effets des externalités positives de l'aviculture sur les écosystèmes, effets qui sont engendrés par des modes de production ou des pratiques agricoles adaptées en d'autres termes, il s'agit d'encourager en les rémunérant dans la durée les pratiques qui permettent d'améliorer la santé et l'efficacité agronomique et environnemental des écosystèmes, il ne s'agit donc plus seulement de compenser les surcoûts des manques à gagner comme les dispositifs actuels de type avec le permettent, mais bien de rémunérer de façon permanente à des pratiques apportant une plus-Value environnementale ou climatiques des exemples existent déjà dans le domaine privé, l'un des plus emblématiques et celui de la société, je vais la citer Perrier Vittel qui a développé dans les années 90 une politique de protection de ces sources en contractualisé avec l'exode des exploitants agricoles pour qu'ils changent leurs pratiques et préserve les nappes phréatiques, dans mon département, le Gers, une société qui produit du popcorn bio à contractualiser avec ces producteurs de maïs, une part du prix d'achat en conséquence des réductions d'émissions d'autres que permettent des techniques de travail simplifié du sol et de couverts végétaux qui améliore la séquestration du carbone dans le sol par ces PSE, il s'agirait également de valoriser le rôle indispensable jouer par les agriculteurs en matière d'aménagement du territoire et d'entretien de nos paysages dans nos massifs montagneux le pastoralisme rendent des services d'intérêt général au territoire à la société, en évitant les incendies les avalanches, tout en étant aussi souvent des lieux de tourisme, entendons-nous bien : le passent au nord le pastoralisme, comme toute activité agricole doit se rémunérer sur son activité économique propre mais l'épée se doivent permettre aussi de reconnaître ce qu'il apporte à l'intérêt général, souvent par exemple les incendies en Corse où la difficulté de leur maîtrise résulte de l'abandon de zones autrefois exploitée, c'est là une démonstration par l'exemple et a contrario de la justesse du concept d'EPS le même sujet se pose dans les mêmes termes pour les territoires ruraux et hyper ruraux en déprise agricole ou menacé de le devenir, la sortie de certaines éleveur des zones défavorisées renvoie à cette problématique d'intérêt général et on sait que le bilan carbone de la disparition des prairies ne sera pas positif, l'agriculture est profitable pour Lance Lansana de la société et les citoyens en bénéficient au quotidien, bien souvent sans s'en rendre compte, pour éviter les incompréhensions, je veux rappeler ici quelques principes auxquels nous sommes attachés à propos des PSU, d'abord on ne doit toujours partir des marchés et de l'attente du consommateur les PSE doivent conforter le développement des territoires au plan économique, social et bien entendu environnemental, les pièces doivent être pensées avec les professionnels et toutes les parties prenantes dans le cadre de démarches de projets territoriaux dans les périmètres peuvent aller de l'exploitation de base au grand territoire il faut conditionner l'épée ce à une activité agricole productive, paix, ceux-ci n'y a pas d'agriculture, pas de mise sous cloche, non plus des territoires agraire. Le PS ne doivent pas faire l'objet d'un cadre réglementaire rigide, il ne s'agit pas de rajouter des normes aux normes adaptabilité et subsidiarité doivent être au coeur du dispositif, la question du paiement des PSE par le consommateur dans les prix ou DPS par le contribuable dans les aides doit être discuté les PSE peuvent aussi être valorisé entre acteurs privés, les paiements ne doivent pas se substituer, c'est un peu une 13ème portant sur lequel j'attire votre attention aux aides PAC que l'on connaît et dont on sait qu'elles vont baisser probablement, très probablement, parce qu'elles répondent à des objectifs radicalement nouveau, les PSE doivent venir en plus, les 150 millions du plan biodiversité présenté en juillet dernier et qui était prévu au budget 2018 pourrait utilement les financer, ça ne touche il aucunement au 1er pilier l'État par l'intermédiaire de l'INRA a travaillé la question du PSE au plan scientifique, économique et juridique, le ministre agriculture nous le dit le nous, nous le dira certainement, mais j'ai noté qu'en 2019 des guides pratiques seraient mises à disposition de l'État dans les agences de l'eau à disposition des collectivités et des privés et qu'il s'agissait d'entreprises, d'associations, de fondations ou autre, une phase de mise au point de tests in situ pourrait intéresser de nombreux territoires le Gers pour être avec d'autres y participer, la reconnaissance de la valeur environnementale produite par les pratiques culturales hein n'est pas à ce jour possible dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce, mais nous pensons que les PSE devraient être traitées à l'aune des engagements de la conférence des parties et donc déboucher sur des classements où M. c'est les permettant de type boîte verte pour nous les manettes les Malek et le PS, ce sont 2 outils complémentaires à l'ne remplace pas l'autre, la création de PSE ne serait impliqué une disparition ou même une diminution à court terme des Budgets consacrés aux mecs les récentes propositions législatives de la Commission européenne pour la future PAC semblent ouvrir la voie à la possibilité de création de ces PSE au sein du 1er pilier possible même au titre du dispositif appelé par la commission Ecosse Kimouyou nous sommes et je tiens à insister là-dessus, pour le moins réservé sur cette possibilité d'autant plus que les aides directes vont diminuer notre position et la suivante, tant que la question des prix producteurs ne sera pas réglé et donc que les paiements Directs seront indispensables les PSE ne pourront ainsi substituer et nous pensons qu'ils devront être financés sur des fonds environnementaux spécifique en tout état de cause, n'attendons pas que l'Europe pour entamer les actions concrètes, fusse-t-elle expérimental en demande un gouvernement d'engager concrètement cette démarche de mettre en débat le dispositif, nous ne prenons en réalité aucun risque améliorer un peu le revenu des agriculteurs tout en répondant aux enjeux sociaux et sociétaux territoriaux et environnementaux qui se posent à nous, collectivement, c'est à cela que peuvent contribuer les PSE je n'ai plus le temps, je voulais vous rappeler les attendus ou les propositions de cette proposition de de résolutions, je les ai évoqués, il ne me reste plus de temps, mais ce que je tenais à dire en conclusion, c'est qu'il faut que nous nous prononcions sur ce coup-contiennent sur ce que sont ces propositions de résolution et pas sur autre chose, nous sommes très prudents le coeur de notre résolution, c'est de demander au gouvernement de s'engager concrètement dans cette direction, dans l'intérêt 1er des agriculteurs et de l'agriculture française, je vous remercie.

Madame la présidente, monsieur le Ministre, mes chers collègues. à la lecture et à l'écoute des propos de Monsieur Franck Manteaux ai et à la lecture de la proposition de résolution sur la création de paiements pour services environnementaux. Certaines idées peuvent paraître séduisante. Il n'en reste pas moins vrai qu'elles peuvent être aussi très dangereuse pour l'avenir de notre agriculture française. Si je partage totalement l'idée qu'il faut arrêter les stigmatisations car ces stigmatisations ne conduisent qu'à monter les gens les uns contre les autres stigmatiser ne conduit qu'à mépriser les le travail des agriculteurs stigmatiser conduit à créer une réelle psychose chez nos agriculteurs, poussant certains trop souvent à commettre l'irréparable. Nos agriculteurs travaillent plus de 70 heures par semaine et certains éleveurs, 7 jours sur 7, dans une société qui perd petit à petit, le sens de la valeur travail et le goût de l'effort, il se voit sans cesse critiqué de chasseurs de primes de pollueurs ou d'empoisonneurs, cela est insupportable pour eux, la grille bashing semble sans limite, poussé par une démagogie des Moog démagogie verte et passant par des taupes, thème qu'il faudrait abattre tels le glyphosate a supprimé sans études préalables ni méthodes alternatives efficaces tout cela ressemble plus à de l'obscurantisme du progrès.

or notre modèle a su maintenir une agriculture répartis sur la totalité du territoire français et cela même dans des zones où la concurrence mondiale, elle y handicaps naturels aurait pu largement la faire disparaître, car ce modèle français est celui du maintien d'un maximum d'agriculteurs sur une Hervé qu'une politique forte à l'installation et un soutien d'une agriculture familiale, mes chers collègues, cette démagogie n'est plus tenable : nous ne pouvons plus continuer à souffler sur les braises et malheureusement je crains que cette proposition de résolution le fassent une fois de plus, en effet, pourquoi chercher à reconnaître des services rendus à l'environnement par l'agriculture alors que les contribue déjà beaucoup, certes le système alimentaire mondial est responsable d'un tiers des émissions de gaz à effet de serre, par contre, selon l'index de durabilité des systèmes alimentaires, la France occupe depuis 3 ans, la 1ère place du classement des systèmes alimentaires les plus durable au monde, mes chers collègues, contrairement à ce qui est véhiculé, nous sommes déjà exemplaire de plus alors que toutes les craintes d'une diminution importante du budget de la Pac se profile avec le risque de déstabiliser la ferme France pourquoi amplifier cela par une ponction sur le 1er pilier pour financer ces mesures agro-écolo bobo environnementale pourquoi comme dans une course effrénée au concours Lépine de l'idée de laver plus Vert que Vert, mettre sur la table avant les négociations du budget de la Pac, cette résolution mieux à même, mieux à même de négocier l'avenir du budget de la Pac, je ne le crois pas, bien au contraire, ce sera déjà accepté la subsidiarité ce qui conduit à avoir une politique agricole commune, de moins en moins commune et qui accentuera encore les écarts de compétitivité entre notre agriculture française et les autres pays européens concurrents pourquoi vouloir comme il est écrit dans cette résolution : donner l'exemple, alors que nous sommes déjà exemplaire ce texte semble répondre encore à cette minorité d'éternels insatisfaits, qui n'ont pas l'objectivité de reconnaître le progrès de notre agriculture qui a su apporter une alimentation en quantité et en qualité nécessaire alors que partout sur la planète, les pays cherche inlassablement à l'acquérir, méfions-nous, mes chers collègues, l'autonomie alimentaire de la France n'est pas un fait acquis, à cause de condamnation perpétuel doublée d'un manque de lucidité politique, nous ne sommes déjà plus autosuffisants sur certaines productions, la place à des produits d'importation dans nos assiettes sans que personne, et encore moins ses intérêts ces insatisfaits condamne le fait qu'il ne répondent pas aux normes de production à nos normes de production alors, mes chers collègues, j'en appelle à la responsabilité de tous, j'en appelle au bon sens de tous les sens, enfin nos agriculteurs tranquille, arrêtons de vouloir sans cesse leur maîtres des boulets aux pieds, tout en leur demandant de courir un 100 mètres cette profession qui me passionne, en a assez de toutes ces normes de tous ces clichés, laissons-là sans la contrainte sans cesse à exprimer ce qu'elle sait faire de mieux cultiver et élever avec les vicissitudes de la nature pour nourrir dignement son peuple, je ne voterai donc pas cette résolution et je vous appelle à faire de même car je suis agriculteur et pas jardinier de la nature, merci.

Madame la présidente, monsieur le Ministre, mes chers collègues, cette proposition de résolution en faveur de la création de paiements pour services environnementaux Randy par les agriculteurs tient compte à la fois du contexte mouvant et instable que subissent chaque jour les agriculteurs ainsi que la nécessité de chercher de nouveaux outils au service de la protection environnementale ces paiements récompense donc les externalités positives de notre agriculture en faveur de l'environnement ces externalités regroupe les influences directes et positifs du travail agricole, au-delà de l'activité agricole en elles-mêmes, notamment en séquence en séquestrant le CO2 en entretenant les écosystèmes et en même, ce pourrait mener sans des maladies, notre groupe, admet l'intérêt du texte soumis au vote par nos collègues socialistes nous soutenons par ailleurs une vision plus étendue des externalités positives qui inclut non seulement les enjeux de cette proposition, mais également l'ensemble des effets positifs de notre agriculture telle que la création d'emplois, ou encore la contribution les attractivité des espaces ruraux et à développement de la de la sorte, nous nous serions bel et bien, au croisement de 3 problématique majeure de la politique agricole, celle du soutien à la transition environnementale, celle du développement rural et, enfin, et non des moindres, celle d'assurer des revenus décents, issu de l'activité agricole, ainsi il ne faut analyser les politiques mises en oeuvre jusqu'ici pour relever les défis actuels et futurs en matière de santé dans enjeux d'environnement, de lutte contre le changement climatique et protection de la biodiversité et, plus largement, d'adaptation aux nouvelles attentes sociétales et enfin, il nous faut chercher et proposer des pistes vers un modèle agricole permettant de mieux prendre en compte les externalités positives d'une agriculture capable de dégager des revenus viable pour tous les agriculteurs sur ce plan, nous sommes d'accord, la PAC a atteint ses limites et ne parvient pas à endiguer la pauvreté des exploitants agricoles, symbole de ses limites, 30 pour 100 des exploitants avaient un revenu inférieur à 350 euros par mois en 2016 selon la MSA, que la baisse continue de nombre d'agriculteurs, malgré un soutien, un moyen de plus de 30000 euros par agriculteur pour exemple de mesure employée par les pouvoirs publics, le régime de paiement de base aux paiement vers constitue un outil de poids de la PAC pour assurer un niveau de vie équitable aux agriculteurs et représente 30 pourcent de son bus bustier cependant en mars 2018, la Cour des comptes européenne dans un rapport sur l'évaluation du régime de paiement de base conclut que celui-ci fonctionne mais qu'il a un trop faible impact en juin dernier, le Sénat adoptait une résolution européenne pour préserver une pacte forte cette résolution rappelle l'importance de valoriser les externalités positives de l'agriculture, en particulier son potentiel de stockage de carbone au regard des services rendus, tant à l'égard de la société que l'environnement, ce qui devait valoir aux agriculteurs une raie numération même mieux conçus et plus simple des biens publics qu'ils produisent, alors même qu'au début des négociations, la Commission européenne envisage une baisse du budget global de la PAC, le ministère de l'Agriculture, s'est engagé à défendre fermement et sans relâche un budget à la hauteur des défis de que des défis que l'agriculture européenne doit relever des attentes environnementales de la part des agriculteurs et de la population, les attentes économiques des agriculteurs pour bénéficier de meilleurs revenus issus de l'activité et celle des consommateurs qui consomment toujours plus d'aliments issus de l'agriculture biologique nous pousse vers un nouveau modèle économique, social et environnemental à construire un modèle qui favorise la transition écologique du monde agricole et la durabilité des revenus des agriculteurs, c'est pour toutes ces raisons que notre groupe des sénateurs la de la République en marche, regarde avec bienveillance cette proposition de résolution, considérant qu'elle pourrait aller plus loin, nous voterons cependant en faveur de son adoption. Merci, la parole est à madame Cécile Cukierman. Pour 6 minutes. Madame la présidente, monsieur le ministre, mais mes chers collègues, à l'oeuvre à l'heure, pardon, où s'ouvrent les débats sur cette proposition de résolution, la question de l'impact de l'activité agricole sur l'environnement et plus que jamais au coeur des débats politiques et sociaux en France et en Europe, à cet égard la nécessité d'une transition agro-environnementales s'est particulièrement exprimée lors des derniers états généraux de l'alimentation, mais ici, mais aussi lors des débats sur le projet de la loi Egalim ici et à l'Assemblée nationale, ainsi la sécurité alimentaire, la santé publique, le bien-être animal, la préservation des milieux naturels et de la ressource en eau sont aujourd'hui des défis que le monde agricole doit relever mais si la nécessité de transformer en profondeur notre modèle agricole vers une agriculture plus respectueuse de l'environnement est un impératif indiscutable, nous devons y mettre les moyens, c'est d'ailleurs dans ce cadre qu'il faut appréhender les débats sur les paiements pour services environnementaux très en vue au niveau européen dans le cadre de la négociation de la future PAC et dont il est question dans cette proposition de résolution de nos collègues du groupe socialiste, alors que propose-t-elle sur le modèle de ce qui a pu être fait au Costa Rica, elle incite les grandes entreprises agroalimentaires à mettre en oeuvre le principe le principe 0 déforestation il s'agit dans les faits, de rémunérer les agriculteurs qui adapte adopteraient des pratiques favorables à la préservation de l'environnement, ce dispositif reposant sur des contrats qui peuvent impliquer des acteurs privés propriétaire foncier, entreprises, associations et des acteurs publics, cela part donc d'une très bonne intention, mais il faut tout de même noter qu'il existe déjà un mécanisme pouvant être assimilé à un dispositif PSE actuellement en Europe et en France, et même si notre collègue monte G a rappelé la complémentarité qui pouvaient exister entre les mesures agro-environnementales et climatiques de la politique agricole commune et ce PSE, il existe, il n'en demeure pas moins qu'il existe déjà des possibilités d'agir à travers ce que l'on appelle dans ce cas de l'agriculteur s'engage à respecter des pratiques environnementales, précise allant au-delà de la réglementation et en contrepartie, l'administration verse un financement public couvrant les coûts supplémentaires générés par ces pratiques, les pertes de revenus ainsi que les coûts de transaction. Toutefois, les auteurs du texte propose de faire autrement, il ne s'agirait donc plus de compenser des surcoûts ou des manques à gagner, comme c'est le cas avec les dispositifs actuels de de mecs mais de rémunérer une pratique environnementale cela à travers un financement public ou privé, l'idée est séduisante et le de base sur les épée se permet d'interroger la notion de bien commun dans laquelle je classe bien évidemment l'environnement mais il interroge également sur la notion de propriété foncière, quid de la transmission des contrats en cas de cession d'exploitation plus que cela : ce débat pose la question d'un réel accompagnement des agriculteurs dans la transition agro-écologique mais pour séduisant qu'il soit l'épée se pose aussi des questions qui ne semble occulter ou en tout cas peu développée par ce texte, dont nous débattons aujourd'hui comment éviter, en effet, les effets d'aubaine ou les opportunisme l'épée, ce ne sont intéressants que si tout risque de chantage environnementale, c'est-à-dire si vous ne me payaient pas, hé bien je détruirait est écartée et si tous les agriculteurs peuvent potentiellement en bénéficient, de plus, comme le soulignent certains écrits certains otages a réalisation d'épais pourrait entraîner la disparition de pratiques désintéressé, participant à la protection de la nature. à partir du moment où une rémunération pouvait pourraient être envisagées, pourquoi alors ne pas en profiter, il serait peut-être aussi de plus en plus difficile de mettre en place des normes environnementales du fait notamment du principe de contractualisation au détriment finalement d'normes législatives, enfin, il faut être attentif à l'écueil qui voudrait que la protection de l'environnement finissent par constituer l'unique justification de l'intervention publique en agriculture ainsi la question de la correction des défaillances de marché à la base des crises économiques agricoles qui justifie tout autant une intervention, une intervention publique correctrices ne serait plus légitime, ce dernier point est d'autant plus nécessaire vu les propositions qui sont aujourd'hui sur la table des négociations et qui laisse envisager une PAC beaucoup moins commune où les Budgets seraient fortement réduits et où l'on renoncerait à toute politique environnementale ambitieuse et globale, ces contrats peuvent participer à une remise en cause, donc de sa division public de l'environnement et une forme, j'ose le mot de privatisation possible du droit à l'environnement, pour toutes ces raisons, la majorité de notre groupe ne votera pas cette proposition de résolution qui sans garde-fous risque encore de laisser de nombreux agriculteurs en dehors du dispositif, nous pensons au contraire qu'il faut développer une réflexion alternative, cela a été évoqué précédemment, notamment autour du concept de rémunération des externalités positives parce que, bien évidemment, c'est prendre en compte l'environnement c'est prendre aussi la question des avantages sociaux de la place humaine de la question de l'aménagement du temps du territoire et finalement du lien entre territoires ruraux pratiques agricoles et les défis climatiques pour demain le passage d'un modèle intensif à un modèle vertueux doit être à nos yeux, largement soutenu pour autant et je l'ai dit, une majorité de notre groupe ne pense pas que ce soit en passant par Intel dispositifs tels que présentés que cela puisse évoluer et faire avancer les choses telles qu'en tout cas cette proposition et aujourd'hui rédigé, nous nous abstiendrons donc pour la plupart sur cette proposition de résolution, je vous remercie.

Madame la présidente, monsieur le ministre, chers collègues. Pour être rentable d'une exploitation agricole doit-elle être nécessairement négatives sur l'environnement, sur la qualité naître nutritionnelle des produits sur la santé de celles et ceux qui travaillent, la réponse est évidemment non. Avec cette proposition de résolution nous souhaitons faire reconnaître l'action positive que cherche à mener de nombreux agriculteurs, que ce soit pour la santé, pour l'environnement et pour l'aménagement du territoire. Cette reconnaissance doit être doublé, à nos yeux, moral et économique. On n'a jamais tant parlé de l'agriculture, mais on n'en a jamais aussi mal parlé. Les images qui sont associés dans les médias ces dernières années ont très souvent une dimension négative maltraitance animale pesticides scandale alimentaire. Le fossé semble se creuser toujours plus entre la population et ceux qui la nourrissent. Les attentes grandissant de nos concitoyens en matière de préservation de l'environnement et de sécurité alimentaire sont légitimes sont même essentiel, car c'est cette opinion publique qui nous pousse à transformer en profondeur notre modèle agricole. Ce modèle hérité de l'après-guerre a été construit pour répondre à une compris préoccupation unique comment produire suffisamment pour nourrir la population de la génération du baby-boom. Le modèle sur lequel nous devons aller désormais doit répondre à une exigence qualitative et plus seulement quantitative, en effet, qui peut se satisfaire de cette pente qui nous-même. Toujours plus, c'est-à-dire une alimentation à des vitesses saine pour les plus fortunés, bas de gamme pour les plus pauvres personnes. De nombreux agriculteurs n'ont pas attendu le législateur pour améliorer l'efficacité agronomique et environnementales de leurs pratiques. Mais ces actions positives reste trop méconnu, j'allais dire invisible. Dans la création de ces paiements pour services environnementaux nous pouvons redonner de la visibilité à ce qui existe déjà en plus. Cette directes qui existent déjà, comme l'a très bien développé Franck Manteaux, mais au-delà de cette juste reconnaissance symbolique, il vient du Maroc, une dimension beaucoup plus. Terre à terre, améliorer la rémunération des agricultures et des agriculteurs qui font des efforts, parfois des sacrifices au service de l'intérêt général et ainsi en inciter d'autres à les rejoindre. Nous ne pouvons plus laisser seuls nos agriculteurs face à ce dilemme permanent, utiliser des intrants dangereux et polluants dont ils sont les premières victimes ou tirer le diable par la queue, mois après mois, d'autant plus que nous savons tous, l'un n'empêche pas l'autre. Mais trop souvent des agriculteurs qui souhaiteraient sincèrement aller vers des modes de production plus sain en sont dissuadés par les coûts engendrés par une telle conversion il existe bien sûr et vous l'avez été déjà souligné quelques outils pour accompagner c'est c'est transition je pense entre autres mesures agro-environnementales et climatiques vont dans le bon sens mais restent insuffisantes. Pour inciter durablement une modification en profondeur des pratiques, nous devons valoriser de manière permanente les effets positifs de l'Agriculture, sur l'environnement. Nous savons que la politique agricole commune est à un tournant. Elle sera nécessairement impactés par les conséquences d'un Brexit qui n'en finit pas de se conclure. En tant que grande puissance agricole au sein de l'espace européen, la France a une responsabilité particulière pour orienter la prochaine PAC verra un soutien plus affirmé aux bonnes pratiques, nous souhaitons que notre pays aille à la table des négociations avec dans sa besace, des propositions concrètes pour aider mieux si ce n'est plus le monde agricole. Ainsi les PSA représentent plus que jamais une opportunité de concilier différents impératifs. Les agronomes ondées ont d'ores et déjà qu'on. Puis le logiciel du Moselle agricole dans lequel nous devons aller. La rotation des cultures, le travail du sol le travail du sol des herbicides naturels sont autant d'alternatives aux produits chimiques qui a mis de la Terre et les hommes. Il nous propose un modèle non seulement plus respectueux de notre planète, mais aussi qui créera plus d'emplois, avec de meilleures conditions de travail pour nos agriculteurs aussi, nous n'avons pas besoin en tant que législateur d'inventer le modèle agricole de demain, en revanche, il est de notre devoir de tout faire pour le rendre possible. La création de paiements pour services environnementaux rendus par les agriculteurs serait un 1er pas sur cette voie, Intel sujet mérite de dépasser la couverture du nom du qui porte le nom des auteurs et du groupe signataires et de se prononcer sur le contenu de ce livre sans dogmatisme et sans préjugés. C'est pourquoi. Comme mon collègue du plomb car je suis agriculteur et pas jardinier de la nature, je vous invite, chers collègues à voter en faveur de cette proposition de résolution, je vous remercie.

Monsieur le ministre. Mesdames et messieurs les sénateurs, chers collègues, je tiens tout d'abord à saluer l'initiative du groupe socialiste qui nous propose aujourd'hui cette résolution en faveur de la création de paiements pour services environnementaux, ce texte tombe à mon sens, au bon moment à plusieurs titres, les paiements pour services environnementaux suscite des attentes fortes de la part de bon nombre d'agriculteurs, d'associations environnementales et citoyenne, cette attente ces attentes font suite aussi à l'engagement du président de la République que vous avez confirmé, tout récemment, monsieur le ministre, mais des inquiétudes si subsistent sur la mise en oeuvre de cet engagement. Au niveau européen, au vu de l'état actuel des négociations, on peut s'interroger sur l'ambition de cette nouvelle programmation notamment sur le plan de la transition agro-écologique au niveau national, la fin du cofinancement de l'aide au maintien en agriculture biologique, qui était pourtant une forme de PSE nous a envoyé un très mauvais signal. Mais vous n'est, vous n'y étiez pas encore en poste, monsieur le ministre, l'enveloppe de 150 millions sur 3 ans, alloués aux agences de l'eau reste insuffisante, comme le rappelle le texte cette proposition de résolution et donc une occasion de réaffirmer qu'il est essentiel que la France porte une position forte dans les négociations européennes, c'est aussi une occasion de rappeler que le que si la France veut être crédible dans ces négociations européennes, elle se doit de mettre en oeuvre sur son territoire une politique ambitieuse dans ce domaine, il me faut encore une fois le rappeler la réorientation de notre modèle agricole aide d'urgence à l'heure du dérèglement climatique, de l'effondrement de la biodiversité, des attentats à la qualité de l'eau, de l'air des sols mais aussi de la crise des revenus agricoles. le PSE peuvent et doivent, comme le rappelle cette proposition de résolution constituer la base d'un nouveau contrat entre l'agriculture et la société en même temps qu'un outil au service du changement des pratiques agricoles, il faut cependant mettre un contenu précis derrière ce concept dont la définition n'est pas encore stabilisé j'ai co-organisée vendredi dernier ici même au Sénat, un séminaire sur ce sujet, en partenariat avec la plateforme pour une autre PAC cette structure rassemble, il est important, le noter 33 organisations, à la fois des associations et syndicats de producteurs et de et d'agriculteurs des associations environnementales des associations de solidaire d'une solidarité internationale et de citoyens consommateurs leur position sur les pièces recoupe en partie les éléments de cette proposition de résolution mais va plus loin le PSE doivent rémunérer des pratiques concrètes dont l'effet positives sur l'environnement est avérée, il ne doit pas rémunérer une simple imitation d'impact négatif, c'est là le rôle des des outils d'accompagnement au changement de système, comme l'est M. c'est à ce titre, il est essentiel, comme la proposition de résolution le rappelle que la mise en place des PSE ne signifie pas une diminution de l'enveloppe budgétaire des outils d'accompagnement à la transition au regard des éléments qui sont pour moi, ressorti de ce séminaire, cette proposition de résolution reste donc incomplète au niveau budgétaire, la proposition de résolution ne s'engage pas sur la part qui devrait être consacrée au PS pour la plateforme à la avec laquelle on a travaillé, il faudrait, pour être efficace, maître de l'ordre de 40 pourcent du 1er pilier au service de ce dispositif, la plateforme propose également qu'une place soit accordée à l'agriculture biologique dans CPS, en effet, ce mode de production, a des effets positifs avérés sur les écosystèmes le texte semble un peu timide sur ce plan je trouve aussi que cette résolution aurait dû donner des pistes plus concrètes, pour définir des pratiques ambitieuse qui mérite d'être rémunéré, à savoir le captage du carbone via le maintien des prairies permanentes en lien avec l'élevage à l'herbe à linéaire de haies bocages important et la pratique de l'agroforesterie et aussi le maintien d'un couvert végétal permanent et pour moi, évidemment sans utilisations de glyphosate l'allongement des rotations de culture diversifiée à titre d'exemple, la réglementation pratiquée en Suisse, qui nous a été présenté vendredi rendent impossible la monoculture de maïs, un autre exemple de pratique qui s'inscrit également dans la réponse à une attente sociétale forte concerne le paiement pour des pratiques favorables au bien-être animal qui sont d'ailleurs le plus souvent efficace sur le plan de l'environnement, un autre point important, n'a pas été abordé par le texte, la nécessaire simplicité du système : les contrôles packs sont aujourd'hui source d'angoisse pour les agriculteurs qui n'en ont pas besoin une politique efficace doit susciter de la confiance, rappelons aussi Monsieur le Ministre, que nombre d'aides PAC n'ont pas encore été payés notamment les aides bio et lait, M. A. C, c'est aussi de l'héritage que vous faites l'un, par contre, il y a urgence à agir, malgré ses limites, que je viens de souligner ce texte vient au bon moment pour pousser une impulsion sur le sujet s'il pointe à ce titre, l'importance de la mobilisation des syndicats agricoles des collectivités du gouvernement, je souhaite ajouter à cette liste les citoyens et les ONG qui auront tous leur rôle pour peser sur les nécessaires changements de cap, enfin, je voudrais en conclusion, rappelait l'idée avancée par Nicolas Hulot, que l'on n'a pas tout à fait oublier. Pour réussir une politique agricole et alimentaire et alimentaire aboutit un copilotage de la PAC entre les ministères de l'Agriculture et de la transition écologique et solidaire serait une absolue nécessité alors pour ma part je voterai positivement ce texte, la majorité de mon groupe, parce que dans notre groupe, il y a toujours liberté de vote et c'est très respectable, la majorité des membres du groupe se positionnera en fonction de, de nos échanges, je vous remercie de votre attention. Pour minute chers pour 10 minutes chers collègues. Madame la présidente, monsieur le Ministre, mes chers collègues. Nous avons ce jour un débat intéressant sur le paiement des services rendus pour des prestations environnementales. Je voudrais vous dire que firent le constat de départ, je crois que nous n'avons pas de mal, dans ces Micic là nous accorder tant les difficultés de l'agriculture française. Sont présents et ne sont pas réglé. J'ai eu l'occasion séjour dernier de m'entretenir avec un certain nombre d'agriculteurs de représentants syndicaux. Pour parler avec eux. De cette proposition de résolution. Ils m'ont presque ri au nez. En me disant. Il y a déjà depuis un certain nombre d'années des mesures. Proche de ce qui est contenu dans cette révolution. Et aujourd'hui, tous les agriculteurs volontaires, tous ceux qui font le plus d'efforts vers une agriculture qui s'engage vers une révolution environnementale, tout cela n'ont toujours pas perçu ce qui est leur est dû et par l'Europe et par l'État français. Et ils m'ont dit : mais vous avez vraiment du temps à perdre et je crois que vous vous moquez un peu de nous. On fait le travail, on s'investit depuis 30 ans, pour certains, on avance sur les technologies qui permettent déjà aujourd'hui de réduire de 50 pourcent par rapport à l'agriculture conventionnelle, jeudi, de réduire de 50 pourcent l'usage de tous les pesticides confondus. Et ces mêmes agriculteurs attendent depuis 2 ans. Hein, d'être payés pour le travail rendu. De d'avoir un minimum de reconnaissance de la nation et de tous et aujourd'hui rajouter. Une proposition de résolution qui Ferte louable et sur lequel on ne discute même pas, ils nous disent oui, à terme, c'est ceux là où il faut arriver mais avant, il va falloir commencer à avoir un minimum de reconnaissance pour l'agriculture, qui fait des efforts énormes pour feu qui travaille en profondeur et non pas de leur salon qui ne sont pas des donneurs de leçons, mais qui font ce travail au quotidien pour faire avancer l'agriculture qui n'ont ni reconnaissance financière ni reconnaissance morale de la nation, je crois qu'aujourd'hui ce qu'attendent les agriculteurs fait n'est pas vu une énième loi une énième résolutions. Et une résolution en plus petit,

de l'utilisation des règles alors qu'aujourd'hui cette complexité même fait les ordinateurs du ministère de l'Agriculture et c'est fait complexité qui est en cause. Je crois qu'à un moment. Dans cette hémicycle au ministère dans les milieux environnementaux, il va falloir prendre le temps aussi d'écouter un peu les agriculteurs de voir les agriculteurs qui font les efforts de voir les agriculteurs qui ont acquise des connaissances environnementales depuis 30 ans d'expérience. Et des agriculteurs qui ne sont même pas écouté, j'entendais un collègue tout à l'heure qui disait tout l'avenir. D'une technique sous couvert végétal. Et c'est même va agriculteurs qui disent : mais oui encore 4, 5, 10 ans, on aura peut-être plus besoin de pesticides mais aujourd'hui si vous nous enlevez le glyphosate, c'est comme si vous enlevez le cuivre ou Lachaud en agriculture biologique fait face à la réalité que les utopistes ni et ne veulent pas reconnaître. Et je crois qu'aujourd'hui il faut Veyrat véritablement. Simplifier les procédures, Robuchon, disait le même de la cuisine, c'est la simplicité du plat. Eh bien je crois que le summum d'une réglementation environnementale pour l'agriculture, ce sera la simplicité des mesures envisagées et non pas une complexité que. Vous portez tous les uns et les autres, moi je vois avec beaucoup de perplexité de douleur, de voir comment dans les hémicycles. On s'acharne quelquefois à complexifier des lois qui, au départ, partent d'un bon état d'esprit et partent d'une bonne simplicité. Je crois qu'aujourd'hui. Les agriculteurs ont besoin d'avoir les mesures rapides, efficaces qui bon leur permettent de travailler et de gagner leur vie, c'est l'urgence absolue et autre chose et pris un peu comme une provocation. Ensuite, effectivement, ils sont d'accord pour une agriculture. Européenne qui portera ses mesures environnementales, mais qui portera une agriculture européenne vers le haut, et qui ne pénalisera pas l'agriculture française, avoir des mesures franco-françaises s'imaginait qu'on peut laver plus blanc que blanc, nous Français, qu'on est les meilleurs du monde dans les lois, c'est une utopie ça condamne notre agriculture à disparaître, c'est comme s'imaginer qu'on peut avoir une agriculture pastorale. Avec un élevage de loup bien dressés pour venir manger les moutons, tous les jours, on ne peut pas avoir la chèvre et le chou, dans le même parc et il faut un minimum écoutez et le travaux d'des agriculteurs qui s'investissent énormément et prendre le temps aussi un peu d'écouter les scientifiques, j'ai aussi l'occasion d'entendre Des chercheurs de l'INRA. Qui vous dit-il, mais pour les loups on est fou. Les pays dans le monde, femme Les Loups connaissent les loups. ça va avoir des loups dans leur espace, y compris agricoles mais vos méthodes à la française, elles ne tiennent pas debout. Allez voir fleuve qui se passe dans les autres pays du monde, et vous verrez que les loups en nombre raisonnables peuvent vivre au niveau en même temps qu'une agriculture pastorale en France on ne fait pas faire parce qu'on fit machine qu'il suffit de légiférer pour que tout aille bien. Donc, je vous propose mes chers collègues. D'attendre pour cette révolution. Je proposerai à mes collègues, Union centriste de ne pas voter cette résolution. Parce qu'elle arrive trop tôt, réglons aujourd'hui nos problèmes portant une résolution au moment de la réforme de la politique agricole commune, battons-nous pour une agriculture européenne mais ne sacrifions pas l'agriculture française au bénéfice de quelques idéologies. Pour 6 minutes. Madame la présidente, monsieur le Ministre, mes chers collègues, l'agriculture française et européenne s'devra répondre dans les prochaines années, les défis majeurs une demande alimentaire en hausse, plus diversifié et plus exigeante en qualité : une concurrence internationale accrue et un contexte économique instable, la révision de la PAC, une pression foncière constante, la recherche d'une contribution positive à la préservation des territoires et des ressources naturelles des réformes ont déjà été menées, d'autres sont en cours au niveau européen et national, il nous faudra être innovant, plus que jamais sur les réponses à apporter pour satisfaire les attentes de la société et pour soutenir nos agriculteurs cette résolution pose donc une question fondamentale sur l'avenir de notre écriture son rôle, son évolution, la meilleure façon pour les pouvoirs publics de la soutenir en répondant aux nouveaux défis sociétaux, environnementaux et économiques, la création de paiements pour services environnementaux afin de valoriser les externalités positives semble aller dans le bon sens, les agriculteurs sont les premiers utilisateurs de territoire, il joue un rôle fondamental dans la gestion de nos paysages pour la préservation de la biodiversité dans la lutte contre le changement climatique, or force est de constater que ces services rendus ces actions du quotidien, dont l'impact environnemental est indéniable sont trop rarement prise en compte et rémunérés à leur juste valeur l'État la timidement évoqué dans son plan biodiversité, tout comme les régions dans leur soutien à l'agriculture biologique, par exemple, cela reste beaucoup trop restreint les externalités positives des agriculteurs sont beaucoup plus importantes et variées qu'il n'y paraît, l'agriculture aménage et façonne le territoire, elle se nourrit des richesses naturelles de par son importance, l'activité agricole influe directement sur l'ensemble des enjeux environnementaux elle tellement majeur des paysages et influe donc sur cette biodiversité les sols et la ressource en eau, elle est également au coeur de l'enjeu du réchauffement climatique et représente donc un potentiel de production d'énergie renouvelable, intéressant, il est aujourd'hui fondamental d'impliquer et de faire connaître l'agriculture dans les enjeux d'aménagement du territoire et de préservation de l'environnement au travers un soutien plus pertinent parmi les territoires agricoles les plus intéressants en terme de biodiversité je voulais évoquer avec vous, les zones humides, des marais littoraux les vallées alluviales, les zones humides et des tourbières, signataire de la Convention de Ramsar en 1971 la France a ratifié ce traité en 1986 il a pour mission la conservation et l'étude sur rationnelle des zones humides par des actions locales, régionales et nationales, à ce jour 48 sites s'étendent en France sur une superficie de plus de 3,6 millions d'hectares en métropole et en outre-mer ces milieux habite près de 45 pourcent des espèces menacées en Flandre métropolitaine et pourtant, malgré plusieurs plans nationaux successifs leur disparition et leur dégradation se poursuivent, menace de dégradation, voire de disparition intensification agricole endiguement des cours d'eau urbanisation ou simplement abandon j'ai dans ma grande région. Plusieurs sites Ramsar le marais Audomarois et l'un d'entre eux, il abrite 1050 hectares de prairies humides 436 hectares de Terres maraîchères et 171 hectares de roselières on y produit 50 variétés de légumes différents comme toutes zones humides le marais Audomarois est un atout pour ma région et subit de nombreuses pressions liées aux activités humaines, il est sans doute le témoin rare d'un équilibre réussi bien fragile entre la nature et des activités humaines actuellement les aides octroyées pour les zones humides ne diffère que très peu des aides classiques appliquée à l'échelon national et sont loin d'être suffisante pour prendre en compte les spécificités de cette activité agricole et ses bénéfices pour la société, les mesures agro-environnementales ont simplement ralenti les dégradations subies mais demeurent insuffisantes au vu des difficultés réelles et souvent croissante en zone limite la richesse de ses milieux de transition, les inscrits comme des leviers primordiaux dans la lutte contre les changements climatiques et l'adaptation au réchauffement et en conséquence dans les nouvelles modalités encore à inventer d'aménagement de territoire, fondée sur des solutions pour la nature, ces milieux sont au coeur des efforts que l'on faire pour assurer à nos concitoyens une meilleure santé, meilleure qualité de vie, un meilleur accès à l'eau, ils peuvent permettre de développer une économie verte et de créer des emplois, je voudrais également dire un mot monsieur lui d'illustres sur le système hydraulique des voix tringle du Nord et du Pas-de-Calais, autre zone considérée humide, il permet de maintenir hors d'eau à un territoire de 900 kilomètres carrés situés plus bas que le niveau de la mer est en grande partie, entretenu par les agriculteurs qui pourraient percevoir des paiements pour services environnementaux pour cela, cette zone pourrait d'ailleurs faire l'objet d'un traitement d'une considération distinctif créer des paiements pour services environnementaux pour toutes ces hommes dont les polders reviendrait à reconnaître leur grande plus-Value et mettre en avant le travail mené au quotidien parce qu'entretiennent et les préserve les agriculteurs. Et en ce qui me concerne. Gare ces considérations, cela s'inscrit parfaitement dans les travaux menés actuellement par mon collègue de Jérôme Bignon, dans le cadre de la mission parlementaire que lui a confiée le 1er ministre les zones humides et dont les conclusions sont vivement attendues pour les zones précitées et dont les charges strict de structures sont supérieurs à la moyenne nationale. Globalement, et avec discernement, le groupe, les indépendants, soutient cette révolution. Visant à la fois le développement de nouvelles sources de revenus pour nos agriculteurs tout en préservant l'environnement et nos ressources naturelles.

Madame la présidente, monsieur le ministre, chers collègues. Victimes des changements climatiques nos agriculteurs n'ont pas attendu l'État ou encore l'Union européenne pour se soucie guère de leurs matières premières, leurs Terres leur passion. En région méditerranéenne et les incendies, constituent un risque important et mon collègue en a déjà parlé la gestion par pastorale et des milieux âme broussailles et est alors un bel outil afin de lutter efficacement contre les départs de feu. Autre exemple, l'irrigation traditionnelle permet de préserver nos nappes phréatiques et les agriculteurs des Bouches-du-Rhône un savent quelque chose, un effet nous agriculteurs utilisent l'eau du Rhône et de la Durance grâce aux barrage construit dans les années 50 et aux nombreux canaux ces 2 systèmes dits d'irrigation gravitaire ou par submersion, bref les initiatives sont là et portent leurs fruits, elle ne les porte pas au nom d'une nuit de théologie, mais au nom du bon sens, le bon sens paysan, le département des Bouches-du-Rhône est le 1er département français, Anne, agriculture biologique, ce qui marque une attention particulière à l'écosystème. Une résolution par toujours d'une bonne intention, heureusement, mais elle peut aussi crimes décrédibilisé lorsqu'on me propose d'habiller Paul je me demande toujours qui sera Pierre. souvent dans cet hémicycle, nous rappelant à quel point nous devons être vigilants à ne pas créer des usines agace et à rester pragmatique. Nos agriculteurs nous le disent : ils ne veulent pas d'aide et veulent vivre de leur travail, ils sont toujours enclin à préserver nos ressources puisque je le rappelle, elles sont leurs matières premières pour cela, il faut cependant des alternatives. Marchandises et des services environnementaux rendus par les agriculteurs posent également des questions d'ordre philosophique, finalement c'est dire merci de respecter l'environnement et pour cela on va vous rémunérer, cela voudrait dire aussi que, par défaut, un agriculteur ne souhaite pas préserver l'environnement sur le comment, il y a de nombreuses questions si un exploitant souhaite contractualiser avec une collectivité pour services environnementaux, cela pose la question des marchés publics, quels critères pour établir un juste prix qui pour contrôler comment contrôler. Peut-on parler d'obligation de résultat lorsqu'on dépend d'aléas climatiques. Ce que certains appellent les externalités positives doivent devenir la norme sanctionnant plutôt les externalités positives. Qui doivent devenir la norme sanctionnant plutôt les négative car les alternatives existent et pour que c'est alternatives existent concentrons nous concentrons nos moyens dans la recherche et dans l'innovation, nous y croyons pour l'agriculture de demain en conclusion si l'enfer est pavé de bonnes adaptations : attention, ne faisons pas de notre droit un enfer pour nos agriculteurs. La parole est à monsieur Henri Cabanel pour 5 minutes. Madame la présidente, monsieur le ministre, chers collègues, dans l'Hérault, autour de Montpellier, dans le milieu urbain, un automobiliste sur 10 avaient un gilet jaune. Sur le pare-brise à Béziers dans le rural, 9 sur 10, il faut parcourir la France pour comprendre ce clivage qui s'est crevé entre qui s'est creusé, paupérisé abandonné quand on vit là je m'village rural qui est devenu un village dortoir qui a perdu son âme tout autant que son identité, on comprend, on comprend cette fracture qui s'est faite lentement, sournoisement, c'est un bruit, un climat, les populations, je suis inquiet vraiment inquiet de la méconnaissance de cette mutation de nos villages et de la non-compréhension des âges, les âges socio-économiques et environnementaux et évidemment politique, puisque c'est dans ces villages ruraux que la montée de l'extrême droite est la plus forte et la plus c'est pourquoi je prends une vraie complémentarité entre l'urbain et le rural et pas seulement de bonnes intentions, teinté de Kunduz Kohndo au-delà des réformes sociales et fiscales qu'il faut engager avec courage pour répondre à cet appel au secours, il faut d'abord concentrer les efforts sur les populations périphérie réconcilier les citoyens de l'urbain avec ceux du rural passera par une vraie prise de conscience par les urbains de la plus-Value de territoires ruraux pour l'environnement, les paiements pour services samedi Romain environnementaux un sont un des outils cette proposition de résolution mettent en exergue cet outil né dans les années 1990 mais jamais développé, on peut dire, comme notre collègue lourd que c'est peut-être trop tôt, mais cela fait déjà 30 ans Danone différentes auditions de l'INRA à la FNSEA, les témoignages ont montré que beaucoup Young travailler ça jamais trouvé de solutions, les agriculteurs français ont compris depuis des années, les mutations auxquelles ils étaient confrontés, fragments de projet, a souligné, mais il faut le répéter, changement climatique, qui génère une augmentation des risques et stabilité des revenus, crise des vocations, le tout attisé par une pression sociétale et sur fond d'Agay bashing intolérable car il est facile de critiquer certaines pratiques, il est primordial de souligner la volonté de beaucoup d'agriculteurs qui se sont engagés dans une agriculture durable si les agents sont évidemment les modalités sont plus complexes : 1 septembre 2017 votre ministère a eu les résultats d'une étude menée par le Centre d'étude et de prospective et par horaires de brèches pour porter un regard croisé sur les mesures agro-environnementales et l'épaisse. Le service environnemental est défini dans l'étude, comme je cite un système transparent pour une fourmi une fourniture additionnelle de service ami environnementaux à à travers des paiements conditionnels à des fournisseurs volontaire, mon cher collègue, Laurent du plan du plan volontaire et non obligatoire depuis 2017 si l'AS radio les PSE à un sont au même stade, celui du nos convergences positives mais sans concrétisation car plusieurs questions se posent : le ciblage des agriculteurs, les critères de paiement, les montagnes, les méthodes d'évaluation, nous avons conscience des difficultés liées à ces problématiques difficultés techniques tout autant que politique, car ce sont bien des choix politiques qui donneront une vraie impulsion au PS

mais il nullement question de superposer une norme à des contraintes à d'autres normes et contrainte, non, il s'agit de donner la possibilité à des agriculteurs qui sont persuadés du bien-fondé pour l'environnement, de nouveaux modes de production, d'être rémunérés pour leurs voix pour leurs l'se repose sur une degré d'acceptabilité essentiel pour fixer le montant à payer aux agriculteurs qu'il faut identifier le coût d'opportunité c'est-à-dire évaluer notamment la prise de risque pour le changement de système de production, il faudra ajuster le ciblage des mesures aux un jeune du territoire définir l'échelle les parties prenantes, le taux de paiement, Ray Lema incitatif je veux espérer que nos collègues sceptiques comme droit de notre volonté d'apporter un revenu supplémentaire aux agriculteurs qui font ce choix vertueux ceci : ceux-ci doivent être réellement encouragé, soutenu, si c'est un message d'espoir et d'encouragement évident adressée à la filière cela est également un message fort adressé aux populations urbaines, l'environnement, les paysages, l'effort les les sentiers. Dont elle bénéficie gratuitement à un prix, il est le fruit de prospection collective, celle des pouvoirs publics, mais aussi celle de personnes privées, le plus souvent des agriculteurs tant décrié, qui l'a le plus grand anonymat y participent les bergers par exemple ou les milieux lutte contre les incendies avec leurs gestes locaux du quotidien écobuage le brûlage évidemment le pastoralisme, qui, par exemple, serait une solution pour les territoires sorti des Laëtitia chaîne comme ceux du Gers ou de l'Aude n'entre mission de résolution, vous l'avez compris appelle donc l'État à mettre en oeuvre dès maintenant avec l'ensemble des parties prenantes, un cadre incitatif et de mesures concrètes pour développer les PSE dans notre territoire, beaucoup d'agriculteurs, ils sont prêts, merci.

Madame la présidente, monsieur le Ministre, mes chers collègues, la proposition de résolution déposée par nos collègues sénateurs vise à créer des paiements pour services environnementaux rendus par les agriculteurs. Cette proposition sera un nouvel outil d'aide aux agriculteurs pour créer des nouvelles ressources financières pour les aider à faire face à l'instabilité des revenus et pour limiter la crise des vocations. Cette aide serait en échange versés pour des services rendus, pour l'environnement et seraient complémentaires on magique des mesures agro-environnementales et climatiques, mis en place en 2015. Avant toute chose. J'aimerais rappeler l'objectif recherché lors de la création des en 2015, les mecs qui ont été créés et financés par le fonds européen Feder et géré par un pacte, région, État et professions, l'objectif de ces fonds était de développer des nouvelles pratiques agricoles combinant des performances économiques et environnementales préserver la qualité de l'eau de biodiversité des sols et de lutter contre les changements climatiques. Il existe plusieurs types de mec, en fonction des exploitations par secteur et en fonction de l'environnement, les mayas les EMA et grande culture pour pouvoir en bénéficier, les agriculteurs ont pris l'engagement de diversifier leurs à seulement et d'augmenter la durée des rotations et de réduire les intrants produits azotés phytosanitaires, les mecs des surfaces pastoral qui ont eu pour objectif d'aider financièrement des agriculteurs pour qu'il maintienne le pâturage et les fauche derme dans les milieux semi-naturels ainsi nous améliorons nous améliorerons la qualité de l'eau, nous luttons contre l'érosion des sols et préserver en la biodiversité. Les mecs polyculture élevage qui visait à interdire le retournement des prix des prairies naturelles pour diminuer la part de maïs consommatrice d'eau, limiter l'achat de concentrer pour revenir en autonomie alimentaire et assurer la reprise et le maintien de ces exploitations dans des zones spécifiques. Puis les mecs pour l'aide à la conversion au au maintien de l'agriculture biologique, les mecs ont réellement été créé. Pour avoir des effets positifs sur les écosystèmes, avec une obligation de résultat. Elles ont été comprises par les agriculteurs parce qu'elles vont vers une agriculture raisonnée et de qualité, l'agriculture que recherchent de plus en plus le consommateur mais était trop bien comprise puisqu'en février 2017, un article de La France Agricole nous alerter sur les chèques en blanc signés dans le cadre des mecs. En effet, le fonds Feder alloués pour la période 2015, a du même 2020 a été épuisées dès la fin 2016 des acomptes ont été versées, mais les soldats engagés étaient ou sont versés avec 3 ans de retard déjà que les dossiers étaient relativement compliqués à remplir pour l'exploitant agricole qui avaient souvent recours à des organismes extérieurs et donc des frais. De plus, pour justifier les retards de paiement, les agriculteurs ont voulu le sentiment que les contrôles étaient de plus en plus régulier de plus en plus sévères, 3 ans pour toucher ces sommes avec des crises du marché agricole en plein en pleine plein plein moment les agriculteurs se voyaient appliquer des majorations sur des paiements tardifs de la MSA qui parfois dépasser l'aide attendue et promise d'un côté l'État par le biais de la MSA reproché à l'agriculture, l'agriculteur de ne pas régler ses factures à temps, alors que ce dernier attendait de l'État, les aides promises. Les mecs ont donc perdu la confiance des agriculteurs et nous pouvons regretter parce que les Taïwanais, principal responsable. Alors pourquoi créer une nouvelle aide avec le même objet, J'en reviens maintenant sur les fesses, nos collègues pro-base propose de régler des prestations aux agriculteurs pour services rendus, avec une obligation de résultat, contrairement aux qui, pour eux, ont une obligation de moyens et non de résultats, ils écrivent que les règles ne doivent pas être rigide qu'elles doivent être adaptables, les aides doivent être attribués suivant des critères spécifiques est proportionnel aux bénéfices qu'il génère pour l'environnement. Autant cela peut se concevoir pour la source de l'entreprise, Vittel, Perrier, qui a été cité en exemple l'entreprise en effet a dû calculer ses pertes si la source était pollué pendant une période de 6 mois. Autant, cela me paraît impossible à calculer pour les sources d'eau potable de nos communes qui ne font pas de profits. Autre exemple : l'obligation de résultat, si en montagne, nous n'avons plus d'agriculteurs, nous pouvons craindre la reprise de la végétation et des moyens développés pour assurer l'entretien. Bref, cette disposition me paraît bien compliqué à mettre en place à l'échelle nationale et dans un souci d'équité des bénéficiaires de la profession. Et nous n'avons pas de réelles réponse sur ce point dans la proposition qui est faite de plus nous pouvons craindre un changement de vocation des agriculteurs, je m'explique : supposons que nous arrivions à estimer les risques en cas de pollution de l'eau dans les différents syndicats ou le match, le coût d'entretien des espaces montagnards signa plus agriculteurs que ces montants soient aujourd'hui supportés par des fonds européens par le biais des puis qu'au bout de 5 ans, nous ayons le même exercice les fonds cesse au profit d'un autre système, nous pouvons aucun que des exploitants réclament aux différents organismes syndicats d'eau communes etc le remboursement des sommes porté alors par l'Europe. Je suis convaincu que les agriculteurs ne veulent pas devenir des salariés d'État, il va vivre de reproduction et avoir des exploitations rentables.

la parole est à monsieur Didier Guillaume, ministre de l'Agriculture et de l'alimentation. Madame Madame la présidente, mesdames et messieurs les sénateurs et sénatrices je voudrais d'abord vous dire qu'aujourd'hui est un grand jour, puisque ce matin en conseil des ministres nous avons validé les ordonnances qui vont, espérons-le, permettre une meilleure répartition de la valeur pour nos agriculteurs qui vont encadrer les les promotions fait dans les grandes surfaces et qui sont un D point supplémentaire pour essayer de faire en sorte

je voudrais à ce moment de mon propos, saluer l'initiative qui a été prise par Monsieur Moto G et ses collègues pour cette proposition de résolution n'est pas une PPL je lui proposition de résolution, c'est un acte qui va être posée, souhaitons-le, afin de mettre en lumière l'importance du lien entre agriculture et environnement et vous l'avez tous signalés sur tous les bancs, que les agriculteurs étaient en avance qu'il savait ce que c'était que défendre l'environnement, protéger l'environnement, oui, ils le font tous, alors, n'ayons pas peur, ne soyons pas frileux et si on de tracer des perspectives et de faire en sorte que nous marquions non pas dans une loi qui va avoir des effets immédiats mais dans un texte que la représentation nationale est favorable et indique clairement face à la population face à celles et ceux qui parfois font de l'agri-bashing que l'agriculture et l'environnement sont intimement liés et sont définitivement lié parce que les agriculteurs le veulent, parce que la population le volet parce que de toute façon, si on voulait être pessimiste, il n'y a pas le choix, mais c'est pas du pessimisme qu'il faut, c'est de l'optimisme et dans cet optimisme, les agriculteurs ont fait leur mue et en fait, leur but dans les dans les transitions, c'est la raison pour laquelle le gouvernement est favorable à cette proposition de résolution qui correspond aux orientations voulues par par mon ministère les objectifs que j'ai déjà présenté ici à à, à plusieurs reprises, je viens de le dire, garantit un revenu aux agriculteurs ça peut y contribuer, évidemment, tous les agriculteurs veulent vivre de leur travail de leurs revenus, évidemment, mais enfin heureusement qu'elle la PAC heureusement qu'elle les aide parce que c'est ce qui permet malgré tout de tenir et parfois difficilement la tête hors de l'eau, parce qu'il faut protéger accompagner des agriculteurs compte l'agri-bashing oui sans cesse trop de campagne sont menées compte l'agriculture contre les agriculteurs et cette lutte contre la grippe bashing, nous devons en être, nous les les fervents promoteurs en tout cas à mon poste et le gouvernement et là sans cesse pour faire le bouclier entre l'agri-bashing et les agriculteurs et puis c'est aussi évidemment réussir la transition agro-écologique, c'est tellement évident de que cette transition écologique est irréversible, elle aussi, et que les agriculteurs sont tout entier parti alors certains plus vite que d'autres, d'autres en soit choisit la voie du bio, d'autres de la agriculture raisonnée, d'autres d'une agriculture qui utilise moins de pesticides, moins d'eau, c'est le cas de tous, l'agriculteur de de France et c'est la raison pour laquelle, moi jamais je ne m'opposer ces agriculture et ses agriculteurs mais les uns et les autres avancent à leur rythme, certains dans certaines régions, c'est plus facile que d'autres, dans certaines filières et agriculture, c'est plus facile que d'autres, mais il n'empêche que je ne connais pas, aujourd'hui, un agriculteur qui ne veut pas aller dans cette direction, un agriculteur qui met des à des intrants dans dans le sol pour polluer un agriculteur qui veut abîmer l'environnement non parce qu'ils vivent les pieds dans la terre et ils vivent au milieu de de leurs champs. ces attaques incessantes vis-à-vis des agriculteurs sont vraiment je vous le dis insupportable et donc c'est très proposition de résolution s'inscrit dans les orientations que nous pouvons tous avoir et que nous voulons pour notre agriculture, les services environnementaux rendus par des agriculteurs et promouvoir leur mise en oeuvre, je vous l'ai dit je soutiens cette cette démarche l'épée à ce même si de nombreux points doivent encore être précisées j'en dirais quelques-uns, il y aura d'autres, d'autres débats CPS, ce sont un outil innovant pour réussir la transition agro-écologique de notre. Il faut pas le voir comme une contrainte, pas du tout, ce n'est pas une contrainte supplémentaire, il y a 0 contrainte supplémentaire dans les PS, simplement c'est ça fait partie du du dispositif des dispositifs que nous avons pour qui sont eux incitatif et qui peuvent aider nos nos agriculteurs, ils permettent de reconnaître et de valoriser les actions des agriculteurs en matière d'aménagement du territoire, qui pourrait être contraint de d'entretien des paysages, c'est le cas bien sûr des agriculteurs ne sont pas des jardiniers, des paysages qui sont des agriculteurs, des éleveurs, des des arboriculteurs etc reconnaissons aussi que les agriculteurs sont ceux qui entretiennent nos prairies ceux qui entretiennent nos paysages ceux qui entretiennent au. Nos territoires et sur lesquels les, les, les urbains, M. venir se promener à venir faire du tourisme et il faut jamais oublier cela et je veux remercier les agriculteurs pour pour se faire aussi, il faut cependant aller plus loin et les les PSE peuvent nous y aider, sans stigmatiser mais en accompagnant et en reconnaissant l'engagement de ces agriculteurs accompagné et valorisé plus que stigmatiser, c'est vraiment le sens de votre proposition et c'est le sens des DPS, qui peuvent aussi, disons-le, garantir un revenu plus juste pour les agriculteurs, tous travaillaient service méritant salaire la rémunération de cette approche vertueuse pour l'environnement, peut-être tout à la fois portée par des instruments de politique publique, comme par le marché, il ne faut pas oublier l'un ni l'autre, à la fois le public est à la fois le privé, je pense en particulier à l'agriculture biologique est tout à la fois portée par une politique publique et par une meilleure valorisation des des produits par le par mais au-delà de ce soutien de de principe il faut encore levé plusieurs interrogations concernant leur leur mise en oeuvre le colloque qui a été organisée vendredi dernier : je veux saluer notre collègue le sénateur Joël Labbé, qui a organisé ce ce couac a fourni un certain nombres de pistes pour apporter une traduction politique concrète, mais c'est une Pierre, là encore, un édifice qu'il faut bâtir et jouer vraiment vous remercier et vous saluer monsieur l'abbé pour le travail que vous faites dans ce domaine en général n'est particulièrement pour ce colloque, j'entends votre demande de soutien qui rémunérer les résultats et non les moyens mis en oeuvre, j'en comprends la logique, il existe d'ailleurs aujourd'hui des mesures agro-environnementales et climatiques, les mecs, vous l'avez évoqué basée sur une logique de résultat Ne sont pas des mesures de moyen pur et je veux vous alerter malgré tout sur la demande de généralisation de cette logique car les résultats en matière d'environnement et d'action climatique ne sont généralement pas immédiat et souvent complexes à mesure et c'est la raison pour laquelle cette partie-là de votre texte mérite d'être d'être encore travailler et et précisé mais je voudrais revenir parce que. Plusieurs d'entre vous ont évoqué le versement des aides, notamment des aides bio tout à l'heure, ça a été fait par plusieurs, plusieurs sénateurs, je veux vous vous dire qu'à l'heure qu'il est pour 2016 99 pourcent des aides sont payés et il reste à verser 100 millions d'euros sur 9 milliards 200 millions et que pour 2017 98 pourcent des aides sont payés à l'heure où nous parlons, il reste à payer 150 millions sur 9,2 milliards d'euros. C'est trop, mais je ne peux pas laisser dire et l'État a été défaillant et la SPA a été défaillante, je l'ai dit à cette tribune, je le dis à tribune de l'Assemblée nationale, mais là encore, je ne peux pas dire que les agriculteurs n'ont pas été payés. Tous ne l'ont pas été impôts il reste 1 pourcent c'est trop, peut-être 1 pourcent mais 99 pourcent l'a été et je voulais quand même le le le le préciser, c'est beaucoup trop tard, 3 ans, mais nous l'avons tous constaté, nous l'avons tous tous dit évidemment c'est anormal, c'est pour ça que j'ai demandé de hâter le pas 2016 et 2017 seront payés en début d'année 2019, nous reprendrons le rythme du paiement avec un an après, à une à ne plus donc le PS ne doivent pas être une nouvelle usine à gaz, je le disais à l'instant par rapport aux propositions que vous pouvez faire trouver des indicateurs de résultats qui soit pertinent et simple à instrumentaliser à contrôler aujourd'hui nous ne sommes pas arrivés au but et ça peut s'apparenter à une usine à gaz, c'est pour ça que le travail doit encore se poursuivre, parce que si vous avez l'intention et si nous voulons mettre en place et PSE alors qu'il faut qu'il soit fluide qu'il voient ce qu'il soit simple, qu'il soit compris compréhensibles et qu'il soit accessible au plus grand nombre nous adjudant donc également dans un cadre réglementaire contraint, je le, je le disais, et que cela soit dans le cas de la PAC ou hors hors Pack mais concernant la future PAC : la France soutient une PAC qui porte une vraie ambition environnementale, tout en donnant au secteur agricole, les moyens de réaliser cette transition écologique comme vous l'avez très bien dit, je pense que les pièces doivent s'inscrire dans le cadre national, mais évidemment, dans le cadre européen à monsieur le web à l'heure, qui parlait de simplification, je suis entièrement d'accord, et j'espère avoir le soutien de toute le Sénat lorsque pour la future PAC je vais enclencher un travail de simplification et je ne céderai pas je n'arrêterai pas 9000 critères pourparlers pour payer des aides c'est inacceptable 9000 critères, donc j'espère que la simplification, il n'y aura pas toujours une bonne raison pour faire rentrer une région un territoire une filière un secteur parce que si on veut simplifier, alors il faut simplifier et bien souvent quand la plante, la France veut simplifier ça se transforme en une simplification qui est complexe, donc j'espère que tout le monde sera là, et j'aurai besoin de tout le de tout le Sénat pour pour faire cela et donc c'est la raison pour laquelle, dans le cas de ce que vous souhaitez nous sommes, nous soutenons l'architecture qui est proposée par la Commission européenne, dans le cas de la de la future PAC car elle permet de rémunérer à travers le soutien Direct, je veux le redire, les agriculteurs qui en ont encore besoin et je veux l'assumer,

être obligatoire pour les États-membres et volontaire, aujourd'hui, la difficulté c'est que si nous partons uniquement à un ou 2 États et que c'est pas sur l'ensemble de sur l'ensemble de l'Europe, alors il y aura encore des distorsions qui risque de nouveau revenir en en en figure ce dispositif devra donc permettent de rémunérer sur une base incitative et sur une base forfaitaire du Dupont donc des évolutions votre texte ces évolutions ne seront possibles que si elle dispose d'eau aussi bien au niveau de la PAC en matière national d'un budget suffisant, la France est au début des négociations de la PAC, vous le savez j'de l'occasion de m'exprimer devant vous le la France se bat pour que le budget de la PAC soient maintenus, maintenus

Monsieur moto G : le gouvernement a déjà engagé plusieurs actions sur le sur le PSE en 2017, le ministère a engagé un travail de recensement des dispositifs et initiatives publiques et privées, et je veux bien rappeler, publics et privés, parce que là on ne peut pas aller sans le sans l'autre, permettant de rémunérer des services environnementaux en France, c'est déjà, c'est déjà en place depuis 2017 faisant suite dans ce travail, le ministère de l'Agriculture, de l'alimentation, travaille à la réalisation de guide méthodologique, vous l'avez évoqué destinés aux services de l'État aux collectivités territoriales et aux organisations privées associatives afin de voir éclore sur tout le territoire DPS ce dans un cadre juridique et sécurisé, j'aurais rien de pire que de partir dans des, dans des situations qui ne soit pas juridiquement sécurisé, le gouvernement s'est donc engagée dans le cadre du plan biodiversité publié en juillet dernier à consacrer 150 millions d'euros d'ici 2021 pour des outils de paiements pour services environnementaux CPS viseront prioritairement à valoriser les pratiques bénéfique à l'environnement, notamment la préservation des sols et la restauration de la biodiversité partout, je veux dire à mon collègue Jean-Pierre de que les zones humides de trinquent qui sont totalement peuvent rentrer totalement dans ce dans dans ce dispositif, qui est en train de se mettre en place et le ministère de l'Agriculture et de la transition écologique travaillent conjointement sur, sur ce plan, je veux donc conclure, en vous assurant que le gouvernement est engagé dans cette direction et Éva travaille encore dans les mois et les, les, les mois qui viennent, ou les années qui viennent, afin de développer toutes les démarches permettant de soutenir les nombreuses prestations environnementales rendu par les agriculteurs, c'est déjà le cas, je le gouvernement donne un avis favorable positif à cette PPR mais nous voyons très bien qu'à l'heure où il est, il faudra encore aller plus loin pour développer. Pour préciser pour que ça puisse être mise en en en cohérence avec l'ensemble du droit français et européen et pour qu'un jour cela puisse être généralisé, je vous remercie. Nous allons procéder au vote sur la presse. Position de résolution, la conférence des présidents a décidé que les interventions des orateurs, explications de vote, je vais mettre aux voix la proposition de résolution et j'ai été saisi d'une demande de scrutin public par le groupe socialiste et républicain sur la proposition de résolution, il va être procédé au scrutin public, tant les conditions fixées par l'article 56 du règlement et le scrutin sera ouvert dans quelques instants.

Le scrutin est clos. J'invite les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.

Voici le résultat du scrutin numéro 40 sur l'ensemble du texte, et compte tenu de l'ensemble des délégations de vote accordé par les sénateurs aux groupes politiques et notifié à la présidence, nombre de votants 344 nombre de suffrages exprimés 329 pour l'adoption 131 contre 198, le Sénat n'a pas adopté. Chers collègues, je vais suspendre les la séance sera reprise à 18 heures 30 pour l'examen de la proposition de loi relative à l'obligation de déclaration d'un préavis de grève des contrôleurs aériens dans le cadre de l'ordre du jour réservé aux groupes les indépendants, la séance est suspendue.

La séance est reprise, la parole est à madame Nathalie Delattre pour une mise au point au sujet d'un vote. Oui, mais je vous en prie, madame la présidente, effectivement, au sujet de cette mise au point, c'est pour le scrutin numéro 39 Franck Menonville et moins main souhaitions voté pour, merci de votre prise en compte. Jean forme le Sénat que la commission mixte paritaire qui s'est réunie sur le projet de loi de finances pour 2019 n'est pas parvenu à l'adoption d'un texte commun. L'ordre du jour appelle la discussion de la proposition de loi relative à l'obligation de déclaration d'un préavis de grève des contrôleurs aériens, c'est une demande du groupe, les indépendants. Dans la discussion générale, la parole est à monsieur Joël Goerrian, auteur de la proposition de loi pour 10 minutes. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, la proposition de loi que nous vous invitons à prouver préserve d'une part, le droit de grève des contrôleurs aériens qui est un droit constitutionnel tout en assurant, d'autre part, la continuité du service public dans les aéroports, nous poursuivons ici 2 objectifs : tout d'abord, garantir la bonne organisation du trafic aérien, mais surtout assurer la protection des droits et la sécurité des passagers, il y a un peu moins de 4000 contrôleurs aériens en France qui sont responsables de la gestion et la surveillance des décollages et des atterrissages des avions du survol de l'ensemble de l'espace aérien national, ils sont en liaison constante avec les contrôleurs des pays voisins, leur métier est lourde responsabilité, ils travaillent soit dans un aéroport, soit dans l'un des 5 centres de contrôle régionaux leur compétence est d'une importance cruciale pour la bonne marche du trafic aérien qui impose des suggestions particulières. Cette proposition de loi conforte le droit de grève nous souhaitons seulement aborder les conditions d'exercice de ce droit, qui quand il est utilisé de manière impromptue a des conséquences épouvantables sur les usagers et les entreprises françaises. La France est à l'origine de 67 pourcent des mouvements de grève des contrôleurs aériens de toute l'Union européenne, causant en 97 pourcent des retards liés à ces grèves cette proportion ne fait qu'augmenter. En 2008, les grèves des contrôleurs aériens ont augmenté de 300 pourcent ce record en termes de jours de grève. Des implications négatives directes sur les passagers sur l'économie de notre pays et sur la compétitivité de nos entreprises, selon Price Water House Coopers 12 milliards d'euros ont été perdus sur la période 2010 2016 pourcent pour le seul secteur du tourisme c'est-à-dire. Un milliard d'euros d'une perte annuelle. Le pourtour de la Méditerranée se trouve très affecté et de nombreux jeunes en recherche d'emploi, perte des opportunités dans le tourisme. Les 2 jours de grève de 2015 le 8 et 9 avril ont engendré une perte de recettes supérieures à 20 millions d'euros pour le transport aérien français avec annulation de 1300 vols, soit 10 millions d'euros par jour de grève, alors je vous laisse imaginer ce qu'. Présente 254 jours de grève l'impact pour les compagnies aériennes françaises Air France et en Europe, ce chiffre à 66 millions d'euros en 3 ans, avec 3300 vols annulés et à 35 millions d'euros à cause des retards à chaque grève, les compagnies étrangères contourne le ciel français qui est un ciel très étendu, sur la période 2014, 2016. Ces 6 millions de kilomètres additionnels qui ont été parcourus qui entraîne bien sûr un lourd impact environnemental. Le coût important de ces grèves, si l'État a cédé à certaines revendications. Plusieurs grèves préavis de grève ont été levés avant même d'avoir été mis en application éviter temporairement une crise est une très bonne chose, mais n'apporte pas de solution durable, le cadre juridique français doit être plus protecteur des usagers. Il doit prévoir pour les voyageurs, une meilleure information en matière d'intention de grève des agents en cas de grève, la loi de 1984 sur le service minimum comme. Pourcent des survols ainsi qu'un certain nombre d'arrivées de départ dans un rapport, précisé par décret. Ce service minimum est essentielle et son maintien est indiscutable, cependant, son mode de gestion actuelle et pénalisant et induit des effets disproportionnés, le mode de gestion du service minimum ne prévoit aucune information sur le nombre de grévistes, compliquant ainsi les régulations de précaution. Effectués par les entreprises de transport aérien cela cause des retards et des annulations à la dire minute du fait du manque de prédictibilité une très fine un trèfle faible nombre de grévistes, l'effet de désorganisation. Lié au mode de gestion est telle que les retards, voire des annulations sont très importante. De 2015 à 2017, par exemple, le contrôle du trafic aérien français a fait face à 32 journées de grève sur les 40 recensés en Europe dont 16 de séjourner portait sur des revendications qui ne qu'on sorte qu'on s'en est pas les contrôleurs aériens, un système de notification. Préalable est donc indispensable, il permettra aux entreprises de transport aérien, d'éviter des hallucinations à chaud et une partie des retards causés par une minorité. Ainsi nous au moindre iront les pertes financières qui resteront bien sûr toute façon conséquente, la Commission européenne dans un rapport récent, recommande un préavis syndicale de 21 jours et un préavis individuel de 72 heures pour les contrôleurs aériens. Européen : vous le voyez, mes chers collègues, dans cette proposition, nous sommes très loin du compte. Quel est au fond l'objectif de l'article unique de la présente proposition de loi, il a pour but de tendre la loi Diard au service de la navigation aérienne, sous une forme appropriée. Il impose pour les contrôleurs aériens, une obligation de déclaration individuelle préalable de grève d'au moins 48 heures et non de 72 heures comme l'Europe le demande. Mes chers collègues, est ce que vous trouvez normal que des passagers français et étrangers, sans qu'il soit informé préalablement apprennent seulement au moment du décollage que leur vol est annulé. Des familles avec leurs enfants se sentent pris en 2 en otage, souvent démunis de toute alternative Dender ou de garde d'aéroports surchargés. Des passagers qui doivent support. C'est des frais d'hébergement supplémentaires parfois des frais d'annulation ou de transport qui ne leur seront jamais remboursés, ce coût caché des grèves dans le secteur aérien ne jamais chiffré mais il pèse sur les familles et les entreprises, ce coût caché des grèves est aussi psychologique et il se compte en heures de stress et de mal être. Cette situation, mes chers collègues n'est pas que l'érable et donne une image déplorable de notre pays, elle contraste avec l'essence du droit de grève. Telle qu'il est régi par la loi sur les transports. Qui repose sur l'assurance. Contre les atteintes disproportionnées aux libertés des usagers, la protection des besoins de la population et la continuité du service public. Mes chers collègues, les témoignages d'usagers victimes d'annulations et de perturbations de vol montre à quel point. Ce sont ces situations ont atteint à degré intolérable. Sur les réseaux sociaux, on trouve énormément de témoignages d'usagers victimes très souvent ils attribuent à tort à Air France la responsabilité de l'annulation, certains affirmant qu'ils ne partiront plus jamais avec cette compagnie. Depuis le dépôt de cette proposition de loi, j'ai eu des rendez-vous avec des passagers. Qui m'ont fait part de leur désarroi pour vous montrer concrètement l'ampleur du problème je voudrais vous dire quelques témoignages. Voici Aude. 5 de ce volontiers annulé en 2 mois, elle le dit. Les contrôleurs aériens prénom d'otages, l'ensemble des personnes qui souhaitent ou doivent voyager, mon entreprise a perdu 3 contrats au profit de compétiteurs et. Tanger nous envisageons le dépôt de bilan. Voici Evry un usager de l'aéroport de Marseille, je le cite : il faut que les contrôleurs aériens pense ce petit qui gagnent moins de 1500 euros et qui se prix toute l'année pour s'offrir un petit voyage et qui à cause de devront le se priver de cela. Myriam et votre grève de ses grands-parents agriculteurs, toute la famille avait cotisé pour leur offrir la croisière de leur rêve pour les 50 ans de mariage, son grand-père souffrant d'un cancer au moment du départ, le vol a été annulé le paquebot a quitté le quai sans ses grands-parents à l'écrit, si nous avions su s'24 heures plus tôt, nous serions partis en voiture aucun remboursement. Un rêve qui est devenu un cauchemar. Jérémy, au chômage depuis 2 ans, a finalement obtenu un 3ème entretien pour un emploi où il ne restait plus que 2 candidats, il écrit mon vol EasyJet. Vient d'être annulé tous mes espoirs s'envolent je suis désespéré. Justine a travaillé d'arrache-pied pendant un an pour passer un concours qui se présentent tous les 2 ans, elle a misé sur les tarifs attractifs d'une compagnie low cost ne ce qu'elle ne pouvait pas anticiper, alors que se trouve à l'aéroport. C'est qu'aucun avion ne partirait ce jour-là. Ahmed, qui n'a pas pu assister à la naissance de son fils, bloqués à. Sa banque à son volant, Ryan Air a été annulée à la dernière minute, de même pour l'il y a ce même vol ne lui a pas permis d'être témoin au mariage. Sa soeur jumelle, etc, etc, etc autant de cas individuels qui se multiplient et qui monte, il y a là du désarroi et on ne peut pas l'accepter avec l'augmentation des vols locaux. Mais sa collègue, il faut avoir compte. C'est ce que la croissance du trafic aérien et de plus en plus. Importante mais a conduit des personnes de revenus de plus en plus modestes à devenir des usagers. Or, ils sont aussi les plus menacées par la vraie l'imprévisibilité des annulations, car ils n'ont pas les moyens de les capacités de s'assurer. Ce sont de petits revenus, ce sont des personnes modestes qui se trouve impacté par le fait de ne pas avoir été prévenu à l'avance de l'annulation d'un vol. Pour eux, mes chers collègues. Pour Aude pour Aymeri pour Myriam pour Jérémy pour Justine et pour les milliers de victimes du fait d'une situation qui aurait pu être évité, j'en appelle à vos sentiments humanistes en soutenant cette proposition de loi, elle est celle du bon sens bon sens. Elle préserve bien entendu toute la portée du droit de grève. Droits sacrés en démocratie mais elle protège mieux les usagers et les entreprises, elle met fin à la capacité d'une minorité à mettre en souffrance des personnes innocentes. Elle rend notre système de transport aérien plus efficace l'alors en plus sûr, mais surtout elle rendra plus humain, je vous remercie de votre attention. La parole est à monsieur Alain Fouché. Porteur pour la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable pour 10 minutes chers collègues.

Madame la présidente, Madame la Ministre, Monsieur le président de la commission mais, chers collègues, la proposition de loi que nous examinons ce soir un objectif simple : mieux organiser le service de la navigation aérienne en cas de grève au profit des usagers Joël Gariod vient de l'évoquer, nous avons tous été témoins de scènes insupportables dans les aéroports et vu des passagers dont le vol vient d'être annulée attendre désemparés, des heurts sans qu'aucune solution ne soit proposée, la grève des contrôleurs aériens ne sont pas bien sûr la seule cause des annulations et des retards de vols puisque ceux-ci sont aussi imputables aux conditions météorologiques, aux difficultés de gestion des compagnies aériennes ou à la saturation des capacités de contrôle aérien, dans un contexte de très forte croissance de trafic aérien, toutefois, les mouvements sociaux qui toutes les services de la navigation aérienne, je crois qu'une cause non négligeable des perturbations en France qui au demeurant est le pays qui de tient le record européen du nombre de grèves de contrôleurs aériens, le rapport sur le contrôle aérien que notre collègue Vincent Capo Canellas a publié cet été, est assez éloquent sur ce point entre 2004 et 2016, la France a enregistré 254 jours de grève a été responsable 67 pourcent des jours de grève, qui se sont produits, en Europe, la France se distingue notamment par le fait que de nombreuses grèves de contrôleurs aériens ne sont pas lié seulement à des revendications propres au métier de navigation aérienne, mais sont des grèves de solidarité avec la fonction publique, des pressions des préoccupations communes à l'ensemble des flux, les fonctionnaires et qui n'ont rien avoir été aéronautique enseignement hospitalier, etc, comme je l'indiquais c'est grève provoque des annulations et des retards de vols importants si la plupart. Du temps, les compagnies aériennes sont d'incapacité d'informer leurs passagers des annulations de vols en amont il arrive du fait des difficultés anticiper le nombre de grévistes et organisé le service en conséquence que certains vols soient annulés à chaud, alors que les passagers sont déjà présents dans l'aéroport, voir dans les avions, ce qui est particulièrement difficile à vivre pour eux se tissu explique par le fait que le cadre actuel du droit de grève des contrôleurs aériens ne permet pas à la DGAC d'organiser au mieux le service afin de limiter au maximum les perturbations pour les passagers, quel est ce cadre et pourquoi est-il insuffisant le déclenchement de la grève sous peine de sanctions, par ailleurs, ces agents sont soumis à une obligation de service minimum en cas de grève, cela signifie qu'un certain nombre d'entre eux sont réquisitionnés par l'administration afin que certaines missions soit assurée notamment les missions de défense et de secours pourcent de la capacité de survol du territoire aérien soit maintenu et que des aéroports naturellement sur l'ensemble du territoire soit ouvert pour assurer un certain nombre d'arrivées et de départs de vol est le service minimum permet d'assurer le maintien d'un certain volume d'activité en cas de grève il ne fonctionne pas de manière optimale, aujourd'hui, en effet, les agents de la DGAC ne sont actuellement pas tenue de déclarer individuellement s'il participe ou non à une grève et, par conséquent, l'administration ne connaît pas à l'avance le nombre de grévistes, qu'il y aura, or, étant donné que les activités de surveillance de la navigation aérienne présente des gens vieux de sécurité important, l'administration doit par précaution demander aux compagnies aériennes de supprimer un certain nombre de vols, alors même que cela peut finalement ne pas être nécessaire, 2 exemples : il arrive en effet que la grève soit peu suivie et que le nombre de vols annulés, soit trop important par rapport aux capacités de contrôle à l'inverse, lorsqu'une grève c'est davantage suivi que ce qui était envisagé, cela se traduit par des retards, voire des annulations de vols, car les capacités de contrôle sont saturés, problèmes humains, problèmes financiers, c'est ce manque de prévisibilité pardon que la proposition de loi cherche à corriger en obligeant les personnels de la navigation aérienne, a déclaré individuellement leur intention de participer à une grève au plus tard 48 heures avant son début et à en informer leur employeur qu'il renonce à participer à cette grève, ou s'ils souhaitent reprendre leur service 24 heures avant, c'est quand même pas compliqué comme texte une telle obligation de déclaration individuelle de participation à une grève existe déjà dans le secteur des transports s'agissant des salariés des entreprises de transport terrestre par exemple la SNCF par exemple Madame la ministre de la RATP, les salariés des entreprises de transport aérien, notamment Air France, vous l'aurez compris mes chers collègues, l'objectif de cette proposition n'est en aucune manière de remettre en cause le droit de grève des personnels de la navigation aérienne, c'est clair, les agents pourront continuer à faire grève, mais qu'ils devront préalablement le déclarer au préalable, tout ça pour des raisons évidentes de sécurité, la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable, monsieur le président, a approuvé cette proposition toute en améliorant sa rédaction sur plusieurs points, tout d'abord, la commission a restreint le Champ d'application de l'obligation de déclaration préalable de participation à une grève afin qu'elle ne concerne que les personnels qui concourent directement à l'activité de transport aérien de passagers et de tous les personnels de la navigation aérienne, comme c'était le cas, en effet, si le Conseil constitutionnel reconnaît la compétence du législateur pour limiter le droit de grève en vue de le concilier avec d'autres principes à valeur constitutionnelle, ces limitations doivent toutefois être proportionnée à l'objectif fixé par ailleurs, la Commission a prévu que les informations très important issues des déclarations préalables soient couvertes par le secret professionnel ainsi leur utilisation à d'autres fins que celles d'organiser le service pendant la grève ou leurs communications à des tiers serait passible d'un an d'un prisonnier mort ou de 15 millions de 15000 euros d'amende en cas de millions c'est beaucoup 15000 euros c'est déjà beaucoup, un an d'un prix zone ment ça puis quand même, enfin, la commission a adopté plusieurs amendements visant à harmoniser la rédaction de la proposition de loi avec les dispositions législatives existants et à modifier entité intitulé pardon de la proposition de loi afin qu'ils correspondent mieux mieux au dispositif qu'elle prévoit voilà, mes chers collègues. Des éléments que je souhaitais porter à votre connaissance, cette proposition de loi est utile, elle est même indispensable qu'elle le réglera réglera certes pas toutes les difficultés auxquelles les passagers sont exposés, elle permettra de mieux organiser le service de la navigation aérienne en cas de grève. Au profit des usagers. Pour des raisons de sécurité, aussi je j'donc à voter cette proposition de loi qui était excellente. Merci, monsieur le rapporteur, la parole est à Madame Élisabeth Borne, ministre chargée des transports. Alors je vous en prie Madame amis.

Madame la présidente, mesdames et messieurs les sénateurs. Vous le savez et Monsieur le Sénateur, Rio, ainsi que monsieur le rapporteur Foucher long justement rappelé le transport aérien est essentielle pour répondre aux besoins de déplacement de nos concitoyens. C'est également un secteur vital pour notre économie, puisque si l'on tient compte de la construction aéronautique, ils représentent 4,3 pour 100 de notre PIB et emploie directement plus de 320000 personnes. Je tiens à vous redire la constance de mon engagement en faveur de ce secteur. C'est pourquoi j'ai voulu organiser au travers des Assises nationales du transport aérien, une grande phase de concertation et de réflexion approfondie avec l'ensemble des parties prenantes ma détermination à faire de ces assises, le socle d'une stratégie pour le transport aérien français n'a pas varié. Depuis 3 ans, le transport aérien connaît une forte croissance en Europe, souvent concentrés sur certains axes, et qui n'avait pas été prévue dans les hypothèses d'établissement des plans de performance des prestataires de navigation aérienne européen. Cette croissance fait suite à plusieurs années de stagnation au cours desquelles la priorité avait été mise à l'échelle européenne sur la maîtrise, voire la baisse des taux de redevance pour les services de nana de la navigation aérienne. C'est ainsi que les effectifs de contrôleurs aériens ont diminué de 10 pourcent et que des investissements ont dû être reportées. Malgré cette situation, je sais que l'impératif de sécurité est la priorité numéro un de l'ensemble des acteurs de l'aérien. C'est bien sûr la mienne et celle de mes services. Cependant, avec la reprise du trafic, le système de contrôle aérien dans bon nombre de pays européens se retrouvent en tension en raison du manque de capacité pour traiter tous ses vols. Cela crée, en particulier en période estivale, de nombreux retards au coeur des routes européennes. Nous avons se partager ce constat au cours du dernier conseil des ministres Transports en nous appuyant sur le rapport d'Eurocontrol, qui a mis l'accent sur les situations particulières de l'Allemagne du bénédiction du Bénélux ou encore de la France. Certains de ces retards résultent d'aléas météorologiques. D'autres sont directement du au modèle d'exploitation de certaines compagnies aériennes. cela est d'autant plus prégnant que l'organisation par opérationnel des transporteurs visant à faire voler le plus possible, chaque avion un aléa localisés peuvent perturber le programme complet d'une journée. Cependant, c'est un fait, le contrôle aérien reste responsable d'une partie de ces retards, en raison notamment du retard de la modernisation des systèmes, des besoins en ressources humaines et, parfois, il faut le reconnaître des jours de grève. Je salue ici le travail de votre collègue, le sénateur Capo Canellas, hélas, qui a su éclairer dans son rapport, tous ces aspects et d'nous pourrons tirer collectivement des enseignements. Le gouvernement est attaché à remédier aux causes structurelles de ces retards des axes de progrès ont été définies en concertation avec les représentants du personnel, c'est ainsi qu'un protocole social a été signé avec 4 organisations syndicales de la direction générale de l'aviation civile, représentant plus de 70 pourcent des personnels. ce protocole cadre à l'issue d'une négociation globale fixe les mesures retenues pour accroître la performance du contrôle aérien sur les années 2016 à 2019. Cette démarche montre la volonté partagée de faire évoluer l'organisation du travail, en concertation avec les organisations syndicales. Il prévoit notamment des expérimentations sur de nouvelles organisations du travail dans ta d'entre elles ont été engagées dans certains centres depuis plusieurs années. Ces expérimentations ont en particulier permis d'absorber les dernières hausses du trafic aérien et je voudrais à cet égard, salué le professionnalisme et l'engagement des agents de la navigation aérienne. Ces expérimentations doivent se poursuivre et devront être dans d'autres centres. Nous devrons certainement aller plus loin encore, désormais, pour accompagner une croissance durable du trafic aérien, le recrutement d'effectifs opérationnels en quantité suffisante sera nécessaire en France comme ailleurs en Europe, sachant qu'en France, le gouvernement a poursuivi l'effort de recrutement conduisant à remplacer la totalité de des départs de contrôleurs aériens. Il a également été décidé un très important effort d'investissement pour le renouvellement des systèmes de navigation aérienne. Monsieur le sénateur Capo Canellas, vous l'avez souligné dans votre rapport, nous agissons à partir de 2019 nous investissons près de, de, de 300 millions d'euros au profit de l'ensemble de ses systèmes de navigation aérienne. Je veillerai à ce que les mesures adéquates soient prises pour assurer en particulier la mise en service en 2021 2022 du nouveau système for Flight. C'est sur ces bases que la France aborde la négociation européenne en cours, qui fixera le cadre économique et la régulation associée sur les 5 années à venir, toutes ces thématiques font et continueront à faire l'objet d'un dialogue social danse visant à accroître de façon concertée, la performance de la navigation aérienne. Il demeure que la navigation aérienne doit gérer des mouvements sociaux, ceux-ci sont de différentes natures, ils peuvent en effet être commun à l'ensemble de la fonction publique, on a ainsi dénombré 14 mouvements de ce type en 2017 et 3 au 1er semestre 2018. Il peut s'agir également de grèves locales. Il y en a eu 30 de ce type en 2017 et 10 au 1er semestre 2018. Ces épisodes ont eu n'ont eu un impact sur les opérations des compagnies aériennes et par là même le service aux passagers, qu'il s'agisse de survol ou de vols partant ou arrivant en France. L'accessibilité de l'espace aérien aérien français et de ses principaux aéroports reste assurée grâce aux dispositions de la loi du 31 décembre 1984 sur le service minimum qui était essentiel pour garantir les besoins vitaux de la France et le respect de nos engagements internationaux, en particulier en matière de droits de survol de notre territoire. En application de cette loi, une obligation de résultat s'impose. Le texte prévoit en effet que doivent être assis a su assurer, je cite, en toutes circonstances les services nécessaires à la continuité de l'action gouvernementale et l'exécution des missions de la défense nationale, la préservation des intérêts aux besoins vitaux de la France et le respect de ses engagements internationaux, notamment le droit de survol du territoire l'émission nécessaire à la sauvegarde des personnes et des biens, le maintien des liaisons destiné à éviter l'isolement de la Corse, des départements et territoires d'outre-mer et la sauvegarde des installations et du matériel de ses services. Un service minimum est enfin garanti sur certains aéroports dont la liste est fixé par décret. Ce service minimum est mis en oeuvre au moyen d'astreinte à demeurer en fonction. C'est bien ce service minimum déjà fixé par la loi, qui garantit la continuité du transport aérien en toute circonstance. Il me paraît également important de rappeler dans cette enceinte que le préavis de grève de 5 jours applicable à tout service public est évidemment applicable au service de la navigation aérienne sont stricte respect est indispensable tant pour négocier que pour mettre Malte réellement en oeuvre les dispositions du service minimum. Ce délai de 5 jours permet également d'informer des compagnies aériennes, voire de leur recommander de réduire leur programme de vols il y a en effet préférable que des vols, soit annulée en amont plutôt que de faire attendre des passagers sans information dans les aérogares. La proposition de loi de monsieur le sénateur Guy Rioux que vous examinez aujourd'hui vise à ajouter une pièce à ce dispositif, en demandant à nos personnels de signaler individuellement leur intention de participer à la grève 48h avant le début du mouvement, pour plus de prévisibilité. Plus précisément, elle étend les dispositions aujourd'hui applicable aux entreprises de transport aérien aux personnels des services de la navigation aérienne qui assure des fonctions de contrôle d'information de vol et d'alerte et qui concourent directement à l'activité du transport aérien de passagers. De telles dispositions permettrait certainement de partager avec les compagnies aériennes, une information plus fiable et plus précises sur nos capacités de contrôle disponible les pratiques actuelles conduisent en effet à certaines approximations dans l'évaluation de la capacité de de survol garantie en l'absence d'un dispositif permettant de savoir avec précision qui se déclarent grévistes ou non. L'information des passagers restera assuré par les compagnies aériennes qui sont seuls en capacité de définir leur programme de vols à partir des informations que le contrôle aérien leur communique. Vous le savez, le droit de grève est un droit constitutionnel. Par ailleurs, je mesure bien qu'un dispositif de déclaration préalables individuel permet dans certains cas d'ajuster au plus près le volume des astreintes à demeurer en fonction ce qui évite qu'un trop grand nombre d'agents fassent l'objet de ces mesures d'astreinte au final, on l'aura compris, le dispositif envisagé vise à se doter d'une plus grande prévisibilité afin d'organiser le service au mieux et de limiter au maximum les perturbations pour les passagers. Chacun conviendra que le sujet qui nous occupe est éminemment sensible, dans la mesure où il touche à des libertés aussi essentielles que celle de se déplacer et au droit de grève. Dans ces conditions, j'estime qu'il mérite un examen approfondi, ainsi qu'une concertation poussée, à mon sens, on aime en effet l'impact des dispositions proposées par monsieur le sénateur guerre Yo doit être clairement mesurées et discuter, il me semble également nécessaire de partager l'analyse précise du bénéfice escompté et les limites éventuelles de la modification législative envisagée. Comme vous le savez la semaine dernière a été l'occasion d'élections professionnelles au sein de la fonction publique, dans ces conditions, aucune concertation suffisamment complète n'a pu être menée, même si j'ai bien noté monsieur le rapporteur, que vous aviez reçu les organisations syndicales dans le cadre de vos auditions. Aussi, je suis convaincu qu'un travail sur un sujet aussi important que l'exercice du droit de grève doit être réalisée de façon approfondie et être enrichie par un niveau de concertation adéquates. la question que vous posez, monsieur le sénateur Kerriou exige que l'ensemble des parties prenantes, y travaille avec un esprit de dialogue et d'écoute, cela mérite selon moi un temps de débat significatif avec les organisations syndicales et les compagnies aériennes. Les événements récents qui ont eu lieu dans notre pays des colère et désespoir qui se manifeste encore aujourd'hui nécessite de la part des élus que vous êtes et des personnes responsables que nous sommes une une méthode fondée sur un dialogue et une écoute renouvelée et le 1er ministre le rappelait, jeudi dernier, à cette même place, certains problèmes demandent des solutions rapides et d'autres nécessitent des concertations plus large. C'est dans cet esprit que je discuterai ce soir avec vous, de votre initiative parlementaire en vous invitant à toute la sagesse dont vous savez faire preuve mais également en appelant à votre sens des responsabilités dans cette, dans une période comme celle que nous vivons, qui impose plus que jamais l'unité du pays, je vous remercie. Merci madame la ministre, dans la suite de la discussion générale, la parole est à monsieur Frédéric Marchand pour 7 minutes. Madame la présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues, nous examinons ce soir, la proposition de loi de notre collègue Joëlle Gayot relatives au droit de grève des contrôleurs aériens qui consiste à obliger les contrôleurs aériens mais aussi d'autres personnels des services de la navigation aérienne, a déclaré individuellement leur intention de participer à une grève au moins 48 heures avant son commencement et à informer leur employeur s'ils y renonce, ne nous y trompons pas : la problématique soulevée par cette proposition de loi est réel en en effet depuis plusieurs années les Grève du contrôle aérien français ont perturbé le ciel européen à de nombreuses reprises et notre pays est à l'origine de plus de 60 pourcent des mouvements de grève de contrôleurs aériens de toute l'Union européenne, causant une très grande majorité de retards liés à ces grèves, il est aussi indéniable que des actions répétées engendrent des perturbations pour des millions de passagers, ça a été dit, qui se voit contraint d'annuler des réunions des vacances des nuits d'hôtel, voire même pour certains de nos collègues, annulée, réunion ou présence dans cet hémicycle, bref, j'ai bien à l'esprit que les désagréments engendrés par ces grèves sont très importants pour les voyageurs, j'ajoute même que l'impact environnemental de ces mouvements est également significatif puisque sur la période 2014, 2016, il est estimé que 6 millions de kilomètres additionnels ont été parcourus en conséquence des grèves des contrôleurs aériens en France cette proposition part du constat que la France est le pays en Europe qui connaît le plus grand nombre de grèves de contrôleurs aériens, je voudrais simplement ajouter que les mouvements sociaux explosent partout en Europe, à la suite d'une augmentation record du trafic, conjuguée à la baisse des effectifs qualifiés cette combinaison touche plus particulièrement la DSN a aujourd'hui plus gros pourvoyeurs de délais en Europe, notre collègue Alain Fouché Anedic dans son rapport que les grèves ne sont pas la seule cause des retards des vols puisque, outre les conditions météorologiques et les difficultés de gestion qui incombe aux compagnies aériennes, ceci résulte principalement du manque de personnel dans un contexte de très forte croissance du trafic aérien et de la vétusté des instruments de gestion de la navigation aérienne qui induisent un manque de capacité de contrôle, même si elles représentent 20 pourcent des causes de retard, notons que selon la CFDT, qui s'appuie sur les chiffres fournis par Eurocontrol, les grèves ne représentent que 1 pourcent du total des délais européens alors que les compagnies sont responsables à elles seules de 55 pourcent de ces retards et les problèmes d'effectifs des prestataires de contrôle de 15 à 20 loin de moi l'idée de remettre en cause les chiffres indiqués dans le rapport, mais simplement souligner qu'il existe manifestement des causes multiples à ces retards et un désaccord profond sur la logique et les chiffres avec une organisation syndicale réputé réformiste de même, je tiens à souligner que le Syndicat national des contrôleurs du trafic aérien a effectué une mise en garde, arguant que si cette proposition de loi devait être adopté, cela mettrait forcément un coup d'arrêt à la concertation pour améliorer les conditions de la navigation aérienne dont ce syndicat convient que c'est bien évidemment une nécessité aussi dans un contexte de tension sociale Madame Elis, madame la ministre, vous l'avez rappelé que nous vivons, il convient d'aller vers l'idéal, en passant par le réel en balayons pas d'un revers de main la position des organisations syndicales, par ailleurs, le personnel qui dépend de la direction des services de navigation aérienne est composée de fonctionnaires qui ne peuvent participer à une grève que s'ils sont couverts par un préavis émanant d'une ou plusieurs organisations syndicales représentatives, transmis à l'autorité hiérarchique 5 jours francs avant le déclenchement de la grève, ce délai de préavis et systématiquement respecté par les organisations syndicales et s'ils ne l'étaient pas l'administration pourrait prendre des sanctions disciplinaires à l'encontre des agents grévistes en outre cela aussi été dit ces mêmes agents sont soumis depuis la loi du 31 décembre 1984 à une obligation de service minimum qui permet concrètement que certains services essentiels puisse continuer à être assurée pendant les grèves, il existe donc aujourd'hui des mesures qui permettent un service minimum, même si j'en conviens, elles peuvent être améliorées. En conclusion, je dirais que l'objectif de cette proposition de loi est certes louable, puisqu'il s'agit d'assurer un meilleur service et d'éviter au maximum les désagréments causés aux voyageurs européens par les grèves françaises, néanmoins je dirais aussi que cette proposition loin induit une méthode Coué City veut qui ne me paraît guère de nature à apaiser le climat social déjà tendu dans ce secteur, mais aussi, et cela n'aura échappé à personne dans toute la France avec le mouvement qui traverse le pays depuis plusieurs semaines et dont on ne saurait faire abstraction, sauf à se condamner à être hors sol de la même manière, le calendrier de cette proposition de loi me semble pour le moins inopportun cet avis étant d'ailleurs partagée par des organisations représentatives des compagnies aériennes, avec qui j'ai pu échanger sur le sujet en effet en 2019 auront lieu les négociations sur le protocole social entre le personnel de la DGAC et ça hiérarchie à ce titre, les questions soulevées dans cette proposition de loi pourront être mis sur la table dans le cadre du dialogue social, mes chers collègues, nous vivons depuis plusieurs semaines, un climat de tensions extrêmement vives dans le pays, cela a été dit sur tous les bancs de notre assemblée, c'est d'abord et avant tout le fruit de plus de 40 ans de politiques qui n'ont pas pris assez en compte la vie des citoyens et des salariés aussi, même s'il apparaît nécessaire de mieux encadrer le droit de grève des contrôleurs aériens, dans ce contexte, cette proposition de loi me semble de nature à créer de l'incompréhension et des polémiques qui seront interminables, voire de mettre le feu aux poudres il me semble donc beaucoup plus opportun de traiter ces questions dans le cadre du futur protocole de négociations sociales entre le personnel de la DGAC et ça hiérarchie qui sera lancé en 2019 pour toutes ces raisons, mes chers collègues, le groupe la République en marche s'abstiendra. Pour 6 minutes. Madame la présidente, où notre pays affronte une grave crise sociale et institutionnelle avec le mouvement des Gilets jaunes qui dénonce d'un même mouvement, la vie chère la déconnexion des élites et les inégalités sociales et fiscales, le Sénat donc a inscrit à l'ordre alors de du jour, un texte qui peut apparaître comme une énième provocation au monde du travail et aux salariés du de ce un texte qui sous-entend que les difficultés du transport aérien ne serait pas le fruit du libéralisme exacerbé de la soumission ce secteur au seul prisme de la rentabilité, indépendamment des exigences de sécurité et de service public mais bien au contraire, la faute des salariés du contrôle aérien par leur usage intempestif de leur droit constitutionnel de se mettre en grève lorsqu'ils estiment que leur outil de travail et leurs conditions salariales sont menacés, sincèrement, ce n'est pas sérieux alors que le protocole social doit être vu l'année prochaine que ce secteur est déjà soumis à la mise en oeuvre d'un site d'un service minimum extrêmement contraignants et efficace qui permet la réquisition de personnel dans des conditions très large, les auteurs de cette PPL souhaite aller toujours plus loin pour excusez-moi, casser les droits des salariés, nous considérons pour notre part, qu'il s'agit d'une atteinte disproportionnée un droit constitutionnellement reconnu une atteinte inadmissible aux droits fondamentaux des salariés ainsi les dispositions de ce texte organise un système de déclaration individuelle de grève 48h en amont du mouvement, le salarié ne devrait également pas y renoncer, moins de 24 heures avant, sous peine de sanctions disciplinaires, ces dispositifs sont bien plus subtil que l'interdiction pure et simple de la grève en rendant son exercice plus difficile et en l'individualise en ses promoteurs permettent que s'exerce sur les salariés des pressions inacceptables, alors que l'exercice du droit de grève est par essence collectif de tels dispositifs ne sont pas nouveaux, ils ont été introduits par la loi pour les transports terrestres en 2007 et pour les transports aériens concernant le pape personnel navigants en 2012, nous avons à chaque fois saisi le Conseil constitutionnel, alors certes, celui-ci a estimé que cette tisser loi n'était pas contraire à la Constitution, cependant, nous considérons que de telles décisions sont de nature purement politique et qu'elle se place en contradiction avec les jurisprudences des autres cours de justice dans l'arrêt Air France de 2003 la Cour de cassation a ainsi reconnu qu'il ne pouvait être imposée à un salarié d'indiquer à son employeur, son intention de participer à la grève avant le déclenchement de celle-ci dans l'affaire de la société Rhodia chimie, la cour d'appel de Grenoble a également jugé en 2002 que la société ne pouvait interroger chaque salarié sur ses motivations, sans exercer une pression inacceptable sur chaque salarié pris individuellement, nous continuons donc d'affirmer que des déclarations préalables de grève porte une atteinte caractérisée et inacceptable, le droit de grève et qu'elles ne répondent pas aux exigences d'amélioration et de renforcement du dialogue social, les amendements déposés sur ce texte semble revenir sur ces dispositifs pour les remplacer par une sorte d'alerte sociale que s'est-il passé entre-temps. Avez-vous pris conscience qu'attiser la colère sociale aussi frontalement et sans fondement, était un mauvais calcul, nous sommes d'accord avec vous, au moins sur un point : soumettre l'exercice du droit de grève des contrôleurs aériens à la double contrainte d'un service minimum et d'une déclaration individuelle revient à rendre l'exercice d'un droit constitutionnel impossibles, d'ailleurs la position du Conseil constitutionnel pourrait évoluer lors d'une éventuelle saisine sur cette PPL mais soyons clairs ce texte répond en réalité à une demande des compagnies britanniques, irlandaises et hongroise qui ont porté plainte contre la France auprès de l'Union européenne afin de protester contre la grève des contrôleurs aériens français, voilà la vérité encore une fois, on veut faire primer le jeu du marché sur les droits des salariés, nous ne pouvons l'accepter, je voudrais juste pour finir, vous parlez des véritables maux du transport aérien et des causes réelles de retards et d'annulations, les grèves ne constitue qu'une partie à un film, cela a été dit des dysfonctionnements entraînant de retards de l'ordre de 1 pourcent le reste est lié aux compagnies environ 55 pourcent à la météo, environ 20 pourcent et au manque d'effectifs, environ 15 à 20 pourcent ce qui détériore la qualité du service aérien, c'est bien le dogme de la concurrence, le manque de moyens humains et la faiblesse des investissements publics le renforcement même à tout, de service public comme cela va se poursuivent avec la privatisation d'ADP prévue par la loi, alors que le rapport de la commission des finances, ouvrez d'autres portes et pointait notamment la vétusté des matériels et instruments de navigation cette PPL ne retient que la limitation du droit de grève, véritables chiffon rouge pour la droite sénatoriale, à nos yeux, la priorité reste bien au contraire, il faut le démontrer reste, bien au contraire, de moderniser et d'investir dans le contrôle aérien dont l'importance pour la sécurité des passagers aériens est incontournable il nous faut sortir de la spirale infernale du dumping social et de l'étau de l'austérité à tous les étages, il convient également de restaurer les conditions d'un dialogue social de qualité pour entende et réponde enfin aux revendications légitimes et justes, des organisations syndicales et des salariés, donc vous l'aurez compris mes chers collègues, nous nous opposerons à cette PPL. Merci, la parole est à Madame Nicole Bonnefoy, pour 10 minutes je vous en prie, mes chers collègues, on respecte les orateurs. Merci madame la présidente, madame la ministre, monsieur le rapporteur, chers collègues, nous examinons aujourd'hui donc une proposition de loi relative à l'obligation de déclaration d'un préavis de grève des contrôleurs aériens qui pour nous n'est pas satisfaisante ni sur la forme ni sur le fond, pas satisfaisante sur le fond car nous considérons que les grèves du contrôle ne sont pas le problème majeur du transport aérien en Europe comme un atteste d'ailleurs c'est pas moins de rapport dans fourni sur le sujet, récemment publiés par EDF et Eurocontrol, en effet, selon les différentes estimations issues de ces 2 rapports, les raisons imputables au contrôle aérien dans lesquelles nous trouvons des problèmes d'effectifs, ça a été souligné des conditions météorologiques et des faits de grève n'entraînerait que de 5 à 10 pourcent des retards de vols, si les 2 premières causes sont les plus importantes en nombre, je me rappelle, problèmes d'effectifs et conditions mais météorologique, les faits de grève, eux, ne sont que très marginaux, ainsi on peut donc noter que la durée moyenne de retard causé par un mouvement de grève des contrôleurs aériens est inférieure à 55 secondes par vol la conflictualité sociale dans le secteur du contrôle aérien des donc pas l'élément le plus pénalisant pour la compétitivité des compagnies françaises mais plutôt et ça a été dit, le manque de moyens humains alloués au centre de contrôle si les impondérables et les imprévus sont inéluctables en matière de contrôle aérien de par la nature même de l'activité exercée l'prof, la proposition de loi que nous examinons aujourd'hui permet de détourner le regard d'autres problèmes engendrés, eux, par les compagnies aériennes, ainsi quand, dans l'exposé des motifs, cette proposition de loi s'attarde sur la situation de famille en détresse dans les aérogares, il convient de rappeler que ce problème n'est aucunement le fait des contrôleurs aériens, mais plutôt de celui des compagnies low-cost dont le modèle économique ne permet que très rarement, d'assurer l'hébergement des passagers en pareille situation, cette proposition de loi n'est pas plus satisfaisante sur la forme, au moment où bon nombre de noeuds concitoyens réclament et ça a été rappelé un dialogue social rénové et efficient, en effet, alors que l'accord social quadriennal du secteur du contrôle aérien civil sera renouvelé au cours de l'année 2019, il nous paraît plus adéquat d'utiliser ce levier, qui a fait ses preuves depuis 1986 car nous le répétons, ce texte n'améliorera pas la situation du contrôle aérien civil en France mais au contraire le complexe suffira inutilement en cas de grève en fragilisant des droits acquis de longue date, comme d'ailleurs le souligne notre collègue Vincent Capo aucun hélas dans son amendement. En effet contraindre chaque agent à informer individuellement ses supérieurs et hiérarchique de ses intentions, Catane quant à la participation à une action sociale reviendrait à individualiser de manière insidieuse, le droit de grève plutôt que d'imposer aux contrôleurs aériens, une obligation de réquisition qui ne pèserait que sur, il est préférable de travailler sur l'amélioration de l'efficience du service minimum par le biais d'un dialogue social réinventer et plus Direct entre les différentes parties prenantes et il ne vous a pas échappé, mes chers collègues, c'est ce que les corps intermédiaires réclament et les citoyens eux-mêmes, donc pour toutes ces raisons, le groupe socialiste se prononcera contre cette proposition de loi.

Madame la présidente, Madame la Ministre, Monsieur le président de la Commission, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, on a coutume d'assigner à la France, souvent de manière hâtive, le trophée peu valorisant de championne du monde de la grève, bien entendu, untel jugement assez largement notre histoire sociale n'est-ce pas mon cher collègue, dont l'un des produits, le préambule de la Constitution du 27 octobre 46 qui à juste titre le droit de grève comme un droit fondamental, si ce droit doit être défendu sans concession sa compatibilité avec le principe de continuité du service public n'en est pas moins fondamental, or, si le contrôle de la circulation de la navigation aérienne constitue bien un service public assuré par des fonctionnaires, ce dernier de manière difficilement compréhensible à certaines règles de droit commun en ce qui concerne le service minimum, cela a été dit en 2012, la loi dite Diar avait instauré le principe d'un préavis individuel de grève de 48 heures pour tous les salariés des entreprises ou établissements qui concourent directement à l'activité de transport aérien de passagers, en particulier lorsque leur absence est de nature à affecter la réalisation des vols je pense pouvoir affirmer mes chers collègues, qu'il est difficile de nier que les contrôleurs aériens participent au service public du transport aérien de passagers extrêmement technique, cette profession est indispensable à la fois pour la souveraineté de notre espace aérien pour la sécurité des passagers pour la coordination des vols et pour la bonne tenue du ciel européen où la France possède une place centrale, or cette profession n'est pas soumise au principe du préavis de grève individuel de 48 heures alors que même les mouvements sociaux qu'elle organise on des conséquences massive pour nos concitoyens, la proposition de loi notre collègue Joël Gariod nous ouvre donc la possibilité de corriger, on va dire que cet oubli en exigeant également des contrôleurs aériens après avis individuelles de grève de 48 heures un alignement logique sur les règles auxquelles sont soumis les autres personnels qui participent directement à la réalisation du service de transport aérien de passagers. Je veux pour preuve le fait que les contrôleurs aériens n'ont jamais été entravés dans leur exercice de leur droit de grève puisque le corps des ingénieurs de contrôle de la navigation aérienne n'a fait partie de ceux qui en font le plus grand usage dans la fonction publique d'État entre 2004 et 2016, les contrôleurs aériens ont effectivement accumulé plus de 250 jours de grève, entraînant une perte d'environ 300 millions d'euros par an pour les compagnies aériennes, mais surtout des conséquences néfastes pour des millions de passagers sans parler des conséquences financières, puisque l'activité de contrôle et facturé aux compagnies aériennes, outil d'une redevance pour service rendu chaque journée dépourvue de contrôle coûte ainsi à l'État entre 3 millions et 4 millions et demi d'euros sans parler des conséquences et des pertes financières pour le tourisme français comme l'a dit mon collègue Deriot. Cette situation, qui conduit la France à être responsable du tiers des retards dus aux contrôles en Europe n'est plus acceptable et d'autant plus moins compréhensible pour nos concitoyens, que les contentieux contrôleur aérien bénéficie de conditions de travail de rémunération objectivement très favorable et déjà revalorisé en 2016 par le dernier protocole social de la DGAC. Naturellement, nous comprenons leur cohérence avec les lourdes responsabilités dans les contrôleurs aériens ont la charge, toutefois, dans ce cadre, il nous semble être une juste contrepartie que nous puissions avoir une meilleure visibilité sur l'organisation des grèves effectuées par les contrôleurs aériens, la mesure de l'enjeu dépasse largement les frontières nationales, puisque la France est le centre névralgique de la circulation aérienne en Europe, devant le Royaume-Uni et l'Allemagne, nous disposons en effet du premier espace aérien du ciel européen avec plus de 8600 contrôles effectués chaque jour, chiffres dont l'augmentation est constante depuis maintenant plusieurs années, c'est d'ailleurs pour cette raison que le coût temporel, la journée de grève sur le trafic est beaucoup plus important en France, environ 35000 minutes qu'en Allemagne, en Italie ou en Grèce. Au-delà des questions intérieures cette position nous impose donc une forme de responsabilité, à commencer par une meilleure une amélioration, pardon, de l'information sur l'organisation des mouvements sociaux dans le secteur aérien pour toutes ces raisons large majorité du groupe RDSE soutiendra la proposition de loi du groupe des indépendants en attirant toutefois l'attention sur le fait qu'il faudra explorer les autres pistes suggérées par notre collègue Vincent Capo Canellas pour améliorer l'état du trafic Canaries aérien en France, totalement dans le cas du du prochain protocole social que a dit ma collègue de la DGAC nous par son par exemple à la réforme en profondeur des rythmes de travail des contrôleurs aériens pour les effets attendus en termes de fluidification du service sont particulièrement prometteurs, mes chers collègues, Henri Bergson estimé que tout problème bien posée était déjà à moitié résolu en la matière, nous avons fait 50 pourcent du chemin en en discutant et en le courage de parcourir les 50 derniers en votant ce projet de loi, je vous remercie.

Madame la présidente, madame la ministre, monsieur le rapporteur, mais mes chers collègues. Un certain nombre d'orateurs avant moi ont bien voulu citer le modeste rapport que j'ai été amené à présenter à la commission des finances et qui a été publiée fin juin, juste avant que nos collègues Herriot ne dépose cette proposition de loi, j'ai fait l'effort tout à l'heure de reprendre la recommandation que j'allais mourir formulée, qui était la suivante. Appliquer la loi Diard au contrôleur aérien en l'adaptant aux caractéristiques du service minimum auquel ils sont déjà Astra. C'est-à-dire de voler à appliquer la loi Diard, deuxièmement l'adapter aux caractéristiques du service minimum auquel ils sont déjà astreint, ce rapport a fait du bruit par rapport au nombre de jours de grève que j'ai été amené à citer, il a également fait du bruit par rapport à une exigence que j'ai rappelées, c'est-à-dire celle de donner à la France est une grande nation aéronautique au monde la plus belle pour moi et pour nous, sans doute la 2ème sans doute aujourd'hui mais lui donner la capacité de faire voler les avions dans les meilleures conditions pour les passagers pour les compagnies d'éviter les retards et j'surtout, surtout, de faire passer le trafic qui va croissant, à peu près 4,8 pourcent d'augmentation cette année et peut-être entre 2 et demi et 5 l'année prochaine et donc le contrôle aérien est essentielle : il y a les compagnies et les installations au sol, il s'agit de gérer le survol de gérer la circulation des avions en l'air, et c'est là le rôle majeur de nos contrôleurs aériens qui sont reconnus mondialement et l'École nationale avait son civil a un rôle pilote dans le monde entier et nouent des partenariats de par Son Excellence, et nous avons d'excellents contrôleur aérien et nous avons un service public dont on peut s'enorgueillir s'enorgueillir c'est aussi regarder ses failles, ses difficultés j'en ai cité plusieurs dans ce rapport, qui avait une volonté constructive, c'est-à-dire de poser un certain de sujets. J'ai indiqué qu'il fallait réfléchir sur le nombre de contrôleurs aériens et j'ai d'abord indiqué qu'il fallait aujourd'hui desserrer la contrainte parce que le trafic augmentant, nous avons besoin de plus de contrôleurs aériens, j'ai indiqué qu'il fallait maintenant se mettre en situation aussi de moderniser les logiciels et matériels pour faire passer le trafic et puis enfin, j'ai appelé au dialogue social à plus de mobilité à plus d'agilité dans l'organisation, il son travail pour s'adapter au trafic et à ce titre-là, j'ai pointé la question des jours de grève, et là-dessus, j'ai effectivement fait cette recommandation, c'est-à-dire de permettre que, on se donne les moyens, avec des contrôleurs aériens et pour moi, ça passe par du dialogue social de mener cette modernisation qui est à dire d'ajouter à un service minimum qui existe à des réquisitions qui existent, qui seront encore prises pour ce vendredi, parce qu'il y a un mouvement d'ajouter l'obligation de ces dégâts grévistes à la j'insiste juste sur ce point parce que c'est quand même une singularité, c'est-à-dire que, il nous faut conjuguer un service minimum qui existe, à la différence de la RATP, la SNCF etc et cette obligation de se déclarer gréviste de conjuguer les 2 systèmes d'où quand même un minimum de dialogue qu'il faut avoir, je crois, et un certain nombre de questions juridiques qui peuvent se poser, je veux simplement dire que ça a été dit par certains, le moment et pas forcément le meilleur, alors on m'objectera qu'c'est jamais le bon moment mais c'est vrai, on l'a rappelé il y a eu les élections professionnelles honnête à la fin de l'année quelques semaines des vacances et puis surtout, il y a le climat que chacun connaît dans le pays qui a été rappelé ici je veux surtout dire que mon rapport était un tout et que c'est dans cet ensemble-là, je pense qu'on doit progresser, c'est-à-dire modernisation des logiciels et matériels, dialogue social et puis cette affaire du droit de grève, avec une augmentation, je pense qu'il faut gérer du nombre de contrôleurs qui me paraît être aujourd'hui une nécessité. Ce que je veux simplement dire c'est que on est confronté à cette réalité, déficit du nombre du nombre de contrôleurs des physique techniques et puis besoin d'agilité social et que tout ça doit être menée en parallèle, la DSN a il a besoin de se projeter dans un avenir partager avec l'ensemble des contrôleurs je voudrais livrer 2 2 interrogations disons que la position de mon groupe est est une position favorable, c'est une mesure que j'avais moi-même proposé. Je ne suis pas certain qu'il y a aujourd'hui l'accompagnement social et le temps dialogue nécessaire encore et je ne suis pas certain que le dispositif soit encore totalement au point mais ça va dans le bon sens, je veux dire que de manière générale et en particulier dans le secteur, je crois au dialogue social, il me semble que c'est ensemble que les personnels de la DSN a avec les équipes de la direction générale de la direction réussiront à franchir ce palier qui celui l'augmentation du trafic. Attention aux clichés, moi j'ai compté à peu près 20 pourcent des retards qui sont dus aux grèves, c'est beaucoup. Mais ce sont 20 pourcent et ensuite il faut se rappeler que le droit de grève est un droit constitutionnel, évidemment qu'il faut garantir, d'où la difficulté, on travaille dans le social, on travaille dans un domaine conflictuelle il faut gérer à ce dialogue social et il faut essayer de prévenir la conflictualité, c'est aussi notre devoir, la ministre a rappelé tout à l'heure, mais je veux dire aussi que, il y a un certain nombre de questions qu'il faut approfondir quand même me semble-t-il, comment concilier le service minimum qui existe déjà et cette obligation nouvelle qui est nécessaire, ça me semble un point difficile, je ne souhaite pas que l'obligation s'est déclaré gréviste viennent affaiblir le système des réquisitions, c'est tout de même une interrogation, ça a été rappelé, sur la gauche, tout à l'heure, qu'on n'assure la solidité de l'édifice juridique et ça me paraît être un élément majeur. Ce que je veux enfin dire, c'est que nous avons une spécificité en Europe si nous aboutissons à ce résultat-là parce que aucun des services de navigation aérienne en Europe n'a réussi aujourd'hui à concilier ces 2 systèmes et ça mérite me semble-t-il, quelques égards et quelque temps de concertation qui n'ont pas forcément eu lieu jusque-là voilà donc je voudrais simplement résumé ma position en quelques mots et celle de mon groupe qui est favorable, mais dire que nous aurions souhaité qu'il y ait plus de concertation avec les organisations professionnelles et syndicales que on approfondisse les questions juridiques qui sont liés à la juxtaposition de 2 systèmes qui sont tout de même complexe et que, s'agissant de droit social et s'agissant d'un service majeur pour la France, qui est un grand pays, aéronautique, il va falloir maintenant créer les conditions pour que chacun des acteurs se réunissent aille de l'avant se mobilisent autour d'un projet industriel et d'un projet aéronautique majeur qui est attendu par les compagnies et je souhaite que ce calendrier qui me paraît un peu resserré ne nuisent pas à l'objectif que nous pouvons poursuivre ensemble, qui est de faire que, à l'arrivée, nous ayons progressé éviter la conflictualité qui peut être enregistrée trop souvent mais surtout permis d'avoir un système pérenne et qui fasse que les voyageurs qui sont au centre de l'objectif est au centre du dispositif se retrouve avec un service public amélioré, je vous remercie. Merci, la parole est à monsieur Max mourir. Monsieur le président,

dames, la ministre, monsieur le rapporteur, monsieur le président de la commission, mais certes, mes chers collègues, je n'ai pas la connaissance pointue du sujet de Vincent Capo Capo Canellas ceux qui viennent de s'exprimer ni le talent de Pierre Soulages pour peindre tableau à noir mais je voudrais rappeler ce que signifie concrètement le sujet dont nous avons à traiter ce soir courriel à 23 heures informant de perturbations possibles pour un avion aux aurores et vous invitant à repousser votre voyage lignes téléphoniques pour les passagers, saturé, bien sûr, où après des minutes cadencé par les 4 saisons de Vivaldi et vous ai répondu que la compagnie de dispose pas d'informations concernant votre vol, arrivé au petit matin, angoissé, dans un arrêt ports bondés attente jusqu'à plusieurs heures dans des salles de l'aéroport ou pour les moins chanceux, ce qui fut mon cas, le 22 mai dans un avion cloué au sol, donc vous ne pouvez pas sortir et pendant ce temps, on est allé chercher un contrôleur aérien quelque part à l'autre bout du département enfin, remboursement des billets perdus rarement à la hauteur du cou engagé voilà, mes chers collègues, les conséquences de l'exercice du droit de grève des contrôleurs aériens pour nos concitoyens dans les dispositions actuelles

qui proviennent de fonctionnaires français ce constat et les grèves qui ont 4 ans c'est le printemps dernier, comme chaque année, nous appeler mais, chers collègues, agir, je soutiens donc pleinement la proposition de loi déposée par notre collègue Joël guerrier j'ai d'ailleurs déposé avec ma collègue Christine Boos Bonson Tido une proposition de loi dont les dispositions sont tout à fait semblable, nos objectifs sont clairs obliger les contrôles aériens a déclaré individuellement leur rétention de participer à la grève ajuster l'organisation des services de transport et rieur, conserver le blé, l'exercice de leur droit de grève, éviter de prendre un otage des passagers et d'intensifier des situations de crise qui pourraient être évités avec un peu de bonne volonté à ceux qui tenteront de faire croire que ces formalités pour ta tête à l'exercice du droit de grève, je répondrai que le nombre de jours de grève dans les transports n'a sans doute pas baissé depuis que la loi diable s'avisent minimum sont entrées en vigueur et, par ailleurs, on ne peut comprendre que seuls les fonctionnaires qui, je le rappelle, sont des agents du service public, et j'insiste sur le mot service soit le maillot qui perturbe cette chaîne tous les autres métiers de la chaîne de préparation du vol ont une obligation de déclaration qui permet aux établissements et entreprises qui les emploient d'appréhender l'ampleur de la grève, et donc de déployer les mesures nécessaires au respect du service minimum et que les contrôleurs aériens dans ce cadre et d'autant plus important que, comme l'a rappelé Alain Fouché, le rapporteur, une journée de grève coûte à la DGAC, entre 3 et 4 millions d'euros, je souhaiterais simplement insister sur le fait qu'il ne s'agit que Testore une obligation d'information, de participation et de grève, une simple obligation d'information, mes chers collègues, mais elle permettra de lutter contre le manque de prévisibilité et de contenir des perturbations dommageable humainement et financièrement alors, mes chers collègues, bien entendu, restauration d'une obligation de déclaration de participation à une grève des contrôleurs arrière aurait pu s'inscrire dans ce texte plus large incluant aussi d'autres services publics comme les services postaux auquel je sais que ma collègue Christine Avart des particulièrement attachés, bien entendu, je comprends les doutes concernant l'opportunité de l'examen de ce texte en période d'élections syndicales qui vient de s'achever, j'ai moi-même est alerté pas c'était syndicat sur le risque de fragilisation des plus réformiste d'entre eux, j'entends ce risque très relatif, mais puisque l'occasion nous étonner de prendre des décisions qui vont dans le bon sens, mes chers collègues, il faut agir, Madame le Ministre, vous nous appelez au sens des responsabilités, responsabilités, responsabilités et puisque nous avons le sens des responsabilités, nous allons achever un travail inachevé, la flamme réformatrice de notre pays, ce serait-elle éteinte sur les ronds-points, nous ne le souhaitons pas le pire risque : celui de ne pas prendre de risques, c'est ce qu'indiquait Nicolas Sarkozy lorsqu'il est institué, le service minimum, voilà pourquoi je vote dorée comme des collègues du groupe, les républicains, cette proposition de loi sectorielles, certes, mais utile pour nos concitoyens.

Madame la présidente, madame la ministre, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, je voudrais d'abord saluer le travail remarquable effectué par nos collègues, Joël Gariod et Alain Fouché, respectivement auteur et rapporteur de la proposition de loi que nous examinons aujourd'hui. Au mois de juillet dernier, 4 compagnies aériennes ont déposé plainte auprès de l'Union européenne contre la France pour violation du respect du principe de liberté de mouvement à l'intérieur de l'Union, il n'y a pas que sur nos ronds-points que la liberté de mouvement pose problème sur la période 2004 2016, la France a enregistré 250 jours de grève de ses contrôleurs aériens, le second pays européens sur le podium en la matière et la Grèce, loin de nous égaler elle n'enregistre que 46 jours de grève sur la même période, d'ailleurs semble s'aggraver ces dernières années, les grèves des contrôleurs aériens ont été 4 fois plus nombreux cette année par rapport à 2017 perturbant, plus de 6000 vols 16000 vols depuis le début de l'année et pénalisant, plus de 750000 voyageurs. Ces grèves à répétition retenti sur notre économie et pénalise nos partenaires étrangers, selon un récent rapport de la commission des finances, la France est ainsi responsable de 33 pourcent à elle seule Des retards dus au contrôle aérien en Europe, l'absence de préavis de grève effectifs empêche la bonne information des passagers français et étrangers sur l'état de leurs vols, bien souvent, ils apprennent leur annulation à la dernière minute aussi la révision des statuts de grève des contrôleurs aériens pour améliorer l'information des voyageurs des compagnies et des institutions apparaît telle comme une nécessité, la proposition de loi que nous fait Joël au vise à étendre les obligations de déclaration de grève applicable aux salariés des entreprises de transport terrestre au transport aérien les contrôleurs aériens et une partie du personnel des services de la navigation aérienne devront déclarer leur intention de participer à un mouvement de grève au moins 48 heures à l'avance et informer leur employeur en cas de renoncement à la grève au moins 24 heures avant. Ces nouvelles grèves permettront aux personnels de navigation dès leur entrée en vigueur d'anticiper les contraintes organisationnelles et de réduire autant que faire se peut les retards et annulations de vols, bien entendu, en aucun cas d'une atteinte au droit de grève des contrôleurs aériens, nous mesurons leurs contraintes dans un contexte de hausse du trafic et de baisse des ressources pour autant, il est vital pour nos économies, comme pour celle de nos voisins, de préserver la régularité, l'efficacité et la bonne gestion des liaisons aériennes. J'ai entendu une de nos collègues, déclarait que cette proposition de loi constitue une atteinte au droit de grève constitutionnellement reconnu. Je crois que nous devrons faire auprès d'elle amende honorable, il est certain que le sénat français n'a pas la fibre humaniste, la sophistication technique non plus qui lui permettrait de parvenir à appliquer un droit de grève aussi généreux, aussi favorables aux salariés que dans les pays de cocagne dirigée par ses amis Maduro Castro Guillaume Ping qui partagent son idéologie. et dont chacun connaît le respect, j'aurais pu citer si j'avais fait un peu d'histoire, la sophistication encore plus grande à laquelle était parvenu la défunte URSS que vous avez toujours soutenu oui donc un niveau l'URSS et que vous avez toujours soutenu jusqu'à son décès prématurés qui vous à désespérer. Ces pays par conséquent dans chacun connaît le respect absolu des droits de l'homme qui les caractérise et qui serait sans nul doute, mises en oeuvre en France, si son parti arrivait au pouvoir, pour le plus grand bonheur, bien entendu, de nos concitoyens, mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa pour répondre aux difficultés du secteur : les assises du transport aérien, organisé par le ministère des Transports en mars dernier, devraient rendre leurs conclusions d'ici peu, nous sommes demandeurs d'une véritable stratégie nationale en matière de transport aérien, ce secteur représente 25 milliards d'euros de chiffre d'affaires et 100000 emplois il connaît de vraies difficultés, pris en tenaille entre des charges importantes, une concurrence effrénée exercée par les compagnies du Golfe, le low-cost et nos voisins européens, dont les charges sociales sont moins onéreuses que celles supportées par les compagnies françaises à titre d'exemple, pour Air France, l'écart des charges représenterait entre 400 à 700 millions d'euros, selon les pays. à l'échelle nationale, les liaisons aériennes contribue au désenclavement des territoires, nous saluons à ce titre, la volonté du gouvernement de soutenir le développement des lignes d'aménagement du territoire, avec un montant de 15 millions d'euros supplémentaires, soit 4 fois le montant consacré à ces liaisons en 2018, nous saluons également l'initiative de notre collègue Vincent Capo, hélas, qui, après avoir publié un rapport remarqué auquel vous avez fait allusion tout à l'heure, Madame la Ministre a conduit à l'adoption au Sénat dans le cadre du PLF pour 2019 une disposition visant à alléger le poids des taxes aéronautiques sur les billets des vols intérieurs, chers collègues, je vous l'annonce sans surprise le que le groupe, les indépendants républiques et territoires votera cette proposition de loi je vous remets. Merci, la parole est à madame Catherine Procaccia pour 100 minutes.

Madame la présidente, madame la ministre, monsieur le président, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, merci à Joël du Rio pour le dépôt et l'inscription de cette PPL et a d'excellents rapports d'Alain Fouché, qui dit tout, il me permettra, je l'espère, d'obtenir ce soir une réponse à la question écrite 6485 que j'ai déposé le 2 août Madame la ministre, qui est pour l'instant restées lettre morte et et en même temps de rappeler ici les précédents débats dans cet hémicycle, madame, je vous interroger sur les intentions du gouvernement pour limiter l'impact des grèves des contrôleurs aériens français qui restreignent non seulement la liberté de mouvement des Français mais aussi celles des compagnies aériennes, ma collègue a rappelé que 4 compagnies européennes AIG Ryanair, EasyJet et Wiz Air ont déposé une plainte contre la France auprès de l'Union européenne 16000 vols auraient été perturbées au 1er trimestre impactant en plus de 2 millions de voyageurs: ces compagnies ne conteste pas le droit de grève des contrôleurs aériens, mais le fait que le survol de l'Hexagone leur soit dans ce cas, interdit la France pourrait être condamné au nom de la libre circulation, comme elle l'a déjà été en 1997 lorsque l'Espagne nous avaient attaqués pour obstruction de ses exportations de fruits et de légumes, faut-il attendre une condamnation pour qu'enfin le gouvernement impose une déclaration préalable de grève de 48 heures qui amélioreraient sans aucun doute la situation des voyageurs et des compagnies, les orateurs qui m'ont précédé, ont rappelé que le droit de grève des contrôleurs aériens date de 1984 85 que dans les faits, il autorise la réquisition des fonctionnaires d'État que sont nos contrôleurs afin que la totalité des survols et au moins 50 pourcent des arrivées et des départs soit assurée, la réalité, nous l'avons tous dit est tout autre et les grèves se superpose celle des aiguilleurs du ciel, en tant que telle, mais aussi en tant que fonctionnaire auquel se surajoute des grèves locales sur certains sites, j'ai même le sentiment que la situation s'est dégradée ces dernières années en 2007 j'étais rapporteur de la loi qui est communément appelé service minimum pour les transports terrestres à laquelle plusieurs d'entre vous ont fait référence et c'est à ce titre que je veux intervenir cette loi voulue par Nicolas Sarkozy n'est en réalité qu'une loi de dialogue social visant à prévenir les conflits et ils surviennent de permettent la mise en place d'un service minimum garanti grâce à une connaissance plus fine des personnels présents des grévistes devant eux se déclarer 48 heures à l'avance et surtout elle impose une concertation préalable avant la grève, cette loi a clairement améliorer la situation, les transporteurs terrestres peuvent organiser le trafic et les usagers sont mieux informés, sans pour autant que les grèves, comme l'ont dit certains se soit réduite, c'est pour ça d'en juin 2009 j'ai déposé une proposition de loi visant à à étendre ses dispositions au transport aérien et maritime, elle fut signée par une cinquantaine de collègues dont Alain Fouché, ici présent, qu'il ne se souvient peut-être même pas à l'époque, lors des auditions la DGAC m'avait assuré que l'extension contrôleurs aériens était inutile, les dispositions existantes suffisant amplement en janvier 2010 lors d'un débat organisé à mon elle initiative sur l'extension du service minimum à l'aérien le ministre des Transports de l'époque me répondaient je cite les grévistes ne sont pas obligés de se déclarer à l'avance, ce qui conduit souvent à annuler plus de vols que nécessaire, comme vous l'avez dit, Madame la Ministre, messieurs les rapporteurs, monsieur le président, il ajoutait, peut-être faudrait-il modifier en ce sens de la loi de 1984 mais lui ne l'a pas fait et inutile de compter sur ses successeurs socialistes, il suffit d'ailleurs d'écouter mes collègues présents ce soir et en 2012 quand la loi Diard a été votée, elle ne concernait pas non plus les aiguilleurs du ciel, aujourd'hui, je l'espère, nous allons voter cette PPL que je soutiens, même si pour moi il manque un élément essentiel, le volet prévention des conflits, avant le déclenchement de la grève, c'est d'ailleurs un peu ce que vous proposez, madame la ministre avec la concertation, je ne peux oublier les débats un peu surréaliste tenus dans cet hémicycle, sur le droit de grève dans le secteur aérien, mais nous en avons eu ce soir un bref raccourci, je ne doute pas, Madame le Ministre, que vous êtes conscient de la nécessité de faire quelque chose, même si vous n'êtes pas autoriser ce soir, a donné un avis favorable à cette PPL il faut que le texte soit aussi voté par l'Assemblée nationale et sans doute amendé, comme le veut aussi notre collègue Vincent Capo Canellas car que ce va-t-il se passer si la France est condamnée, comme je l'évoquais en introduction, mieux vaut-il pas se concerter élaboré un texte qui pourrait être accepté par les contrôleurs aériens que de prendre des mesures, contraint et forcé, au dernier moment qui provoqueront des grèves sans doute encore plus dur, cette loi ne mettra pas fin aux grèves, mais elle permettra de mieux organiser un service essentiel pour la France et pour l'Europe. Au MoDem Lavardin, il y avait encore une oratrice mais que déjà mais, oui Christine Lavardin pour 4 minutes je vous en prie. Merci madame la présidente, Madame le Ministre, ça aurait été dommage puisque nous allons retourner sur Terre, je suis désolé mais 261 jours, soit 8 mois et 17 jours 261 jours que des facteurs se sont mis en grève dans les Hauts-de-Seine, du jour au lendemain, sur le fondement d'un préavis qui courait depuis 2015, plus de 2 mois avant que le ministère de l'Économie et des Finances, qui assure la tutelle de l'établissement La Poste prenne connaissance du problème grâce au courrier parlementaire, en effet, les indicateurs de performance mensuelle établie à la maille départemental ne reflétait pas la forte dégradation de la qualité du service public à la maille locale près de 3 mois sans aucun courrier dans certains quartiers lettres des communes de Boulogne-Billancourt, Neuilly-sur-Seine, Levallois-One hier au plus fort du mouvement, près de 800000 plis en souffrance stockés en attente d'un tri d'une distribution et en conséquence des prix daté du mois d'avril, qui ne sont arrivés à destination que début septembre, combien de petites entreprises d'artisans, de commerçants, de professions libérales qui ont perdu des clients démarchés à cause de cette défaillance du service public, combien de patients qui n'ont pas reçu à temps les résultats de leur analyse médicale ou leur convocation à l'hôpital, combien de futurs acheteurs qui ont connu d'immenses difficultés à conclure leur offre de près combien d'automobilistes qui reçoivent désormais des amendes majorées pour un soi-disant refus de paiement dans une société de plus en plus immatériels nombres de documents officiels continuent cependant à être échangé entre particuliers, entreprises, associations ou administration sous forme matérielle par la voie postale, les exemples sont nombreux, cartes bancaires, codes de cartes bancaires qu'Ahmed Cheikh facture extrait date de naissance, résultat médical, avis d'imposition amendes de police et la liste encore plus longue, la réception de ces documents avec retard peut avoir des conséquences pénalisantes majoration d'amende radiation de la Sécurité sociale impossible dans toutes ces situations de se tourner vers une solution alternative, en effet, force est de constater que, malgré l'ouverture de la totalité du marché du courrier à la concurrence depuis le 1er janvier 2011, aucun acteur n'est venu concurrencer La Poste sur le marché des plis de moins de 50 grammes, le service postal universel défini à l'article L-1 du Code des postes et des communications électroniques précise qu'au titre de service public, le service universel postal est assurée dans le respect des principes d'égalité de continuité et d'acceptabilité et d'adaptabilité pardon en recherchant la meilleure efficacité économique et sociale, compte tenu des mouvements sociaux survenus ces derniers mois et pas que dans les Hauts-de-Seine en plusieurs points du territoire, la juste conciliation du droit de grève et de la continuité du service public postal n'a jamais semblé aussi indispensable, c'est l'objet de la proposition de loi qui a été cosigné par plus de 80 d'entre nous, la réglementation du droit de grève des agents publics en droit français, manque d'unité, cela a été dit et le bénéficiaire du service public, à savoir l'usager se trouve confronté à des textes divers et variés, selon l'expression du préfet du professeur Pierre Delvaux et qui ajoute dans son commentaire du célèbre Darren du 7 juillet 1950 l'ampleur et le succès des mouvements de grève dépend essentiellement des conditions de fait et des rapports de force et échappent dans une large mesure à l'emprise des limitations juridiques ces limitations juridiques qui vont de l'obligation de déposer un préavis à l'interdiction d'une grève tournante, en passant par la réquisition manque singulièrement d'unité ainsi, selon le service public concerné, il y aura une obligation de préavis ou une obligation de service minimum le délai de ce préavis ne sera pas le même selon le service public de 48 heures dans l'Éducation nationale à 5 jours pour un agent territorial pourquoi dans le nouveau monde, madame le ministre, ne pourrait-on pas unifier l'ensemble de ces limitations dans un souci de simplification, pourquoi ne pas légiférer au lieu d'attendre du gouvernement des juges, des décisions jurisprudentielles variable selon les magistrats, selon le temps, selon les partis pourquoi surtout ne pas unifiée et étendre les règles du service minimum, la proposition de loi de ce soir du groupe, les indépendants républiques et territoires nous invite au débat. Merci madame Masséna. Madame la ministre souhaite y apporter des réponses aux différents orateurs, je vous en prie. Merci madame la présidente, alors je voudrais tout d'abord pour assurer Madame la sénatrice, il n'y a aucun risque que la France soit condamné, dans le cas de la plainte qui a été déposé par 4 compagnies aériennes qui ont peut-être aussi un certain nombre de sujets, faire part d'années pardonnez vu des passagers, de la France a toujours été assuré, il n'y a aucune règle internationale qui indiquerait que ce survol doit être assurée sans aucun délai, donc aucun risque de condamnation de la France est un peu de la communication de la part des compagnies aériennes en question je voudrais redire ça a été dit par certains orateurs mais le redire, ayons en tête que oui, il y a des perturbations dans le transport aérien, mais ne sous-estimons pas l'impact des événements météorologiques, d'autant qu'ils sont appelés sans doute à se développer. Et donc, il faut aussi se préparer à gérer ce genre d'événements météorologiques. Qu'il y a eu des sous-investissement. Qu'il y a un problème d'effectif dans le contrôle aérien. Et par ailleurs il y a aussi. Des problèmes d'organisation d'un certain nombre de compagnies aériennes qui conçoivent leur rotation de façon trop juste le moindre grain de sable par exemple météo conduisant à des effets boule de neige qui perturbe et qui pénalise de nombreux passagers alors oui en effet il y a aussi la question des grèves, je pense que les chiffres sont maintenant largement partagé, mais je voudrais rappeler qu'il existe. Un service minimum. Dans. Les services du contrôle aérien et je pense que c'est un petit peu unique, ne l'oublions pas, avec effectivement la possibilité d'astreinte pour les agents concernés, il existe par ailleurs un préavis comme il en existe pour tous les agents de la fonction publique, il est sans doute utile de réfléchir à des dispositifs de prévention des conflits qui pour le coup, existe dans d'autres secteurs, mais pas dans le transport aérien, il est sans doute utile de réfléchir à des dispositifs permettant de mieux anticiper des conséquences d'une grève par exemple avec des déclarations préalables des agents concernés, on voit que c'est une architecture qu'il s'agit de bâtir et moi je vous redis ma conviction que ce type d'architecture que ce genre de dispositif seront d'autant plus efficace et d'autant mieux acceptée qu'ils auront été précédée par une concertation, je vous remercie. la discussion générale est Close, mes chers collègues, je vous propose que nous passions à l'examen du texte de la Commission, il y a 4 amendements qui ont été déposées, cela nous permettra de terminer ce texte avant de lever la séance, si tout le monde en est d'accord, hé bien nous poursuivons

à ajouter une contrainte qui est l'obligation de se déclarer gréviste et donc il me semble qu'il est logique, en parallèle, on veille à la prévention des conflits des conflits sociaux pour éviter le nombre de grèves et qu'on essaye de favoriser le dialogue social, ça me paraît être une forme d'équilibre qu'il nous faut rechercher donc le présent amendement vise à introduire une procédure obligatoire de prévision des conflits sociaux, avec un délai de 15 jours, qui permet de se donner le temps de vérifier y a une bonne raison de faire grève et de permettre aussi à la direction peut-être d'apporter des éclaircissements et de nouer un dialogue dans des formes qu'il faudra définir par décret, il s'agit de réduire la conflictualité sociale, cette procédure de prévention des conflits sociaux sociaux sur bien évidemment au dispositif de réquisition et à l'application de ce texte instaurant l'obligation de se déclarer gréviste voilà donc c'est une procédure qui qui sera complémentaire de ce que la DGAC fait déjà, à savoir les protocoles sociaux trier, donc ils sont signés avec les organisations syndicales et qui vise à améliorer la performance globale du système, voilà ce que je propose. Merci, quel est l'avis de la Commission, monsieur le rapporteur.

et cet amendement est est le suivant, puis il y a 2 qui se suivent et vise en définitive comme je le dis à réécrire la proposition de loi afin de revoir les conditions d'exercice du droit de grève des contrôleurs aériens. Ces amendements proposent d'une part, d'adapter le dispositif du service minimum afin de faire en sorte que les réquisitions de personnel depuis au maximum que 50 pourcent de l'effectif opérationnel prévue le jour de la grève, il était question avant de de

le un modifie la loi, donc c'est un habit de défavorable qui les 2 sont liés. C'est un avis favorable, l'épave favorable, défavorable, très bien, Madame la Ministre, quel est l'avis du gouvernement. Merci madame la présidente, donc, cet amendement vise précisément à mettre en place un dispositif de prévention des conflits. Auquel je ne peux qu'être favorable comme je l'évoquais en l'état, votre proposition modifie très significativement la façon dont doit se dérouler la négociation préalable à la grève pour les conseils personnels concernés de la navigation aérienne, vous prévoyez l'instauration d'un délai de 15 jours qui viendrait s'ajouter au délai de droit commun de 5 jours pour les préavis de grève tous ceux-ci modifient très fondamentalement fondamentalement les conditions d'exercice du croate du droit de grève dans le secteur et donc moi je pense que ça doit réellement faire l'objet d'une concertation à la fois sur chacun des dispositifs et sur le cumul de l'ensemble de ces dispositifs donc je vous propose le retrait de cet amendement et sinon avis défavorable.

on veille quand même, a demandé que, avant, on se donne les moyens du dialogue et la concertation avant d'aller à la grève semble semble minimum assailli, monsieur le rapporteur je suis confus parce qu'on m'avait répondu sur l'amendement que je n'ai pas présenté l'amendement suivant, effectivement, il apporte une modification substantielle et là je suis d'accord, je veux bien qu'on dise que j'aurais écrit le texte là j'ajoute juste un dispositif de prévention des conflits, c'est tout, c'est pas réécrire le texte et apporter un élément complémentaire qui me semble aller dans le sens qui est recherché, c'est-à-dire de diminuer la confiture été diminué avant de grève. madame Procap certes, je vous en prie pour explication de vote. Je crois avoir dit qu'effectivement ce qui manquait dans la PPL c'était ce mécanisme de prévention des conflits, qui impose un dialogue alors je rappelle à mon collègue rapporteur que dans la proposition de loi qu'il m'avait cosigné ce mécanisme de prévention des conflits existait et ce dialogue existait et il paraît nécessaire, alors qu'un jour je ne sais pas si c'est le bon délai mais je crois que ça fait partie des éléments qui sont importants, si on ne veut pas avoir de réaction particulière et à avoir la le sentiment d'imposer immédiatement un droit de grève, la de remettre en cause le droit de venir là, on veut d'abord prévenir les conflits en dialoguant et après mettre en place le système de préavis pour ma part, à titre personnel, je voterai l'amendement de mon collègue Vincent. Y a-t-il d'autres d'explications de vote. Je n'en vois pas je vais mettre aux voix l'amendement de rectifier avec 2 avis défavorables qui est pour son adoption.

Qui est contre. S'il est adopté. L'amendement de rectifier, être adopté, je vais mettre aux voix l'article unique qui est pour son adoption. Qui est contre. Il est adopté, après l'article unique, un amendement a rectifier bis monsieur capot hélas. Merci madame la présidente, alors là je conviens, monsieur le rapporteur aisément que celui-ci est plus substantielles puisque, on a expliqué tout à l'heure, on vient combiner le service minimum qui existe, c'est-à-dire les réquisitions qui peuvent être pratiquées par l'ADSL a qui ne s'en privent pas et on la comprend et qui peuvent être appliquées sur un taux important au-dessus de 50 pourcent du nombre de contrôleurs peuvent être réquisitionnés, voire bien plus encore aujourd'hui déjà et donc, il s'agit d'elle, a ajouté le dispositif qui concerne, elle, l'obligation de se déclarer gréviste à ce système de réquisition et je propose ici de limiter le pourcentage de réquisitions à 50 pourcent c'est-à-dire de nous dire : on aura

de faire des réquisitions et il me semble que combiner les 2 c'est-à-dire l'obligation de se déclarer grévistes et des réquisitions avec un taux de réquisition au-dessus de 50 pourcent ça pourrait être excessif, droit, je propose de faire un mouvement de ce côté-là et de limiter les réquisitions à 50 pourcent du personnel, ce qui est déjà un service minimum conséquents. Quel est l'avis de la Commission, monsieur le rapporteur. rédige complètement l'article 1 du punitive écrase de texte et supprime l'obligation de déclaration préalable et.

Quel est l'avis du gouvernement, Madame la Ministre. en fonction, le jour de la grève, la loi de 84, je voudrais le rappeler fixe une obligation de résultat sur la continuité d'un certain nombre de services, assurer la fixation d'un plafonnement des astreintes et contradictoire avec l'obligation de garantir l'exécution du service minimum en toutes circonstances, selon les termes mêmes de la loi s'il était retenu le plafond que vous proposez, pourrait conduire dans certains cas à une diminution du niveau de service minimum qui aurait des impacts en particulier sur la desserte de certains aéroports métropolitains ce plafonnement ne manquerait pas d'avoir des incidences sur le traitement d'un certain nombre d'événements ponctuels, je pense au festival de Cannes au Grand Prix de Monaco, qui expose certains aéroports à des très fortes variations d'activité circonstances circonstances il peut s'avérer nécessaire de disposer d'une capacité plus élevée, nécessitant d'astreindre des personnels supplémentaires, ces situations ont fait l'objet à plusieurs reprises de jugements des tribunaux administratifs qui en ont validé le bien-fondé la limitation, vous proposez ne permettrait pas au service du contrôle aérien, d'y faire face, avec les conséquences économiques, médiatiques, mais y compris en terme d'ordre public que l'on peut imaginer et, par ailleurs elle oblige, exposerait la France à ne pas pouvoir respecter ces zones dégagement internationaux donc pour toutes ces raisons, je vous propose le retrait de votre amendement sinon je mettrais un avis défavorable. Monsieur cap au

je dirais que l'argument du 7 Festival de Cannes me paraît pas le plus performant, même s'il existe, il faut veiller à ces grands événements médiatiques, bien évidemment, c'est pas l'ancien maire du Bourget qui vous dira le contraire, pour d'autres, d'autres événements, voilà, donc je veux bien le le retirer, je voulais simplement souligner que la combinaison des 2 systèmes a induit quand même une petite fragilité. Oui, je l'très vite, j'en ai parlé lors de la discussion générale, il s'agit de demander que tous les ans le Parlement puisse disposer et que les contrôleurs puissent voir par écrit l'état d'avancement de la modernisation de leur outil de travail, ça me paraît utile lorsqu'on leur fixe de nouvelles contraintes qu'en fait on s'intéresse au sujet principal aussi, qui est que nous n'avons pas assez modernisées, aujourd'hui, nous aurons bientôt dépenser 2 milliards pour un système qui aujourd'hui n'est pas encore en situation de performance, hein, et nous avons un vrai sujet pour passer la capacité pour augmenter la capacité de traitement des vols et que la France a une difficulté que j'ai souligné dans mon rapport, je ne l'ai pas fait de manière polémique, je ne l'ai pas fait dans la volonté de stigmatiser qui que ce soit et j'ai souligné un certain nombre de fragilités auxquelles nous devons réfléchir, c'est-à-dire que, si j'ose dire, à ce prix-là, il faudrait quand même qu'on y voie clair maintenant sur à quel rythme on arrivera à se doter de matériel et de logiciels dans les autres pays ont pu bénéficier, jusque-là, je dirais beaucoup de respect pour ceux dont c'est le métier, et cette mission est particulièrement difficile, il y a aussi des enjeux industriels et je sais que la ministre et l'équipe de de l'ADSL et la DGAC sont conscients des enjeux, donc je propose qu'en parallèle de l'effort qu'on demande aux contrôleurs sur le droit de grève, on les dote et on se dote collectivement d'une visibilité sur la modernisation de ce service qui était malgré tout le sujet important, un sujet important de cas. Quel est l'avis de la Commission, monsieur le rapporteur. Madame la présidente, madame la Ministre, mais on cet amendement prévoit que le gouvernement présente chaque année au Parlement un rapport sur l'état d'avancement des programmes de modernisation des outils de contrôle de la navigation aérienne, ce rapport doit notamment présenter le délai de mise en oeuvre de ces outils de contrôle ainsi que leur père ferment opérationnel cette demande de rapport fait suite au constat alarmant dressé effectivement par notre collègue Vincent Pau, hélas, dans son rapport sur le contrôle aérien, publié en juillet dernier, qui montrent que l'obsolescence des instruments de navigation aérienne, les responsables de nombreux retards de vols et que les programmes de modernisation de ces instruments ont pris beaucoup de retard, représente un coût très important cette préoccupation nous a d'ailleurs été relayé par l'ensemble des syndicats, que j'ai auditionné nous partageons cette inquiétude et c'est pourquoi la Commission a émis un avis favorable à l'adoption de cet amendement, qui permettra au Parlement d'être régulièrement informés de l'avancement de ces programmes de de modernisation. Madame la ministre, quel est l'avis du gouvernement. Merci madame la présidente, Bailly effectivement mener à bien ces grands programmes de modernisation de nos outils de contrôle aérien est un impératif, moi je regrette le retard qui a été pris effectivement, y compris des contraintes budgétaires qui ont pu s'imposer à certaines époques, en tout cas je pense qu'il est indispensable de doter nos contrôleurs aériens des meilleurs outils et je pense qu'il est parfaitement légitime que le Parlement souhaite avoir

Qui est contre, hé bien il est adopté largement adopté. Enfin, un dernier amendement le 4 rectifier monsieur Merci pour la présidence, en 2 mots, il s'agissait de modifier le titre, c'est une question sémantique proposerez-vous, je veux bien l'entendre passer du titre qui était déclaration propositions de loi sur la déclaration d'un préavis de grève des contrôleurs aériens à une proposition de loi relative à la performance des services de la vie, pourquoi, parce que je pense que c'est un tout, c'est-à-dire que la performance bien sûr le dialogue social, c'est aussi à taux de traiter de sujets qu'on vient d'aborder, voilà je soumets à votre sagacité. Monsieur rapporteur, quel est l'avis de la commission. Madame la présidente, madame la mêlée, cet amendement vise à modifier l'intitulé de la proposition de loi afin que celle-ci soit nommé Proposition de loi relative à la performance des services de la navigation aérienne, il s'agit d'un amendement de conséquences par rapport aux amendements précédent qui tendent à réécrit en totalité la proposition de loi, compte tenu des positions de la commission, que la commission a exprimé sur ces amendements et de la volonté de maintenir le dispositif prévu par la proposition de loi d'obligation de déclaration préalable de participation une grève, la commission a émis un avis défavorable à l'adoption de cet amendement. Quel est l'avis du gouvernement, Madame la Ministre. pour in fine et rendre un meilleur service aux passagers, donc moi je suis favorable à cet amendement. S'il n'y a pas de demande d'explications de vote, je vais mettre aux voix cet amendement avec un avis défavorable de la commission et un avis favorable du gouvernement qui est pour son adoption.

Je vais mettre aux voix l'ensemble de la proposition de loi y y a-t-il des demandes d'explications de vote, je n'en vois pas Madame Procaccia pardon. elle sera très courte, donc je voudrais simplement que Madame bah la ministre puisse profiter du j'espère du vote de cette PPL pour avoir un véhicule qui puisse lui être nécessaire comme ça l'a été à d'autres occasions, ici au Sénat pour qu'éventuellement rapidement, dans quelques mois ou dans une année, vous ayez le véhicule nécessaire que vous pourrez faire évoluer et enfin arrivé à cette performance de service en intégrant un certain nombre d'éléments qui, pour l'instant ne sont pas encore dans la loi, et aussi en Molière en le système de déclaration du droit de grève. Y a-t-il d'autre demande d'explications de vote. Non, hé bien je vais mettre aux voix l'ensemble de la proposition de loi dont l'intitulé est ainsi rédigé : proposition de loi relative à la performance des services de la navigation aérienne, qui est pour son adoption. Qui est contre. Elle est adoptée CVS. Je vais suspendre la séance, elle sera reprise à 21 heures 50 pour le débat sur le débat emplois non pourvus en France quelles réponses, quelles actions la séance est suspendue.